La séance est ouverte, messieurs les ministres, mes chers collègues, le compte rendu analytique de la précédente séance a été. a pas d'observation, le procès verbal est adopté sous les réserves d'usage j'informe que des candidatures pour siéger au sein de la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées de la commission des affaires sociales, la commission des lois ont été publiés ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement, l'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi de finances rectificative adoptée par l'Assemblée nationale pour 2022.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, monsieur le Ministre. Mesdames et messieurs les sénateurs. Je suis très heureux de vous retrouver ici au Sénat pour l'examen du paquet, pouvoir d'achat sur son volet : projet de loi de finances rectificative. Nous avons franchi une première étape et je tiens à vous en remercier, avec l'adoption du projet de loi, pouvoir d'achat, je tiens à vous remercier pour la qualité des débats qui ont permis d'adopter un texte qui est attendu par tous nos compatriotes je souhaite évidemment que nous puissions avancer dans cette même atmosphère constructive hein lors de cette discussion du PLFR. Dans quel contexte est-ce que cette discussion se tient. D'abord, dans un contexte économique dans lequel l'économie française résiste. Nous venons d'avoir les chiffres de la croissance du 2ème trimestre plus 0,5 % pour le 2ème trimestre 2022, la France obtient avec ce chiffre, un des meilleurs résultats de la zone Euro et ce résultat de 0 5 pour 100 prouve que l'économie française résiste mieux que les autres économies européennes aux turbulences économiques actuelles, il confirme également que, comme l'avait annoncé le gouvernement, l'économie française atteint atteindra drap bien les 2 5 % de croissance en 2022, c'était l'objectif que nous nous étions fixés tous les Français pour tous nos compatriotes pour toutes les entreprises, c'est une victoire obtenue dans des temps difficiles. L'inflation continue danser contexte économique difficile de progresser. Et nous sommes bien comme je l'avais indiqué il y a quelques mois, au coeur du pic inflationniste, l'inflation reste à un niveau élevé et elle restera à un niveau élevé jusqu'à la fin de l'année 2022. En revanche, je confirme que nous continuons à anticiper une baisse de l'inflation dans le courant de l'année 2023 grâce à la réorganisation des chaînes de valeur à la diversification des approvisionnements en matières premières, auquel nous travaillons avec. Les Les autres mini-sous autorité de la Première ministre et du président de la République et grâce aux effets de la politique monétaire. Ce pic inflationniste, donc un cap difficile à passer, qui justifie toutes les mesures d'accompagnement qui vous sont proposés aujourd'hui quelles sont ces mesures sans rentrer dans le détail de chacune d'entre elles, je voudrais expliquer la philosophie et la teneur des mesures qui vous sont proposés aujourd'hui. Il y a d'abord tout un volet qui porte sur l'énergie. C'est légitime parce que la moitié de l'inflation au moins s'explique par la flambée des prix de l'énergie, l'électricité, le gaz ou les carburants, nous avons donc décidé de maintenir le bouclier énergie jusqu'à la fin de l'année 2022 avec le gel du prix du gaz et le plafonnement du prix de l'électricité à 4 % ces décisions qui ont été prises à l'Automne 2021, explique que la France est aujourd'hui le taux d'inflation le plus faible de la zone Euro, nous avons anticipé et nous avons pris des mesures massives qui nous ont permis de combattre avec efficacité l'augmentation des prix. Je rappelle également que nous allons évidemment continuer à nous battre au niveau européen pour dissocier définitivement le prix de l'électricité du prix du gaz ce système européen dans lequel le prix de l'électricité décarbonés est indexé sur le prix des énergies fossiles, c'est-à-dire sur le prix du gaz est un système inacceptable du point de vue écologique. Et complètement contre-productif d'un point de vue économique, il a également un coût social qui dort en insupportable, nous avons engagé cette bataille avec le président de la République depuis plusieurs mois, nous ne lâcherons jamais rien jusqu'à ce que le prix de l'électricité soit définitivement dissocié du prix du gaz. Toujours sur l'énergie, des propositions ont été faites à l'Assemblée nationale sur la question du fioul. 3 millions de nos compatriotes se chauffe au fioul. Il était donc légitime et je salue la sagesse des députés de prendre les mesures fortes sur le fioul et la compensation pour nos compatriotes de ce chauffage au fioul. Nous avons donc adopté une aide de 230 millions d'euros pour les ménages qui utilisent ce combustible pour se chauffer, je confirme que nous lèverons le gage sur ces 230 millions d'euros et que nos compatriotes auront bien 230 millions d'euros à se répartir pour amortir le choc de l'augmentation des prix du fioul. Je propose que les parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale souhaite associée à la définition du ciblage des ménages qui pourront bénéficier de cette aide supplémentaire, 3 millions de nos compatriotes une enveloppe très significative de 230 millions d'euros, faut-il la cibler sur quel ménage mais plutôt que de discuter uniquement entre membres du gouvernement, je propose que les parlementaires soient associés à ce choix politique, de la répartition de l'enveloppe des 230 millions d'euros en faveur de 3 millions de nos compatriotes. 3ème sujet toujours sur l'énergie, c'est le prix des carburants qui est probablement ce qu'il y a de plus visible et de plus sensible pour nos compatriotes aujourd'hui. L'Assemblée nationale a proposé de passer la ristourne sur les carburants à 30 centimes d'euros, en septembre au lieu de 18 centimes trente centimes en octobre 10 centimes en novembre et 10 centimes en descend, je sais que d'autres propositions toutes intéressantes et argumentée, ont été formulés par les sénatrices et les sénateurs je pense néanmoins qu'il est sage de s'en tenir à la solution retenue par l'Assemblée nationale qui a le mérite de couvrir tous nos compatriotes, y compris les retraités, y compris ceux qui ne travaillent pas, je suggère donc nous retenons cette proposition qui fait que, avec les remises accordées par certains pétroliers ou par certains distributeurs, nous pourrions avoir un prix du carburant à 1 à la rentrée de 2022 au lieu des prix que nous connaissons aujourd'hui, je pense que beaucoup de nos compatriotes attendent désormais très concrètement, d'aller à la pompe et d'avoir ce chiffre-là, je recommande donc que nous en tenions à cette solution pour tout ce qui me disent légitimement qu'il faut faire plus pour ceux qui travaillent, je rappelle que d'autres dispositifs seront mis en place, nous avons accepté, notamment à l'Assemblée nationale, le doublement du plafond d'exonération la prime carburant versées par les employeurs, qui va passer de 200 à 400 à 400 euros, or c'est précisément une prime qui ne vise que les salariés que les personnes qui travaillent, nous avons également 2ème mesure pour les personnes qui travaillent permis le cumul de cette prime carburant avec la prise en charge de l'abonnement transport collectif pour tous ceux qui, dans les territoires ruraux prennent leur voiture pour aller jusqu'à la gare, puis de la gare, prennent le train pour aller jusque sur leur lieu de travail et qui aujourd'hui ne peuvent pas cumuler l'indemnité carburant avec l'indemnité, transports collectifs, grâce à la décision : l'Assemblée nationale, des hommes, hein, ils pourront cumuler les deux c'est une 2ème mesure prise très précisément en faveur de ceux qui travaillent et qui prennent leur véhicule pour aller travailler, enfin 3ème mesure que je tiens à citer, nous avons revalorisé le barème kilométrique de l'impôt sur le revenu de 10 % en 2022, et je confirme que nous sommes prêts à revaloriser à nouveau le barème kilométrique de l'impôt sur le revenu en 2023 avec ces 3 mesures qui ciblent spécifiquement les personnes qui travaillent, je pense que nous pouvons conjuguer réduction du prix du carburant à la pompe pour tous les Français et renforcement de ses mesures pour tous ceux qui travaillent et qui sont particulièrement pénalisées 3ème grandes orientations de ce projet de loi de finances rectificative le travail. Nous avons la conviction avec Gabriel Attal avec l'ensemble des membres du gouvernement que la meilleure réponse aux problèmes de pouvoir d'achat, c'est l'emploi, c'est le travail c'est la juste rémunération du travail, cela a été le fil rouge de notre action politique pendant 5 ans, cela restera le fil rouge de notre action politique pendant les 5 années qui viennent jusqu'à ce que nous atteignons ce qui n'a pas été en franc atteint en France depuis un demi-siècle, le plein emploi. Le PLFR vise donc à rendre du pouvoir d'achat à nos compatriotes, par la valorisation de leur travail, grâce à des mesures très ciblées qui ont été complétées par un certain nombre d'amendements de certains groupes présents aujourd'hui, première mesure, la monétisation des RTT je, je vois bien le débat qui a émergé à la faveur de cette proposition soit monétisation des RTT, mais je vous confirme que nous estimons que permettre aux salariés qui souhaitent travailler plus d'augmenter leur rémunération en en monétiser leur RTT nous paraît une mesure juste, efficace et qui mérite d'être retenu la défiscalisation des heures supplémentaires, l'idée de relever le plafond d'exonération fiscale de 5000 à 7500 euros va dans la bonne direction et je vous confirme que nous sommes prêts à rendre cette défiscalisation des heures supplémentaires, porté à 7500 euros définitive. Et il me semble que le caractère définitif de cette mesure garantira là aussi sa justice et je le dis pour ceux qui s'hein. Enquête sur les RTT, c'est le complément de cette mesure pour que l'ensemble des personnes qui souhaitent travailler puissent être mieux rémunérés, ça restera notre philosophie et personne n'arrivera à me convaincre qu'il vaut mieux inciter les Français à travailler moins et à gagner moins, il me semble, de ces temps de difficultés, il vaut mieux travailler davantage et avoir la juste rémunération de son travail, j'attends avec impatience ce débat qui nous permettra d'échanger sur ce sujet, même chose sur les heures supplémentaires. Le groupe Les Républicains a proposé que nous avancions encore plus loin sur les heures supplémentaires, en demandant à ce que les entreprises puissent voir leurs charges sociales patronales réduites, elles le sont déjà, pour être tout à fait précis de 1 euros 50 pour les entreprises de moins de 20 salariés. Le groupe a proposé que pour les entreprises de 20 à 250 salariés, je le dis devant le président Retailleau il y ait à nouveau une réduction de 50 centimes d'euros, qui n'existe pas aujourd'hui pour alléger le coût pour les entreprises qui sont les PME 20 à 250 salariés. J'estime que cette une idée constructive utile pour le pays, à laquelle je suis favorable

ça a un coût, nécessairement, je sais que l'inflation et que les revalorisations qui ont été engagées, peuvent susciter des inquiétudes, mais je rappelle que les députés dans leur grande sagesse. Ont déjà commencé à tenir compte de l'impact de l'inflation sur les collectivités locales et que le gouvernement, qui sans doute n'avait pas fait suffisamment sur le sujet, a accepté de faire davantage, à l'occasion des débats à l'Assemblée nationale. Leur pays. Notamment à l'initiative, je le dis pour le groupe socialiste de Madame Christine Pires Beaune nous avons porté, preuve que le gouvernement être eux oecuménique. Nous avons accepté 180 millions d'euros de dispositifs ciblés qui va s'adresser aux 6000 communes qui sont les plus en difficulté. Qui peine à faire face à la hausse du prix de l'énergie et à la hausse du point d'indice, les collectivités d'outre-mer sont particulièrement concernés par ce dispositif, je sais que vous y êtes sensible et et je sais que nous aurons d'autres discussions sur le sujet, nous avons également accepté de compenser la hausse du RSA pour les départements, nous avons eu de longs débats sur le sujet, nous avons accepté une compensation de 120 millions d'euros, ce qui fait au total déjà 300 millions d'euros de compensation pour les collectivités locales, confrontés aux conséquences de l'inflation sur le prix de l'énergie ou sur le prix d'un certain nombre de fournitures, je suis certain que ce débat ne s'arrêtera pas là et se poursuivra ici avec l'ensemble des groupes. Je vais vous dire ma disponibilité à faire encore plus attention aux collectivités qui en ont réellement besoin pour bénéficier de ce filet de sécurité, je le dis devant le rapporteur général qui, je le sais et particulièrement mobilisé sur ce sujet, mais je sais aussi que j'ai ici devant moi une assemblée de sénatrice et de sénateurs aussi attaché que moi à la bonne tenue des comptes publics et qui savent que pour bien tenir les comptes publics, il faut demander des efforts à tous à l'État, aux dépenses sociales, mais aussi aux collectivités locales, tout n'est pas possible financièrement, ni pour l'État, ni pour les collectivités locales, ni pour les dépenses sociales, j'appelle donc chacun au sens des responsabilités pour que nous ayons une enveloppe qui protège les collectivités locales, mais qui ne menace pas nos finances publiques. Au fond, il y a un sujet qui. Ah défrayé la chronique depuis plusieurs semaines, qui est le sujet de la taxation des superprofits me méfie des termes la taxation par définition et les superprofits parce que je pense qu'il recouvre des réalités qui sont bien différentes et je sais que un certain nombre d'entre vous, notamment le groupe de l'Union centriste ont déposé des amendements sur ce sujet. Je voudrais dire d'abord que je comprends, j'imagine que d'autres, bon dans cette partie, dans de l'hémicycle, l'ont fait également, sinon je serais surpris, voire, pour tout dire le fond de ma pensée déçu. Je veux dire d'abord que, au risque de vous surprendre. Je comprends le raisonnement qui vous a amené à faire cette proposition. Car j'imagine bien que ce raisonnement est d'abord dictée par un souci de justice. sous ce souci de justice qu'il soit sur les bancs de droite ou les bancs de gauche de cette assemblée trouvera toujours avec moi sont plus fervent soutien. Il faut partager le fardeau de l'inflation. Et je ne l'ai jamais contesté. Et j'ai toujours dit comme ministre de l'Économie et des finances, que ce n'était pas à l'État tout seul de porter le fardeau de l'inflation, nous avons déjà fait beaucoup, notamment avec le bouclier énergétique hein les ménages font évidemment beaucoup parce qu'ils supportent une part de cette inflation dans leur vie quotidienne, bah, il est légitime que les entreprises portent elles aussi une part du fardeau de l'inflation. Mais je voudrais rappeler, et c'est là que je me méfie de ces termes un peu brutaux de taxation sur les superprofits. Je voudrais rappeler que l'immense majorité des entreprises, des petites entreprises, des PME, des TPE, des indépendants souffrent de l'inflation, elle va augmenter le prix de leurs intrants, elle voit augmenter leurs prix de leurs approvisionnements, elles ont des délais dans leur approvisionnement, elles sont lésés par le prix des matières premières, elles ont dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans la distribution, dans l'industrie agroalimentaire, des difficultés de recrutement, comme elle n'en ont jamais connu, tenant compte aussi des difficultés de nos entreprises, je voudrais également rappeler. Que lorsque vous regardez les négociations salariales, vous apercevez que beaucoup d'entreprises participent à la lutte contre l'inflation que la meilleure façon pour une entreprise de participer à la lutte contre l'inflation, c'est pas d'être taxé, c'est d'augmenter les salaires de leurs salariés et je veux redire ici avec beaucoup de force que toutes les entreprises qui le peuvent, toutes les entreprises qui en ont les moyens, toutes les entreprises qui ont les marges nécessaires doivent augmenter les salaires et toutes celles qui ont des inquiétudes en me disant, légitimement, mais on ne peut pas se projeter au-delà de quelques mois, on redoute ce que va être l'année 2023, on ne veut pas s'engager de ces augmentations de salaire, je peux entendre ça mais je dis à ces entrepreneurs, vous avez des instruments pour augmenter la rémunération de vos salariés sans menacer la survie d'autres entreprises, ça s'appelle la participation, ça s'appelle l'intéressement, ça s'appelle la prime défiscalisée utiliser ces instruments qui augmente la rémunération sans affecter la survie de l'entreprise. En revanche, quelques entreprises, effectivement, font des bénéfices importants et elles doivent participer à l'effort collectif mais doivent y participer, comme le font CMA CGM totale ou Engie en rendant l'argent directement aux Français plutôt qu'au Trésor public et je pense qu'il est plus juste, plus efficace. Plus conforme aux convictions de cette majorité de procéder de cette manière-là que de céder à nouveau au réflexe pavlovien un gamme si vous voulez, je m'intéresse à mes amis de l'Union centriste, je ne crois pas que ce soit conforme à votre ADN politique que de multiplier les taxes et les prélèvements cette approche que nous proposons, elle est plus juste car elle ne pénalise pas les entreprises, ce que vous allez toutes frappé de manière indifférente, quelle que soit leur situation par une taxe qui découvrira sans exception, elle est plus efficace, car elle va directement dans les poches de nos compatriotes 20 centimes de remise à la bombe, cela mettra le prix du carburant a d'euros 50 à la rentrée et je pense que nos compatriotes préféreront voir un litre d'essence un euros cinquante à la rentrée, plutôt qu'une ligne du Trésor qui est abondé grâce à une nouvelle taxe à la fin de l'année 2022. Enfin c'est plus conformes à notre ligne politique, car cela va dans le sens de la baisse des impôts et cela favorise l'attractivité de notre territoire et à tout ce qui me donne sans cesse l'exemple de la Grande-Bretagne, de l'Italie qui ont accès superprofits je voudrais juste rappeler que eux ont des industries productrices notamment la Grande Bretagne qui extraient du pétrole en mer du Nord et que ces pays-là ont de 10 à 15 points de prélèvements obligatoires de moins que la France, quand on est le pays le plus taxé de tous les pays européens, on ne rajoute pas une taxe supplémentaire à toutes les taxes qui existent déjà. déjà. Nous vous proposons et nous sommes ici pour débattre.

et je sais que sur les bancs du Sénat, il y aura des débats qui sont animés, s'agit pas de faire des meetings politiques mais il ne s'agit pas que la démocratie tombe dans l'ennui dans le respect de la considération de chacun, ayons la volonté d'exprimer avec force et conviction nos arguments, c'est ce qui rendra notre débat intéressant pour nos compatriotes, enfin, nous proposons la suppression de la contribution sur l'audiovisuel public qui rendra 138 euros de pouvoir d'achat aux ménages qui, là aussi, j'en suis certain animera notre débat cette décision est conforme à notre politique constante de baisse des impôts, nous avons travaillé, un dispositif de financement durable audiovisuel public qui est un gage de son indépendance, j'espère que nous parviendrons là aussi à un équilibre constructif sur ces sujets, je voudrais enfin vous remercier de votre présence aujourd'hui nous sommes le premier août. Le débat s'est prolongée très tard dans l'été, donc vous voyez que c'est toujours avec beaucoup de joie que je suis présent dans cet hémicycle pour discuter, dialoguer avec mes amis sénateurs. Allez, on va se calmer, ça sert à rien, je vous rappelle qu'il a, après le débat, il y a 450 amendements donc. On a prévu cette nuit la nuit prochaine, alors on va peut-être faire ça calmement, hein, je salue d'abord la préside la présence du président du Sénat parmi nous et j'appelle monsieur Gabriel Attal Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargé des comptes publics à s'exprimer. Monsieur le président de séance, monsieur le président du Sénat, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Ministre, depuis 2 ans face aux aléas et aux incertitudes, aux soubresauts notre réponse n'a jamais varié à grand défi, grands moyens pendant la pandémie nous avons assumé l'installation de puissant amortisseur le quoi qu'il en coûte, a inspiré l'investissement inédit d'une puissance publique résolus à sauver les entreprises à préserver les compétences des salariés à protéger le pouvoir d'achat en investissement saluée par les économistes mais aussi par les Français et notamment par la France, des entrepreneurs, des artisans, des commerçants qui a redécouvert que l'état et en particulier l'État providence était aussi là pour eux, ce choix de la protection, nous l'avons fait sans jamais perdre de vue notre boussole, la préparation de l'avenir, par delà les crises nous n'avons jamais cessé d'agir avec 2 lignes de force majeure, la valorisation du travail et la transition écologique et énergétique, or nous n'aurions pu ni protéger sur le moment ni préparer l'avenir, si dès le début du précédent quinquennat nous n'avions pas remis de l'ordre dans nos comptes, c'est parce que notre pays a regagné sa crédibilité en repassant dès 2018 sous les 3 % de déficit public que nous avons pu emprunter pour protéger les Français au moment où sévissait la Covid 19, c'est parce que notre pays est sorti de la procédure pour déficit excessif à Bruxelles, que nous avons regagné une certaine crédibilité en Europe et plus convaincre nos partenaires de déployer un plan de relance historique face au retour de l'inflation. Face aux difficultés de la vie chère pour nos concitoyens, nous continuons à agir pour les protéger, nous continuons à prendre des mesures pour être à leurs côtés et pour chercher au maximum à amortir ce coût de l'inflation pour les Français, nous le faisons en maintenant le cap fixé il y a 5 ans, emporté par Bruno Lemaire et nous poussons encore davantage les moteurs de notre stratégie, moins d'impôts, moins de dette, plus de croissance, nous le faisons avec 2 lignes de force qui, je le sais, résonneront particulièrement dans cet hémicycle, la recherche du compromis et la responsabilité. La recherche du compromis, elle est bien connu dans cet hémicycle, malgré ma très jeune expérience en la matière, j'ai pu mesurer à chaque fois que j'ai eu à défendre des textes, travailler sur des textes dans cet hémicycle que nous parvenions à trouver des compromis au service de l'intérêt général, entre des groupes différents, faisant partie de la majorité ou de l'opposition et je suis persuadé qu'il en sera de même dans ce débat, la responsabilité, c'est celle de continuer à préserver nos finances publiques et j'ai entendu ces dernières semaines, un certain nombre de déclarations qui ont été formulés notamment dans la majorité sénatoriale sur l'importance de tenir nos comptes et de rester sur une trajectoire de réduction des déficits, qui est un enjeu absolue de crédibilité un mange aussi de pérennité pour nos services publics, nous maintenons donc notre cap et les Français le voient, c'est pour cela que ce PLFR est un peu à l'affaire de stabilité et de dignité, stabilité de notre politique économique et dignité car face à l'inflation, nous ne mettons pas davantage la tête des Français sous l'eau par le poids des impôts qui augmentent, nous les aidons à vivre quand la vie devient trop cher, mesdames et messieurs les sénateurs, le texte que nous vous présentons aujourd'hui traduit donc un effort massif pour un défi d'ampleur cet effort massif de 44 milliards d'euros se décompose en 3 blocs des crédits budgétaires pour protéger aujourd'hui le pouvoir d'achat des Français, des crédits budgétaires pour continuer de préparer l'avenir des crédits budgétaires enfin pour honorer nos engagements financiers et financer l'alourdissement de la charge de la dette, ces 3 blocs traduisent donc à la fois l'ambition qui est la nôtre et le cadre dans lequel nous agissons, qui est un cadre contraint ainsi, et contrairement à ce qu'indique son titre, projet de loi de finances rectificative, ce texte n'est pas le reflet d'une trajectoire que l'on rectifie ou d'une ligne que l'on corrige à la marge, non, ce texte est impuissant, rédacteur au service des Français de notre économie, de notre cohésion, il est le moteur d'une stratégie visant à permettre aux Français de dépenser moins et de gagner plus, dépenser moins pour l'énergie à la maison, grâce à la prolongation du bouclier tarifaire jusqu'à la fin de l'année, Bruno Lemaire là rappeler dépenser moins pour se déplacer, grâce aux crédits que nous ouvrons pour accompagner les Français en la matière, dépenser moins en payant ses impôts, avec la suppression de la contribution à l'audiovisuel public, les débats à ce sujet seront nourris mais il me semble que les garanties que nous avons apporté avec celle que nous pourrons toujours ajouter dans le cadre du débat, nous permettront de vous convaincre, gagner plus avec le financement des revalorisations des prestations sociales, des retraites ou de la rémunération de nos fonctionnaires gagner plus également, avec les avancées qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale pour valoriser celles et ceux qui travaillent dans notre pays, je pense notamment au relèvement à 7500 euros du plafond d'exonération des heures supplémentaires ou encore à la possibilité de monétiser les RTT, Bruno Lemaire le disait à l'instant, certains parmi vous, notamment dans la majorité sénatoriale propose de pérenniser ce dispositif évidemment fidèle à l'esprit d'ouverture et de compromis que nous avons est particulièrement engagée sur la valorisation du du travail, nous serons évidemment très attentif et réceptif à ces propositions, ce texte répond donc aux chocs d'aujourd'hui, mais il vient également préparer l'avenir, je le disais en maintenant tout d'abord notre trajectoire budgétaire, car un pays qui ne tient pas ses comptes ne peut être demain un pays libre et fort, préparer l'avenir, également, en renforçant notre souveraineté industrielle et la transition énergétique avec le financement de la prise de contrôle à 100 % d'EDF et la prolongation du bonus écologique pour les Français qui changent de véhicule, préparer l'avenir en modernisant notre rapport avec les entreprises et en luttant contre la fraude avec la facturation électronique pour les entreprises, s'agissant de la lutte contre la fraude, là aussi, je sais que la majorité sénatoriale porte notamment un amendement visant à lancer la carte Vitale biométrique, là aussi, nous y sommes favorables, préparer l'avenir aussi en luttant en continuant à agir pour l'emploi avec des crédits supplémentaires pour l'apprentissage 1 milliard 800 millions d'euros pour France compétences et près de 750 millions d'euros pour les primes d'apprentissage ces chiffres reflètent le dynamisme de cette politique, une réussite majeure du quinquennat précédent avec plus de 700000 jeunes en apprentissage alors qu'ils étaient moins de 300000 en 2017, au cours de l'examen de ce texte, nous aurons des échanges, des débats, des discussions sur un certain nombre de mesures ou de paramètres ces débats témoigneront d'une chose : nous avons tous la volonté de répondre présent pour protéger nos concitoyens face au choc économique mondiale que nous traversons, mais il y aura, je crois, au coeur de nos débats, plusieurs grandes questions qui émergeront, première question ce choc conjoncturel doit-il nous conduire à priver nos services publics et notre modèle social des ressources indispensables à leur pérennité en adoptant soit des baisses de taxes ou d'impôts pérenne massive et non ciblée qui ne changerait pas la vie des Français seconde question de choix doivent-ils nous conduire à nous priver de toute marge de manoeuvre pour continuer à préparer l'avenir et investir, vous savez, nous répondons par la négative à ces 2 questions, parce que nous devons la vérité aux Français et la vérité, c'est que la guerre en Ukraine, nous a fait changer d'époque, inflation forte croissance plus faible, nous estimons désormais que le PIB devrait croître de 2,5 % en volume cette année la croissance résiste, comme l'a dit, Bruno Lemaire, mais nous sommes conscients des aléas qui existe au niveau mondial, la vérité c'est que nos finances publiques sont à risque en raison de l'inflation et de la remontée des taux d'intérêt, la charge de la dette que je rappelais au début de mon intervention s'élèvera cette année à 17 milliards d'euros supplémentaires en comptabilité nationale, c'est l'équivalent de 2 fois le budget du ministère de la justice, il faut le dire clairement, la parenthèse de l'emprunt gratuit c'est bel et bien refermée et toutes les décisions que nous prenons, qui ont pour conséquence d'alourdir les déficits et la dette sont prises dans ce contexte là, il faut toujours l'avoir en tête, c'est pourquoi nous préférons toujours des mesures ciblées, temporaires qui réponde véritablement à des difficultés constatées sur le terrain, en clair, nous sommes passés du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte, c'est-à-dire de la logique presque inconditionnel qui a prévalu au plus fort de la crise du Covid à une approche plus ciblée, plus juste et donc plus efficace tout en étant soutenable pour les finances publiques à ce titre, je le dis ici, nous réaffirmons notre objectif maintenir le déficit de de nos administrations publiques à 5 % cette année et le ramener en dessous de 3 % d'ici à la fin du quinquennat nous assumons de tenir les comptes de tenir les comptes pour respecter nos engagements de tenir nos comptes pour conserver notre indépendance pour préserver une force de frappe une force d'investissements budgétaires face aux grands défis que nous devons affronter. Vous des du des, donc les lignes rouges que nous refuserons toujours de France de franchir dans ce débat, laisser filer les comptes et augmenter les impôts. Je vous disais au début de mon intervention que nous nous trouvions dans un moment charnière, ce texte c'est capital capital du fait du contexte dans lequel il s'inscrit capital par les moyens financiers exceptionnels qu'il mettent en oeuvre capitale parce que pour la première fois, nous supprimons un 2ème impôt en 5 ans, avec la réforme du financement de l'audiovisuel public alors que le texte initial faisait le choix d'un financement au travers de crédits budgétaires, le groupe majoritaire de l'Assemblée nationale a opté pour l'affectation d'une fraction de TVA ce mode de financement étant considérée comme offrant davantage de garanties pour les sociétés audiovisuelles et leurs salariés, je sais que le débat aura lieu ici tout à l'heure comme il l'a eu lieu à l'Assemblée nationale, il y a quelques jours, je sais qu'un certain nombre d'entre vous, considère qu'il faudrait consulter davantage, je veux rappeler qu'il y a eu énormément de rapports énormément de travaux qui ont été menées notamment dans cette assemblée, je pense notamment aux très bon rapports Igounet Karoutchi qui a été. Remis il y a quelques mois, il y a eu des rapports auparavant. Monsieur Assouline tout à fait, il y a eu des rapports multiples, il y a eu des travaux multiples et tout le monde s'accorde sur le fait que la contribution à l'audiovisuel public, telle qu'elle existe aujourd'hui est obsolète, injuste et daté et qu'il faut donc la supprimer et donc nous aurons ce débat mais je le dis, qui est un débat important. La. De la même manière, je souhaite que nous puissions trouver et nous souhaitons et Bruno Lemaire, trouver le bon point d'équilibre, s'agissant de la réponse à adopter aux demandes de soutien des collectivités locales fragile dans le contexte d'inflation sur les prix de l'énergie de revalorisation du point d'indice et du RSA, je veux rappeler, comme l'a fait Bruno Lemaire que le mécanisme de filet de sécurité qui a été introduit dans le texte à l'Assemblée nationale est une traduction concrète concrète de l'esprit de dialogue qui nous Amin qui nous anime la rédaction de l'article IV terre est en effet le fruit d'un travail engagé avec l'ensemble des groupes politiques qui ont en bonne intelligence conforter l'amendement proposé par la députée socialiste Christine Pires Beaune je sais que de nombreux amendements émanant de l'ensemble des groupes ont été déposées sur ce sujet, j'espère que notre débat permettra de définir les bons critères permettant de cibler les collectivités qui ont besoin d'un soutien sans constituer une charge démesurée pour le budget de l'état et en ayant en tête que nous aurons rendez-vous au moment du projet de loi de finances pour aborder de manière plus structurelle la question du financement des collectivités locales, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'urgence, l'urgence pour les Français qui le connaissent le plus de difficultés, l'urgence pour les collectivités qui connaissent le plus de difficultés, je ne crois pas que ce soit le moment du grand débat sur le financement des collectivités locales, nous avons un projet de loi de finances pour cela dernière illustration et j'en termine par là, de cet esprit de dialogue, l'Assemblée nationale a voté une dotation de 10 millions d'euros pour soutenir les collectivités en matière de Titres sécurisés et nous savons que beaucoup de nos concitoyens peinent encore à pouvoir bénéficier d'un rendez-vous pour renouveler leur carte d'identité ou leur passeport après discussions avec plusieurs sénateurs, dont le rapporteur général Jean-François Husson, qui a déposé un amendement tendant à renforcer le dispositif nous pensons avec Bruno Lemaire, qu'il est justifié de renforcer ce dispositif et nous soutiendrons donc l'amendement porté par le rapporteur général Husson. Sur les collectivités locales, comme sur tous les autres sujets, faisons en sorte de définir ensemble le meilleur dispositif en cessant d'opposer finances locales et finances de l'État, car à la fin, il n'y a qu'un seul contribuable et qu'un seul site concitoyens celui que nous avons le devoir de servir, je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre. La parole est maintenant Monsieur Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances pour dix minutes, vous avez la parole monsieur le rapporteur général. Monsieur le président, monsieur le président du Sénat, monsieur le président de la commission, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous pensons tous, je crois que l'État doit apporter son soutien à ceux qui sont confrontés. à ce nouveau contexte, des prix qui s'envolent depuis quelques mois. Et qui touche aussi bien nos concitoyens que les entreprises et les collectivités, et singulièrement les plus fragiles, parmi ceux-là. Telle est notamment l'objet de ce projet de loi finance rectificative depuis la crise sanitaire, la France semble s'être habitué à une réponse permanente des pouvoirs publics à chaque crise. Or, il faut trouver le bon niveau de dépenses sans risquer d'entretenir l'inflation ou de rendre ensuite plus difficile le financement de nos dépenses dans un contexte de hausse des taux et de renchérissement de la dette, sans oublier l'état de nos finances publiques, qui continue de se dégrader de manière préoccupante. Le ministre des Comptes publics vient encore de déclarer. Qu'on serait passé du. Quoi qu'il en coûte au combien ça coûte, selon moi, le combien ça coûte, monsieur le Ministre, ça coûte aussi cher, avec déjà 40 milliards d'euros consacré aux réponses apportées à l'accélération de l'inflation cette année avec le risque que cela dure encore un certain temps. Le texte qui nous est soumis, prend acte de la dégradation de la situation économique depuis décembre avec effectivement une prévision de croissance du PIB qui baisse de 4 à 2 Alors qu'elle pouvait paraître plus optimiste, les bonnes nouvelles sont arrivées, il faut le dire, de l'Insee, vendredi dernier, avec une première estimation de croissance au 2ème trimestres 2022 plus rassurante et qui donne du crédit à cette prévision. Mais j'observe que la consommation des ménages continue de baisser et que les indicateurs conjoncturels sont tous plus bas je note aussi que le FMI vient de réviser sa prévision de croissance pour 2023 de 1 virgule 3 à 1 % il nous faut donc rester prudent. Le projet de loi de finances rectificative traduite aussi le contexte inflationniste dans lequel nous évoluons et qui contribue non seulement à dégrader la consommation des ménages et l'investissement des entreprises et par suite, nos perspectives de croissance mais également à accroître le niveau des taux d'intérêt, et notamment ceux des à accroître le niveau des taux d'intérêt, et notamment ceux des obligations souveraines dans l'ensemble, les mesures prises par l'État, bouclier tarifaire remise à la pompe indemnité inflation ont eu des effets positifs sur l'évolution des prix et le revenu des agents. Néanmoins, ces résultats honte évidemment à Robert. Messieurs les ministres, c'est celui de l'aggravation des comptes publics en clair leur détérioration. Certes, le président de la finance rectificative révise à la hausse les prévisions de recettes publiques pour 2022 avec 50 milliards d'euros supplémentaires au titre des prélèvements obligatoires, mais en parallèle, les dépenses publiques augmentent de 60 milliards d'euros. Le niveau nos dépenses publiques n'est donc plus tout à fait en phase avec les objectifs de la date de programmation, les dépenses primaires s'établissant à 5 % au-dessus de leur niveau prévu. Alors, à cet instant, je constate que votre gouvernement laisse filer la dépense, alors même que nous sommes confrontés aux défis tant redouté de la dégradation des conditions de financement de notre dette, la charge de la dette, le ministre-Gabriel Attal vient de le rappeler représentent cette année 18 milliards d'euros supplémentaires, excusez du peu. Alors l'analyse du seul budget de l'État illustre très concrètement la politique du combien ça coûte, du gouvernement, les ouvertures de crédit de 53 8 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 47 6 milliards en crédits de paiement sont les plus élevés jamais réalisée dans un collectif budgétaire depuis l'entrée de la LOLF c'est donc considérable, les seules dépenses pilotables sont, elles, en hausse de 27 milliards d'euros, dont 18 1 milliards d'euros supplémentaires par ce seul projet de loi de finances rectificative alors je le dis, j'ai le sentiment qu'il n'y a plus de pilote pour les dépenses de l'État. Le texte anticipe un déficit de 177 8 millions d'euros, en hausse lui aussi de 25 milliards d'euros par rapport à la loi de finances initiale. En revanche, l'endettement au titre de 2022 se maintient. Pour autant, c'est bien toujours avec une dette que le déficit est financé, à savoir la dette qui a été contracté il y a 2 ans en 2020, l'État avait alors dimensionné ses émissions de dette par rapport au déficit prévu en milieu d'année, et il s'est avéré moins élevé que prévu, l'état donc conserver cette trésorerie surabondante qu'ils proposent d'utiliser pour financer le déficit actuel. Pour résumer, mes chers collègues, ce budget rectificatif prévoit 50 milliards d'euros de dépenses supplémentaires financés par 30 milliards de surcroît de ressources et 20 milliards d'euros de dettes émises il y a 2 ans. Vous le voyez, les dépenses nouvelles s'accumulent pour la 3ème année consécutive, si l'on pouvait espérer que la crise sanitaire soit temporaire, je crois que ce n'est pas le cas de la crise énergétique et environnementale qui s'annonce, on verra peut être le prix des carburants et du gaz redescendre temporairement si les tensions internationales venait à s'apaiser mais il ne faut pas se tromper. C'est un monde nouveau qui s'annonce, auquel il va falloir nous adapter et où les mesures budgétaires ne pourront pas constituer des réponses durables, le soutien du pouvoir d'achat par la dépense publique a atteint ses limites, et ce sera très prochainement, l'heure des choix douloureux. Quelles dépenses publiques voudrons-nous. à quel niveau quelles priorités fixons-nous alors que nous ne pourrons plus financer aussi facilement par la dette et que la dette accumulée pèsera elle dans nos comptes. Compte tenu de ces éléments, vous comprendrez que je n'ai pas proposé à la commission des finances de nouveaux dispositifs qui viendrait s'ajouter à la liste déjà longue de ceux déjà prévus dans les 2 projets de loi, pouvoir d'achat, loi de finances rectificative le texte sorti de l'Assemblée nationale comprend des avancées qui vont dans le bon sens, comme la hausse du plafond, applicable pour la défiscalisation des heures supplémentaires ou bien encore la monétisation des RTT, il faut en effet soutenir les salariés et offrir de la souplesse dans la gestion du temps de travail en ces temps de pénurie de main d'oeuvre. La commission des finances propose d'ailleurs un amendement qui vise à rendre pérenne. le le le la bienveillante le bienveillante ta vie que vous avez déjà délivré sur la hausse du plafond, applicable à la défiscalisation des heures supplémentaires à 7500 euros soutenir la valeur travail et les salariés les plus exposés, les plus précaires, c'est également ce qui a guidé notre choix de remplacer la prime de rentrée exceptionnelle réservée aux ministres ma sociaux par une majoration exceptionnelle, coup de pouce de la prime d'activité. S'il faut mettre fin à la politique du chèque permanent, nous prévoyons en revanche une rallonge de la participation financière de l'État à l'exercice des missions des banques alimentaires, à hauteur de 40 millions d'euros pour tenir compte des importantes difficultés qu'elles connaissent. Sur le bouclier mises en place au titre, l'énergie, nous nous rallierons globalement à ce qui a été décidé, notamment avec le soutien pour tous et plus conséquent, par le biais de la remise carburant je suis aussi favorable à l'extension du bouclier tarifaire aux ménages qui se chauffent au fioul et 230 millions d'euros votée à l'Assemblée nationale ne seront pas de trop. Pour autant, j'estime que nous arrivons au bout de la logique. La transition écologique doit être menée, il nous faut recouvrer notre souveraineté énergétique et l'état de nos finances publiques ne nous permettra pas de poursuivre ainsi au-delà de la fin de cette année. Aussi, par exemple, cette mesure sur le fioul doit-elle être ciblées pour représenter un soutien financier suffisamment conséquente pour ceux qui en ont besoin, éviter le saupoudrage. Nous regrettons vivement la perte de 3 milliards que représente la suppression de la contribution à l'audiovisuel public. Le montant de la TVA, qui le remplace sera autant qu'il ne sera pas utilisé à autre chose et ne peut de toute façon être affectés que jusqu'à fin 2024 en vertu de la LOLF que nous avons voté sous la pression insistante d'ailleurs de la précédente majorité. Le gouvernement doit doit donc utiliser les 2 années à venir pour mener une véritable réforme de l'audiovisuel public, en y associant un mode de financement efficace à cet égard les propositions de la mission menée par nos collègues Jean-Raymond Hugonet et Roger Karoutchi sont sur la table, saisissez-là, messieurs les ministres, vous gagnerez du temps enfin concernant les compensations allouées aux collectivités territoriales. La commission des finances propose tout d'abord de renforcer le filet de sécurité issu des travaux intergroupe de l'Assemblée nationale. Et qui touche le bloc communal, on le fait, comment en assouplissant les critères d'éligibilité et les modalités du calcul de l'aide dans la même logique que la compensation pour les départements de la revalorisation du RSA nous proposons également de compenser pour les régions, le coût de la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle. Nous continuons de refuser les réserves de budgétisation, que le gouvernement se constitue. L'expérience de 2021. Et les nouveaux reports de crédits massifs réalisés début 2022. Plus de 29 milliards d'euros, messieurs les Ministres, montre que les pratiques se poursuivent. Hé bien. Nous proposons de supprimer 4 milliards 5 qui ne nous paraissent pas justifiés, nous oeuvrons assis en faveur d'une gestion budgétaire rigoureuse en évitant de prendre le pli de certaine aisance ou faciliter contraires au redressement nécessaire de nos comptes publics pour offrir à la France et aux Français un meilleur avenir, Monsieur le président, monsieur le président du Sénat, messieurs les ministres, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, le projet de loi de finances rectificative que nous examinons aujourd'hui est présenté par le gouvernement comme le 2ème volet de son paquet, pouvoir d'achat, mais bien sûr, il ne se résume pas à cela : tout d'abord, c'est un collectif budgétaire, qui prend en compte le nouveau contexte macro-économique avec une baisse de la prévision de croissance de 4 à 2,5 % et d'importants ajustements en recettes et en dépenses, ce projet de loi intègre aussi des mesures nouvelles qui ne sont pas toutes liées au pouvoir d'achat, comme par exemple la suppression de la redevance pour audiovisuel public, on en a parlé le report d'un an de la suppression de la fiscalité spécifique au gazole non routier ou encore la renationalisation d'EDF, enfin, surtout, il présente une réponse très partielle au problème de pouvoir d'achat de certains de nos compatriotes l'Insee viennent indiquer que l'inflation avait atteint en juillet 6 virgule avant même ces nouveaux chiffres le choc en 2022 étaient déjà estimé à 66 milliards d'euros, soit environ mille euros par habitant et 4,3 % du revenu des ménages enfin l'OFCE a calculé que sur 5 % d'inflation générale les 10 % des ménages les mieux lotis subissait une inflation de 2 et demi % tandis que les 10 % des ménages est le plus exposé subissait une inflation de 8 virgule cinq la réponse dodo être différenciées, ce que ne fait pas suffisamment de ce PLFR. Du point de vue déséquilibre ce collective aggrave le déficit du budget de l'État, la hausse des dépenses est en effet très significative de 44,2 milliards d'euros, dont la moitié pour le pouvoir d'achat, ce qui ne compense pas la réévaluation des recettes fiscales, la charge budgétaire de la dette augmente dès cette année de 11,9 milliards d'euros, il ne s'agit pas pour moi, évidemment, de remettre en cause la nécessité de soutenir les ménages ou de renforcer l'intervention publique face aux défis qui s'annoncent, notamment en matière de résilience et la transition énergétique, je ne peux en revanche que déplorer que dans la situation particulièrement délicate que nous connaissons avec des comptes publics dégradés, des perspectives de croissance incertaines et une hausse elle certaines des taux d'intérêt, le gouvernement poursuive sa politique de désarmement fiscal aujourd'hui la suppression de la redevance audiovisuelle créerait un nouveau manque à combler de 3,7 milliards d'euros et fragiliserait l'audiovisuel public demain la poursuite de la baisse des impôts de production aggraverait la situation de plusieurs milliards d'euros, alors même que l'essentiel des baisses d'impôts déjà réalisé se sont faites sur le dos de la dette, un regard, une nouvelle fois, rien n'est proposé pour prélever les acteurs économiques ayant les plus fortes capacités contributives afin de rééquilibrer les comptes, aucun projet d'imposition du Patrimoine alors que l'épargne accumulée au cours de la crise par les plus hauts déciles de revenus est très importante, aucune taxation des bénéfices exceptionnels de certaines grandes entreprises. Comment, à ce stade de mon propos ne pas évoquer les résultats des grands groupes énergéticien français au 1er rang desquels Total triplement des profits semestriels à 18 7 milliards de dollars pour une production du même ordre qu'en 2021, une aubaine de marché supporté par nos concitoyens comme l'a écrit Valérie Rabault récemment, comment peut-on accepter, Monsieur le Ministre votre propos taxer Total, je vous cite n'est qu'une facilité et non une mesure de justice, il faut oser, il faut oser, Monsieur le Ministre, dire que la reprise d'un bénéfice exceptionnel, conjoncturel pour le redistribuer vers les populations les plus fragiles de notre pays qui participent d'ailleurs à la constitution de ce bénéfice ne serait pas une mesure de justice et comment mettre en parallèle quelques mesurettes, excusez-moi de le dire ainsi, d'un coût de 500 millions d'euros quand même mais bien mal ciblées. Alors c'est pas votre faute, hein, c'est la faute de quelques députés je ne citerai pas de l'Assemblée nationale. Mais bon, comment le comparer avec finalement les 5 milliards à peu près 10 fois plus minimum que cette taxe pourrait rapporter, il est d'ailleurs savoureux de constater que nos grandes entreprises argue d'une activité internationale lorsque tout va bien et d'un siège social en France, lorsque des crises surviennent de tout cela, les Français ne veulent plus, quand en plus Total annonce qu'une partie de ces profits sera consacrée voyons au développement. Non à la transition énergétique non à l'amélioration des salaires de ses salariés. Peut-être, mais au moins pour 2 milliards d'euros au rachat d'actions au seul but de faire monter la valeur de l'action, alors oui, mes chers collègues, agissons et votons cette taxe exceptionnelle. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Éric Bocquet pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste pour cinq minutes. Monsieur le président, monsieur le président du Sénat, mes chers collègues, messieurs les ministres. Au soir de sa victoire, le 24 avril dernier le président de la République avait eu ces mots : je le cite : ce vote m'oblige, pour les années à venir, cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève. La colère et les désaccords doivent aussi trouver une réponse, il faut enfin considérer toutes les difficultés des vies vécues et les difficultés qui se sont exprimés, nous voici 3 mois plus tard en séance pour débattre d'un projet de loi de finances rectificative qui aurait dû marquer le début de cette ère nouvelle qui nous fut annoncé par l'oracle de l'Élysée, du discours aux propositions formulées le gouffre est béant. Pendant les 2 campagnes du printemps, les fractures profondes qui minent notre société sont clairement apparus et parmi les préoccupations de nos compatriotes, s'est exprimé très fortement la question du pouvoir d'achat. Ainsi, ce sont 40 % des Français qui ne partent pas en vacances cette année dans notre pays, pourtant 6ème puissance économique mondiale. Celles et ceux qui partent, constate la hausse vertigineuse du prix des carburants qui les privera des petits plaisirs des vacances, la sortie au restaurant en famille ou la crème glacée offertes aux enfants au au soleil de la canicule. Sans doute ces d'automobilistes ont-ils apprécié d'apprendre que le groupe Total énergies dont il est beaucoup question ces jours-ci, a réalisé un bénéfice Net de 17,7 milliards d'euros pour le 1er semestre 2022, et que de surcroît on apprend que ce groupe n'a pas payé d'impôts en France en 2020 et en 2021. La Fédération française des banques alimentaires a réalisé il y a quelques semaines, une étude visant à mesurer l'impact de l'inflation, qui vient de franchir la barre des 6 %. Sur les personnes accueillies dans le réseau des banques alimentaires 1er réseau d'aide les banques alimentaires viennent en aide à 2, 2 millions de personnes en situation de précarité, je relèverai trois des constats que cette étude met en évidence, d'abord, une hausse du budget alimentation pour la moitié des foyers interrogé ensuite une hausse des prix qui affecte davantage les familles avec enfants, enfin un report massif sur les produits les moins chers. De l'autre côté du spectre, nous évoquions la santé économique de Total énergies un groupe qui n'est pas une exception, l'ensemble des groupes du CAC 40 ont dégagé collectivement quelque 174 milliards d'euros de bénéfices, du jamais vu dans le capitalisme français et une hausse de 70 % par rapport au précédent record rapporter une échelle plus humaine, plus accessible au commun des mortels, les groupes du CAC 40 ont gagné 5517 euros chaque seconde. Ainsi donc, la question des profits à-t-elle légitimement surgit dans les débats. Nous pourrions tout autant cité NJ qui a engrangé des profits records l'an dernier avec 3,7 milliards le logisticien CGA CGM qui transportent des conteneurs a réalisé 18 milliards de profits en 2021 et a déjà encaissé 7,2 milliards au 1er trimestre de cette année, l'Italie et le Royaume-Uni, cela a été dit-on, tous 2 mis en mis en place une taxe sur les superprofits des énergéticiens à hauteur de 25 % d'autres États européens ont suivi le même chemin, à l'évidence, en France, les actionnaires sont cajoler dorlotés, chouchoutés dans le quinquennat précédent, vous avez fait ce choix de baisser la fiscalité du capital avec la suppression de l'ISF et la mise en place du prélèvement forfaitaire unique pour les dividendes ces choix n'ont eu comme effet que de concentrer davantage encore la richesse, puisque les 10 % les plus riches détiennent la moitié des actifs qui financent l'économie y a-t-il eu au moins un effet sur l'investissement, on peut en douter, monsieur le Ministre vous appelait régulièrement à la modération en matière de distribution de dividendes s'agissant du pouvoir d'achat, vous demandez aux entreprises qui le peuvent, de faire un geste, à l'évidence, ce geste ne sont que des signaux faibles, souvent très faible, Total a annoncé une remise d'été de 12 centimes par litre valable uniquement en juillet et en août, et seulement sur les autoroutes, la compagnie de conteneurs, CMA CGM, offre de son côté une ristourne 500 euros sur les contenus de conteneurs de l'Asie vers la France, à partir d'août et ce pour un an, entre-temps, nous apprenons que le PDG de cette compagnie mais ce Rodolphe Saadé figure désormais à la 5ème place du classement annuel des grandes fortunes, publié par le magazine challenges grâce à une augmentation de sa fortune de plus de 30 milliards d'euros, la source de ces énormes profits n'est pas, on le sait dans l'invention d'un produit révolutionnaire, l'entreprise bénéficie simplement d'une situation anormale hors marché de pénurie et nous devrions nous interdit de taxer ses superprofits ce projet de loi de finances rectificative c'est le gras pour les uns, et quelques miettes pour l'immense majorité des autres, notre société est fracturé, nous l'avons dit et pour combattre le cancer des inégalités, vous prescrivez l'usage du paracétamol. Merci cher. Collègue, la parole est maintenant Madame Sylvie Vermeillet pour le groupe Union centriste pour cinq minutes. Monsieur Monsieur le président, monsieur le président du Sénat, messieurs les Ministres, Monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Le PLFR 2022 se destine à contenir la hausse des prix et protéger le pouvoir d'achat des ménages, le groupe Union centriste souscrit à cet objectif et proposera plusieurs mesures chaque fois ciblée car il a bien retenu, Monsieur le Ministre, Lemaire votre message d'il y a un an, la fin du quoi qu'il en coûte, et le soutien à ceux qui en ont besoin, il y a un mois, plus sombres, vous déclariez tout n'est pas possible, tout simplement parce que la France a atteint la cote d'alerte sur les finances publiques étant bien aussi inquiet que vous, nous sommes très déterminés car la dette est devenue très chère pour commencer : relever de 18 à 30 centimes la remise carburant ne nous paraît pas judicieux pour 5 raisons contrairement à ce que vous souhaitez la baisse ne cible personne et touchera tous les niveaux de revenus, elle bénéficiera même 2 fois plus aux plus aisés, comme le souligne justement le Conseil d'analyse économique, qui constate que les rabais sont des mesures inefficaces et coûteuses de non seulement elle bénéficie à tous les revenus en France, mais aussi, et c'est encore pire à tous les étrangers, touristes ou frontaliers comme le disent mes voisins suisses c'est l'État français qui paye lorsqu'on baisse un prix de 25 pour 100 le producteur en profite pour remonter son tarif IV, que se passera-t-il lorsque, dans quelques mois, le prix des carburants remontera de 50 centimes aurons-nous un nouvel épisode gilets jaunes et 10 milliards de dépenses à la clé le coût pour les finances publiques est inacceptable car la dette finance ainsi sans limites ni condition de ressources, ni condition de nationalité, c'est parfaitement contradictoire avec la fin du quoi qu'il en coûte à à la place de cette mesure dispendieuse, nous proposerons un amendement de Michel Canevet, prenant en charge une partie des frais de déplacement des personnes qui travaillent via l'employeur en contrepartie de réductions de charges patronales nous accordons les mêmes trente centimes de réduction, mais seulement à celles et ceux qui utilisent leur véhicule pour travailler, toujours soucieux des finances publiques, nous proposerons une contribution exceptionnelle sur les bénéfices de l'année 2021, je sais, Monsieur le Ministre, que vous n'y êtes pas favorable puisque vous réduisez vous réduisez les propositions des sénateurs à des réflexes pavloviens. Mais les chiens de garde du Parlement que nous sommes veille pourtant sur la nation avec un esprit de justice fiscale et sociale. Vous-même, monsieur le Ministre, attaché à taxer les GAFA déclariez en décembre 2018 il n'y a pas de succès économique sans justice sociale, alors nous proposons que l'État joue son rôle de régulateur en atténuant les effets des crises auprès de tous par ailleurs ce réflexe pavlovien, le gouvernement ne l'a-t-il pas eu en 2020 lorsqu'il a décidé d'une taxe de solidarité exceptionnel sur les primes des organismes complémentaires de santé afin, je cite, de compenser les profits générés par les mutuelles pendant la crise sanitaire, y a-t-il eu débat sur l'opportunité, non c'était pure justice sociale, mettre en place un prélèvement exceptionnel parce qu'il y avait enrichissement exceptionnel liés à la crise Covid était juste, nous voulons la même chose concernant les sociétés qui voient leurs profits bondir à l'occasion d'une nouvelle crise nos voisins le font l'Italie, l'Espagne, la Roumanie, la Grèce et même le Royaume-Uni, les Allemands ne devrait pas tarder, nous avons accepté de baisser l'impôt sur les sociétés, nous pensons juste de prélever une contribution exceptionnelle parce que la situation est exceptionnelle, le président de la République disait il y a quelques mois, pour moi, la justice sociale, c'est de prévenir les les inégalités, hé bien nous y sommes, nous proposons par ailleurs le report d'un an de la suppression de la contribution audiovisuel public parce que le sujet mérite concertation et que cela n'a pas eu lieu bien sûr le mécanisme de la CRP est obsolète, bien sûr, il s'agit d'une promesse du président de la République, c'est pourquoi nous, nous ne nous opposerons pas à sa suppression, mais pour une fois, prenons le temps de penser à tout et à tous pour permettre de mettre en place un dispositif satisfaisant Le monde de la culture, au passage, nous économiserons 3 virgule 7 milliards qui ne feront pas de mal aux intérêts de notre dette, enfin dans le droit fil de votre judicieux bouclier tarifaire énergétique, Françoise Gatel, présidente de la délégation aux collectivités proposera une aide pour les communes qui voient leur facture énergétique s'envoler sans ressources supplémentaires ainsi qu'Hervé Maurey le dispositif voté par l'Assemblée nationale est trop restrictif car les bases de compensation liée à l'évolution de l'épargne brute exclurons trop de communes aux difficultés multiples voici donc, messieurs les Ministres, chers collègues, la ligne directrice du groupe Union centriste particulièrement attentive à l'usage que nous allons faire de la dette publique, je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est maintenant au président Jean-Claude Requier pour le groupe du Rassemblement démocratique social européen pour cinq minutes, vous avez la parole monsieur le président.

comportant particulier toute la rallonge budgétaire attendu pendant compatriotes après le projet de loi que nous avons gamine et la semaine dernière dans des délais pratiquement comme nous faisons pas d'illusions, le la situation budgétaire de l'État est difficile après 2 ans de pandémie de politique quoi qu'il en coûte, qui a permis de maintenir à flot notre économie au prix d'un bond historique de l'endettement, nous sommes désormais confrontés à un retour de l'inflation causée à la fois par les effets du déconfinement de l'économie par les multiples difficultés d'approvisionnement une hausse historique des prix du transport de containers à l'échelle internationale des tensions sur l'importation de certains produits et en fait un affaiblissement de l'Euro par rapport au dollar liée aux conséquences économiques de la guerre, l'Ukraine et les sanctions qui a fait, qui est plus dur au monde, les Européens que les Américains. La faiblesse de l'Euro renchérit donc automatiquement le prix des ressources libellés dans la main de monnaie américaine le pétrole en particulier, une situation politique nationale et complexe depuis quelques semaines à la réaction du président de la République en avril dernier, une première depuis l'instauration du quinquennat a débouché sur un résultat paradoxal : l'initiative qui permet à certains groupes d'opposition de se prétendre de venir les faiseurs de politique au moment même où notre pays aurait besoin de décider, responsable et lucide, le spectacle parfois ubuesque de l'examen du projet de loi, pouvoir d'achat et de ce PLFR par l'Assemblée nationale on certainement laissé perplexe, beaucoup de nos concitoyens, quant à l'esprit de sérieux de quelques-uns des membres de la représentation nationale, ce n'est pas ici que le Kosovo, la politique, pour ce qui concerne les mesures de ce PLFR notre groupe continuera de chérir sa liberté de vote, ce qui veut dire qu'on n'est pas toujours d'accord tous par exemple sur des mesures aussi importantes que la suppression de la contribution à l'audiovisuel public l'adressé à cet impôt spécifique sont connus, bien que la question du financement soit essentielle, nous verrons dans les prochaines guerre si budgétaire à ce qu'qui soit assurés à la hauteur de ce que les un audiovisuel public de qualité et de la société, mais surtout sur de l'occasion de débattre de ce que doit être, pour un véritable service public, les problèmes de qualité, les rapports entre elle n'est pas, et puis l'arrivisme Arsène de renforcer l'attachement des Français alors audiovisuel commun pour le reste, ce texte comporte des mesures techniques, comme la généralisation de la facturation électronique et des transactions entre assujettis à TVA ou encore des rectifications du décret en particulier le décret d'avoir de quelque 7 milliards d'euros, adopté au printemps pendant la période électorale la poursuite et l'élargissement du Champ des PGE il lui sa difficulté à sortir concrètement un dispositif conçu d'abord comme temporaire, mais largement plébiscité par les acteurs économiques qui souhaiterait que ça continue, Arjen c'est tellement beau de mesure consiste à renforcer le soutien d'organismes internationaux à l'Ukraine, j'ai salue pour ma part la majoration de l'Arctique 14 la dotation Paul Titres sécurisés car on connaît les difficultés rencontrées actuellement par les collectivités pour le traite les renouvellements des demandes de de cardio entités et de passeports des compensations en faveur des collectivités ont été votées : assemblée pour faire face à la revalorisation des points, des fonctionnaires et du RSA, nous proposerons des amendements visant à aller plus loin dans le sens que quand elle nous semble pas suffisamment suffisamment nous proposera également de territorialité davantage certaines aides, en particulier pour ce qui concerne la lutte contre la hausse du prix des carburants,

Merci monsieur le président, non, non, pas du tout, il vous restez 20 secondes hé oui. Merci en tout cas pour votre humour le la parole est maintenant monsieur Rémi Féraud, pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour cinq minutes. Monsieur le président, monsieur le président du Sénat, messieurs les Ministres, Monsieur le président de la commission des finances, et monsieur le rapporteur général, chers collègues, ce projet de loi de finances rectificative comme le texte que nous venons de voter sur le pouvoir d'achat, il se définit par ce qu'il y a dedans les ministres l'ont rappelé, mais aussi et peut être surtout par ce qui ne contient pas sur le pouvoir d'achat, le grand absent, c'était ainsi la revalorisation des salaires et dans ce PLFR le grand absent, c'est la contribution du capital et de ceux qui le détiennent mais il y a une nouvelle situation politique qui permet de vraies avancées au Parlement, cela a été le cas à l'Assemblée nationale pour les collectivités locales et face à l'urgence territoriale, nous espérons bien conservé, voire amplifié les avancées obtenues sur ce point, c'est même le rôle du Sénat. Nous avons aussi je crois, le devoir de faire un pas vers plus de justice fiscale et donc vers une participation des grandes entreprises et des plus fortunés à l'effort du pays, nous ne voulions pas vous décevoir monsieur le Ministre, j'ai compris que nous n'étions d'ailleurs à gauche, pas les seuls à le dire, que cela allait bien au-delà et le gouvernement est aujourd'hui sur la défensive, donc chers collègues, ayons de l'audace, bien sûr, nous pensons indispensable la création d'un ISF climatique dont les recettes pourraient aller vers des mesures plus solidaire de Transition énergétique des recettes qui permettrait d'augmenter le pouvoir d'achat à la hauteur de l'inflation sans entamer le reste à vivre des plus modestes, comme c'est le cas avec les mesures trop limité aujourd'hui et sans toucher au temps de travail, comme le gouvernement s'apprête à le faire avec le concours de la droite, par ailleurs, tout conduit à mettre en place une taxe EPSI exceptionnel sur les superprofits des grandes sociétés de l'énergie et des transports, cette mesure, elle est tellement légitime qu'elle s'est invitée jusqu'au sein de la majorité présidentielle, d'autant que les ressources ne manquent pas quand on voit les bénéfices records annoncés notamment par Total énergies et par la CMA CGM, alors messieurs les Ministres, renoncer au discours de l'impuissance, celui qui se contente de faire appel au bon vouloir des entreprises car ce faux-semblant ne trompe plus personne, regardez l'état de nos services publics et l'explosion des inégalités, rappelez-vous la crise des gilets jaunes, elle n'est pas si ancienne, vous noterez que nos propositions, elles sont très bénéfiques pour les finances publiques, puisqu'elle dégage au total près de 25 milliards d'euros de recettes et je crois qu'il est temps d'ajouter oh combien ça coûte le combien ça rapporte sinon en s'obstinant dans son refus le gouvernement démontrerait qu'il n'est pas celui de la maîtrise des finances publiques, mais aussi celui du déficit, regardez ce qui se passe chez nos voisins européens, un effort bien plus conséquents sur les transports publics, comme en Allemagne ou en Espagne, qui devrait nous servir d'exemple et dans ces 2 pays comme en Italie et au Royaume-Uni, une taxe sur les superprofits voit le jour, cela n'a rien à voir avec le niveau de fiscalité générale sur nos entreprises, alors vous voyez c'est nécessaire et c'est possible et ne ratons pas cette occasion enfin et je conclurai par là ce qui manque au texte mais si, messieurs les Ministres, à votre texte cette un outil de préservation de notre démocratie car fragiliser le service public de l'audiovisuel, aujourd'hui, c'est une erreur, et même une faute, c'est pourquoi nous proposerons une nouvelle forme de redevance audiovisuelle en revenant sur sa suppression pure et simple, présenté à tort comme une mesure de pouvoir d'achat, c'est un enjeu essentiel pour notre démocratie, la qualité, l'indépendance de l'information, la création culturelle, le système que nous proposons, il est plus juste et progressif que l'actuelle redevance mais surtout. Contrairement aux vôtres qui relève de l'improvisation et qui, avec la TVA reprend d'une main ce qu'il a fait semblant de donner de l'autre, notre nouvelle contribution elle elle préserve vraiment le financement le financement spécifique et l'indépendance de l'audiovisuel public ces dernières semaines, des voix se sont levées de plus en plus nombreuses pour dire que sa suppression était une fausse bonne idée, alors quand il s'agit de taxer les superprofits, il serait urgent d'attendre et là pour supprimer un outil démocratique précieux, il n'y aurait pas une minute à perdre, soyons sérieux et chers collègues, au-delà même des clivages partisans, prenons nos responsabilités, je vous remercie. vous avez la parole cher collègue. le texte que nous avons examinons cet après-midi, a fait l'objet d'importants compromis tout au long de sa discussion à l'Assemblée nationale et été adopté il y a plus de 6 jours à une très large majorité par nos collègues députés, je vous parle d'une très large majorité, car la majorité absolue des votants était dépassée de 73 voix, c'est une victoire considérable pour la démocratie, compte tenu de la nouvelle configuration politique, la députée Véronique Louwagie souligné notamment le souhait du groupe, les républicains d'incarner une opposition raisonnables, je ne peux qu'espérer que cet état d'esprit préside également à nos débats je ne doute pas, mes chers collègues, que le Sénat sera fait, faire preuve de responsabilité et trouver les mêmes voies constructive que nos collègues députés. Qu'il remplira avec sagesse et une nouvelle fois son rôle de chambre de compromis, c'est une responsabilité d'autant plus grande que. Ce collectif budgétaire est le corollaire indispensable du texte de pouvoir d'achat que nous avons adopté vendredi dernier à la tombée de la nuit et je crois profondément que nous serons trouver une issue raisonnable en CMP sur le texte, pouvoir d'achat dès ce soir, comme nous le ferons au cours de la semaine sur ce budget rectificatif qui nous est soumis, cet esprit de compromis, le gouvernement, on a fait la preuve puisque, jusqu'à la fin de l'examen en séance publique, à la faveur à la faveur, pardon, d'un amendement proposant d'aider les ménages se chauffant au fioul, vous l'avez rappelé monsieur le Ministre, ce sont 230 millions d'euros, qui d'ici l'hiver aideront nos concitoyens, a passé le retour du froid sans subir de plein fouet la flambée des coûts de l'énergie. Cet esprit de compromis, le groupe pays en prendra également sa part en rejoignant l'initiative de notre rapporteur général de de pérenniser le nouveau plafond d'exonération des heures supplémentaires, monsieur le rapporteur général, votre amendement nous paraît une aide bienvenue à l'emploi quand la prospérité de notre économie et la soutenabilité de nos finances publiques repose en grande partie sur le dynamisme du marché du travail et la productivité de nos entreprises. Cet esprit de compromis, enfin, nous l'avons vu à à l'oeuvre sur un sujet qui nous préoccupe tout particulièrement ici au Sénat, je veux bien entendu parler des collectivités locales. Nous n'oublions pas tout ce qui a été fait depuis 2017 avec une capacité de d'autofinancement brute qui s'est envolée de 23,2 % sur le quinquennat une trésorerie en hausse de 36,4 % des dépenses réelles d'investissements qui ont augmenté de 14,9 %. Tout cela grâce aux mesures inédites de soutien et de compensation dynamique que nous avons mis en place, je n'oublie pas également le dynamisme. Mais d'un grand nombre de recettes fiscales des collectivités, les diamants, la TVA, dont une large part revient. La taxe foncière et j'en passe. Mais en particulier pour le bloc communal, il demeure d'importantes disparités et certains de nos communes ont besoin d'un soutien exceptionnel, c'est pour cela qu'un groupe compromis a été trouvé. Autour du rapporteur général Jean-René Cazeneuve, dont je salue le travail. Il a permis de mettre en place une dotation exceptionnelle pour les communes les plus touchées par la hausse des coûts, nous avons là encore des propositions à faire valoir pour améliorer le dispositif, mais je ne doute pas que nous trouverons tous ensemble et avec le gouvernement, les mesures adaptées pour protéger nos communes menacées par l'envol du coût de l'énergie. Nos collègues ultramarins du groupe RDPI pays. Sont nombreux à saluer les avancées obtenues en première lecture, notamment l'enveloppe exceptionnelle d'aide alimentaire ouverte pour lutter contre la vie chère. Je sais, Monsieur le Ministre, comme vous l'avez fait auparavant, vous regarderez avec bienveillance, notre amendement. Prévoit de l'élargir aux collectivités d'outre-mer, c'est un enjeu de solidarité mais aussi d'égalité, de justice pour la Polynésie française, la Nouvelle Calédonie et l'ensemble des collectivités d'outre-mer, je sais que vous y êtes sensible, monsieur le Ministre, je n'oublie pas votre réaction suite à m'associer sollicitations dernier projet de loi de finances pour aider Air Tahiti Nui alors en grande difficulté, merci monsieur Lemaire. J'ajoute enfin que je partage avec nos amis ultramarins et ma collègue finistérienne Nadège avait le soulagement que constitue la prolongation de l'aide aux carburants pour les pêcheurs, annoncé vendredi dernier par le secrétaire d'État en charge de la mer, c'est une mesure juste qui viendra en aide à un secteur fortement touché par le retour de l'inflation, alors oui, mes chers collègues, comme le disait notre collègue député Mathieu Lefèvre, je suis heureux que nous puissions discuter d'un texte qui revalorise revalorisera les pensions 60 euros par mois qui fera en sorte que les prix du gaz et l'électricité, les Français n'augmenteront pas de 4 % et de 35 % comme cela aurait été le cas, si nous n'avions rien fait. Car notre pays connaît malgré son niveau l'inflation la plus modérée d'Europe, nos voisins enregistre quand certains de nos voisins, enregistre une baisse au 2ème trimestre un taux de chômage historiquement bas à 7,3 %. Ce sont les fruits de la constance de notre politique économique et des mesures de pouvoir d'achat engagées dès le début de la crise. Mes chers collègues, vous connaissez l'expression : il ne faut pas changer de cheval au milieu du gué je pense en particulier au débat que nous aurons sur la taxe exceptionnelle que certains veulent mettre en place, il en va de la confiance dans notre politique économique, de la clarté, de la cohérence de notre modèle fiscal, le gouvernement a demandé aux entreprises des engagements. Nous, souvent être au rendez vous des résultats et sanctionner ceux qui ne devra l'être quand le temps sera venu de demander des comptes. Mais ne pénaliseront pas la reprise alors que notre économie sort tout juste de la crise. Avec ce texte, ce sont 20 milliards d'euros qui seront rendus à nos concitoyens. C'est un grand moment de démocratie parlementaire et ce sera de nos votes que nous devrons répondre quand il faudra dire si oui ou non, nous avons été à la hauteur des enjeux, je vous remercie de votre attention. Merci, cher collègue, la parole est maintenant Madame Vanina. Paoli-Gagin pour le groupe, les indépendants républiques et territoires pour cinq minutes. Monsieur le président, messieurs les Ministres, Monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, tous les marins le savent, la navigation est un art de l'anticipation, le Capitaine d'un grand paquebot doit ainsi attendre 30 minutes entre son coup de barre et son effet sur la trajectoire du navire pour redresser les finances publiques, l'inertie et bien évidemment plus longue, c'est en années sinon en décennies que se résorbe les déficits chroniques et les dettes abyssales alors si ce budget marque la fin du quoi qu'il en coûte, ces effets ne se feront malheureusement pas sentir avant des années Monsieur le Ministre, aujourd'hui, la situation de nos finances publiques et, bien évidemment, tout le monde le sait alarmante, encore une fois, elle est par les décisions que nous avons prises collectivement, notamment au plus fort de la crise pour préserver nos emplois sauvegardés, nos entreprises protéger nos concitoyens notre dette publique est supérieur de plus de 15 points de PIB à celle de 2019 niveau qui nous préoccupait déjà à juste titre, pourtant nous vivons sous anesthésie générale, le contexte des taux négatifs rendait cette dynamique d'endettement finalement artificiellement assez indolore, la charge de la dette ne cessait de diminuer alors que la dette elle-même, de cesser d'augmenter, désormais, la charge augmente dangereusement nous oblige à cibler nos mesures à prioriser nos urgences en l'occurrence l'urgence et sociale, l'inflation qui frappe tout le pays touche plus durement les plus fragiles, le taux moyen qu'il soit à 5 ou 6 % peut en fait correspondre à une augmentation du coût de la vie de près de 10 c'est toute l'injustice de la situation en souffrent davantage de la hausse des prix de l'énergie, de l'alimentation quand on vit dans l'hétéro ridoirs euros avec des revenus modestes, c'est pourquoi le ciblage des mesures sur le coût de l'énergie, et ce pour les plus modestes fait sens l'hiver arrivera vite si l'inflation persiste, elle reste pour le moment, inférieur à la moyenne européenne, c'est en partie grâce à la réactivité du gouvernement, en partie grâce à notre moindre dépendance au gaz russe, mais il n'est pas impossible qu'elle nous frappe par effet retard, il faut donc être clair le budget rectificatif que nous allons examiner n'est pas un budget de rétablissement des comptes publics, il répond à l'urgence de la situation avec un souci d'efficience que chacun appréciera, nous aurons prochainement l'occasion de discuter des grandes orientations budgétaires, nous devons les prendre en responsabilité, en gardant à l'esprit le fait que le spectre de la récession guette notre pays, comme la zone Euro, pour l'heure, j'espère que nous saurons créer des consensus pour protéger le pouvoir d'achat des Français, singulièrement celui des plus modestes dans les territoires ruraux, le projet de loi, pouvoir d'achat a montré que nous en étions tous ensemble capable j'identifie, pour ma part trois sujets épineux, au fond, je crois que nous sommes plutôt d'accord, mais devons-nous répondre à une question de justice fiscale. Qui doit supporter le coût des mesures que nous voterons le 1er sujet : c'est bien sûr la contribution à l'audiovisuel public sa suppression ne fait pas débat la question a été tranchée à la présidentielle, les Français ont choisi au 1er tour de candidats qui supprimait cette taxe, elle n'a plus de sens à une époque où l'audiovisuel passe essentiellement par Internet, mais comment garantir le financement notre audiovisuel public en supprimant une taxe injuste pour les Français et inadapté à la réalité économique du secteur, fraction de TVA ne me paraît pas optimale car ce mode de financement n'est ni stable ni pérenne, son seul mérite est d'être opérantes à court terme, pour ma part, je pense qu'il faut faire contribuer davantage les géants du numérique qui ont changé la donne et je vous proposerai un amendement en ce sens qui pourrait amorcer une nouvelle voie de réflexion, le 2ème sujet épineux, c'est la taxation des superprofits, c'est sans doute un réflexe bien français que de répondre à une crise, par une taxe pourtant d'autres pays, dont le Royaume Uni et l'Espagne se sont empressés de copier notre grand remède nationale. Mais même si la tentation est grande notre réponse doit à mon sens plutôt être le fruit d'une réflexion objective. Multisectoriels, le cas échéant, enfin, sur le dernier sujet épineux, c'est la compensation par l'État des surcoûts supportés par les collectivités, le débat a déjà eu lieu à l'Assemblée, nous l'aurons ici car nous pensons, nous portons tous une attention particulière aux collectivités locales et nous proposerons avec les indépendants des amendements en ce sens sur l'impact de la revalorisation du point d'indice pour la fonction publique territoriale, je veux être clair : la compensation par l'État ne crée pas de dépense publique supplémentaire, il y a bien une hausse de dépenses, mais elle a été décidée par décret, il faut maintenant dire : qui paiera, je crois que l'effort doit être partagé entre les collectivités et l'État qui a déjà beaucoup fait, mais soyons lucides, en matière de finances publiques, c'est toujours le contribuable qui paie in fine et en matière de vote au sein du groupe, les indépendants, République et Territoires, c'est toujours le votants qui choisit, je vous remercie. Merci. Merci de cette conclusion et je donne maintenant la parole à Monsieur Vincent ce goût pour le groupe Les Républicains pour 9 minutes.

Monsieur le président, messieurs les Ministres, Monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Mon pronostic. Ce 1er budget du second quinquennat d'Emmanuel Macron s'inscrit dans un contexte particulier, tant sur le fond que sur la forme, sur le fond, nous vivons une période de hausse de l'inflation sans précédent depuis des années 80 qui met à mal notre économie et aussi le pouvoir d'achat des Français. La crise actuelle fait suite à la guerre en Ukraine à la crise énergétique mais aussi à la crise économique sans précédent que nous avons traversée suite aux périodes de confinement lié à la pandémie sur la forme, maintenant ce collectif budgétaire va avancer dans un contexte politique inédit avec une majorité relative à l'Assemblée nationale, ce qui permet au président de la République de découvrir au bout de 5 ans, ce qu'est la démocratie représentative, le Parlement revient au centre du jeu place qui n'aurait jamais dû quitter et nous nous en félicitons. Le contexte et donc singulier et appelle pour ces 2 raisons de fond et de forme à la plus grande responsabilité de notre part, notre groupe au Sénat n'a cessé depuis 50 de mener une opposition constructive au gouvernement mus par le seul sens de l'intérêt de la France. Dans le nouvel équilibre politique actuel, notre responsabilité dans l'opposition et de convaincre le gouvernement du bien fondé de nos propositions, notre pays ne peut plus se permettre de perdre encore 5 ans sinon il sera sans doute trop tard le contexte d'argent magique et d'argent soit disant gratuit a également changé. Le retour de l'inflation contraint des banques centrales et des institutions monétaires à réagir la semaine dernière, la Réserve fédérale américaine a décidé une nouvelle hausse du taux exceptionnel de 0 75 comme le mois dernier, qui constituait déjà un record depuis 1994 au total, la Fed a relevé son taux directeur de de 25 % depuis le début de l'année, la semaine dernière également, la BCE pour la première fois depuis 11 ans, a relevé son principal taux de 0,5 cela conduit à un relèvement des taux d'intérêt, les taux des USA 10 ans ont dépassé les 3 % en mai et les OAT 10 ans qui nous concerne, ont largement dépassé les 2 % en juin je rappelle juste qu'ils étaient encore négatif au mois de décembre. Aujourd'hui, nous sommes entre 1 50 et 1 virgule 60 % mais je rappelle que, selon l'Agence France Trésor 1 point de taux d'intérêt, c'est de 5 milliards d'euros de charges de la dette en plus et, selon la Banque de France, 40 milliards d'euros par an au bout de 10 ans. à cela s'ajoute l'effet de la hausse de l'inflation sur laquelle 10 % de notre dette est indexé là encore un point d'inflexion, en plus, c'est encore de 5 milliards d'euros de charges de la dette en plus l'intérêt de la dette était depuis de nombreuses années le 3ème poste de défense de l'État après l'enseignement scolaire et la défense, elle est passée de 38 milliards à 51 milliards en un an, elle vient aussi dépassé le budget de la défense et ce, à un rythme, elle pourrait devenir dans peu de temps, le 1er budget de l'État imaginer tout ce que nous pourrions faire avec ces 50 milliards d'euros pour le pouvoir d'achat des Français là et la compétitivité de nos entreprises. Le gouverneur de la Banque de France vient de mettre en garde le gouvernement qu'il, je le cite, illusoire de penser que notre dette encore sans coup et sans limite, il juge que la France ne peut pas se permettre de transmettre un tel poids de dettes à sa jeunesse. Le Haut Conseil des finances publiques, estime pour sa part que notre endettement est un point de vulnérabilité, il y a un mois, monsieur le Ministre de l'Économie et des Finances semblait découvrir le problème en estimant que nous avons atteint le code d'alerte sur nos finances publiques, alors même que, 4 mois plus tôt, il déclaré, je le cite, contrairement à ce que disent tous les Cassandre pour la campagne électorale, l'économie française se porte très bien. Ce n'est pourtant pas faute durant le précédent quinquennat de n'avoir cessé au Sénat, de mettre en garde le gouvernement contre une remontée des taux d'intérêt et nous avons insisté sur la nécessité de réaliser des économies et des réformes structurelles. Comment en sommes-nous arrivés là les différentes crises n'explique pas tout, autant il était nécessaire de soutenir et relancer notre économie durant cette période et nous l'avons approuvé. Autant le quoi qu'il en coûte, a été générale et a couvert les dépenses qui n'avait rien à voir avec la crise. Hausse des dépenses, absence d'économie, la diminution de 50000 postes dans la fonction publique d'État, a été abandonné lors du précédent quinquennat comme la réforme des retraites, alors qu'il s'agissait de promesses de notes du candidat Macron. Il nous promet que la réforme des retraites se fera lors de ce nouveau quinquennat devons-nous le croire, la réforme a déjà été repoussée d'un an à l'été 2023 alors que nous savons très bien que les réformes les plus difficiles doivent être engagés dès la première année. C'est la raison pour laquelle nous proposerons dans ce collectif budgétaire que la mise en place de la carte Vitale biométrique se fasse sans attendre, nous n'avons pas besoin d'une mission parlementaire supplémentaire pour savoir que cela engendrera des économies, les économies sont nécessaires pour financer les dépenses, celles-ci ne doivent pas être financée par le surcroît des recettes, comme l'a très bien dit la Cour des comptes, les recettes imprévues doivent aller au désendettement de notre pays, or toutes les dépenses de ce PLFR sont financés par la hausse des recettes qui est d'ailleurs en grande partie, dit à la hausse de l'inflation. Ce n'est pas sain, surtout quand vos prévisions de recettes sont basées sur une croissance que nous jugeons comme le Haut conseil des finances publiques surestimé. La croissance française pâtit en réalité d'une vraie pénurie de main-d'oeuvre dans de nombreux secteurs, le taux de chômage en France demeure bien plus élevé que la moyenne européenne, selon les derniers chiffres en mai 2021, nous sommes à 7,2 pour 100 de virgule huit % en Allemagne et les États-Unis à 3, c'est la raison pour laquelle il faut permettre d'aider de manière durable, les entreprises à maintenir un niveau d'activité suffisant face aux problèmes de recrutement auxquels elles sont confrontées chaque jour, c'est notamment dans ce sens que nous proposons de pérenniser la hausse la défiscalisation et de la désocialisation des heures supplémentaires. Le travail doit être encouragé, valorisé, c'est une valeur essentielle à nos yeux, dans le même esprit, nous proposons que le rachat des RTT soit pérennisé, mais également que la prime de rentrée cible : les travailleurs pauvres plutôt que les bénéficiaires des minima sociaux qui ne travaille pas. Ce sont aussi des mesures de pouvoir d'achat qui a, celui-ci se gagne avant tout par le travail, nous nous félicitons que d'importantes mesures proposées par les députés des républicains était adopté à l'Assemblée nationale sur le travail, j'ai cité le rachat possible de RTT, la hausse de 5000 à 7500 euros du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires. Même si à titre personnel, je serais plutôt pour un déplafonnement total mais nous y reviendrons pour faire face à la crise énergétique qui impacte fortement le pouvoir d'achat de beaucoup de Français, notamment dans les territoires ruraux, nous nous félicitons de l'accord trouvé de remise de 30 centimes du prix à la pompe, mais aussi de l'adoption de nos mesures de soutien des petites stations services situées dans les zones rurales et des particuliers qui se chauffent au fioul, qui avaient été les grands oubliés du dispositif initial, le filet de sécurité pour les collectivités territoriales adoptée de manière concertée par les députés pour faire face à la hausse de leur facture énergétique et du coup du point d'indice est un 1er pas nous proposerons de l'améliorer notre groupe vous annonce d'ores et déjà Monsieur le Ministre, que nous demanderons l'indexation de la DGF dans le PNF de 2023 enfin, le vote final des républicains de ce budget rectificatif dépendra de l'écoute que vous voudrez bien nous accorder des propositions que vous accepterez, il en va de l'intérêt de notre pays, je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Monsieur Daniel Breuiller pour le groupe écologiste Solidarité territoire pour cinq minutes. Monsieur le président, monsieur le président du Sénat, messieurs les monsieur le Ministre. Monsieur le rapporteur général, monsieur le président de la commission des finances, chers collègues, monsieur le Ministre. Vous décrivez le contexte avec beaucoup de gravité, j'ajouterai d'ailleurs car vous n'évoquait que timidement à la guerre en Ukraine à la dette à l'inflation, la grave crise climatique et son corollaire, l'exigence de la transition écologique. Faire le point est indispensable, mais ce serait inutile si ensuite nous ne choisissons pas le bon cap et quelle est votre cap Monsieur le Ministre, sur la dette 20 milliards supplémentaires porte le déficit public annuel à 177 milliards justifiant le terme de cote d'alerte, mais si cette cote d'alerte est atteinte pourquoi renforcer ce déficit de plus de 3 milliards en supprimant la contribution à l'audiovisuel public pour le pouvoir d'achat des Français taxer les plateformes bloquer les prix des loyers et là vous allègerait le coût de la vie de nos concitoyens sur tous les bancs de notre assemblée des voix demandent que l'enjeu de l'audiovisuel public ne soit pas au détour d'une décision mal préparée d'un article du PLFR dans une société de défiance et de fait que News, les questions d'indépendance et de fiabilité de l'information sont essentiels, comme celle du soutien à la création aux artistes d'innovation, d'éducation, qui sont portés avec exigence par notre service public de l'audiovisuel, ces questions ne se règle pas sans prendre le temps d'un débat avec la représentation nationale avec les professionnels et les usagers, changer de cap, Monsieur le Ministre, plutôt que de supprimer rapidement cette C A P pour la dette encore vous nous expliquez qu'il ne faut pas taxer les superprofits taxer les superprofits de mots que vous récusez mais d'autres pays le font en Europe 18 milliards pour Total est un geste à 500 millions n'est-ce pas le retour de la charité plutôt que le choix de la solidarité et de l'impôt votre CAP, c'est moins d'impôts pour les grandes sociétés et des revenus désocialisées et défiscalisées pour les salariés, mais comme le disait Henry Morgenthau, les impôts sont le prix à payer pour une société civilisée convaincus de cela nous proposeront de taxer les superprofits et plus particulièrement les profiteurs de crise qui nourrissent d'ailleurs l'inflation en augmentant leurs marges, nous proposons aussi de créer un ISF climatique structuré sur Solidarité sociale et transition écologique, il permet la contribution des plus fortunés et ils en seront heureux dans les bilans carbone sont par ailleurs les plus désastreux, il n'est pas socialement acceptable de demander des efforts à nos concitoyens modestes au nom de la gravité de la situation et de constater que le CAC 40 distribue 57 milliards de dividendes record européen ou que les 500 plus riches d'entre nous voient leur Patrimoine, dépasser les 1000 milliards, ces chiffres sont vertigineux pour nos concitoyens, rien ne justifie qu'un éleveur laitier, un maraîcher qui fournit une grande enseigne gagne en moyenne 500 fois moins que le PDG de cette enseigne ou que dans les entreprises du CAC 40 des salaires varient de 1 à 300 entre patrons et salariés, rien ne justifie que la finance soit moins taxé que le travail, personne ne vaut 300 fois plus qu'un autre, et comme le disait le Président Macron notre pays tient tout entier sur ces hommes et ces femmes que nos économies reconnaisse et rémunère si mal, hé bien il est temps de mieux les reconnaître et de mieux les rémunérer, nous vous faisons une proposition simple : augmenter le SMIC à 1500 euros, soutenir les PME, TPE par un fonds de solidarité revalorisation revalorisé de 10 pour 100 le point d'indice des fonctionnaires et porter toutes les retraites et prestations service social inscrite à ce PLFR au niveau réel de l'inflation, un mot sur la guerre qui frappe le peuple ukrainien pour lequel nous re-exprimons notre solidarité et nous approuveront les mesures du PLFR. Nous mesurons les risques d'approvisionnement et nous mesurons surtout la profondeur de la crise énergétique, c'est le prix de notre inaction climatique passer cela appelle certes des mesures d'urgence, mais surtout d'engager le chemin de l'autonomie énergétique, mais là encore, quel est le cap remplacer la dépendance au gaz russe par une dépendance au gaz de schiste américain ce n'est pas acceptable seul cap possible et celui de la sobriété, alliée au développement rapide des renouvelables, nous proposons 10 milliards dans l'isolation thermique des logements plutôt que les 400 millions de ce PLFR pas seulement pour changer une chaudière, mais pour une véritables rénovation thermique des habitats, des locaux d'activité des équipements publics, enfin, sur le bouclier tarifaire, il doit être étendu aux collectivités, dont certaines sont contraintes de fermer leurs piscines quant aux citoyens, les 30 centimes de baisse uniforme sur les carburants vont aggraver le déficit public en dans les propriétaires de devaient suivez à partir en week-end du week-end à Saint-Jean-Cap-Ferrat avec subvention de l'État qui peut défendre ça, cette aide doit être réservé à nos concitoyens qui n'ont pas d'autre choix que la voiture pour se rendre au travail lorsque les forêts brûlent les glaciers disparaissent les départements sont en sécheresse et en restriction d'accès à l'eau, l'agriculture mise à mal, il faut un autre cap celui un cap fructueux pour nos pays, ses habitants et la planète, nous ferons des propositions en ce sens.

Monsieur le président. Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, le budget rectificatif dont nous allons débattre aujourd'hui et demain est le 1er de l'année 2022, il poursuit dans un environnement inflationniste qui se durcit, l'objectif de redonner du pouvoir d'achat aux Français, j'avais un objectif noble que tout le monde ne peut que partager sur ces bancs, ce qui semble consensuel également, mais qui ne devrait pas l'être, c'est le moyen de remplir cet objectif en l'occurrence le recours encore et toujours à la dépense publique, héritée de la pandémie de Covid le syndrome de l'argent magique a malheureusement anesthésier les réflexes de sagesse budgétaire qui aurait prévalu en d'autres temps, par rapport à la loi de finances initiale, les dépenses pilotable augmente de plus de 18 milliards d'euros, c'est colossal. Parent au plus pressé : nous avons collectivement abandonner toute réflexion de long terme quant aux conditions d'une prospérité retrouvée. Car le pouvoir d'achat ne se décrète pas, il n'est, il vient non pas de l'État, mais des gains de productivité de l'économie, la fuite en avant de la dépense publique a ceci de mortifère que ses conséquences néfastes et diffuse ne sont visibles que sur le temps long. Dans son essai, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas le célèbre économiste français Frédéric Bastiat distingué en ces termes le mauvais économiste du bon. L'un s'en tient à l'effet visible l'autre tient compte et de l'effet qu'on ne qu'on voit et de ce qu'il faut prévoir d'où il suit que le mauvais économiste poursuit un petite bien actuel, qui sera suivi d'un grand mal à venir, tandis que le vrai tu es une vraie économiste un grand bien à venir. Au risque d'un petit mal actuel en laissant filer la dépense publique et les déficits et donc en fin de compte, l'endettement du pays, je crains, mes chers collègues, que nous sacrifions ce grand bien à venir d'en parler, Bastia, quand les comptes sont dans le rouge, il faut à tout le moins dépensé efficacement séquences qui disait : quand on veut sortir du trou, il faut commencer par cesser de creuser, cibler en priorité les ménages les plus vulnérables et les territoires les plus affectées par l'inflation, en particulier les communes rurales et les territoires ultramarins, ce n'est pas la direction prise par ce budget rectificatif qui privilégie les mesures générales et à différencier aux mesures temporaires et ciblées, le groupe Union centriste et ma collègue Sylvie Vermeillet les abris brièvement exposé tout à l'heure, fera cette fois-ci encore. un certain nombre de propositions allons à Lyon sobriété budgétaire efficacité économique et justice sociale, je vous remercie.

Monsieur le président, messieurs les Ministres, Monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Disons-le franchement, une fois n'est pas coutume, ce projet de loi de finances rectificatif s'inscrit dans la droite ligne de la droite. à vous écouter, je peine à comprendre le procédé schizophrénie qui consiste à taxer d'irresponsables tout contradicteur qui prône une meilleure répartition de la richesse par la dépense publique. Car, Monsieur le Ministre, vous êtes tout sauf un bon gestionnaire, vous êtes, je le rappelle le ministre, qui a le plus dépensé ces dernières années. Bien sûr, je ne parle pas ici des aides légitimes qui ont été mises en place pour soutenir le pays durant la crise Covid. Je parle plutôt du creusement du déficit que vous opérez à l'aide de vos nombreuses et systémique, baisse d'impôts de production ou d'impôt sur les sociétés. Je ne dis rien de bien original, finalement, je ne fais que reprend les propos de la Cour des comptes, qui impute une partie de la dégradation des comptes publics à des mesures nouvelles qui ont réduit les prélèvements obligatoires. En effet, sur le quinquennat précédent, le taux de l'impôt sur les sociétés est passé de 33 3 à 25 %, soit 15 milliards d'euros par an dans le même temps, une partie des impôts de production pour 10 milliards d'euros par an a été réduite la suppression annoncée de la CVAE effective dès 2023 coûtera aux finances publiques 8 milliards d'euros s'ajoutant ainsi à la longue liste des aides venant conforter la politique de l'offre. Vous organisez volontairement l'attrition des finances publiques et, incidemment, vous creusez Tilmant, le déficit public et la dette. Ces 12 milliards d'euros supplémentaires qui sont inscrits dans ce budget pour faire face aux intérêts d'emprunt. C'est colossal. Vous avez affirmé : Monsieur le Ministre ne pas vouloir d'un compromis qui s'achètent à coups de milliards n'a compromis qui se finance au détriment de nos finances publiques. Il semblerait qu'avec ces baisses d'impôts, de production, vous ayez forger un compromis qui coûtent pourtant très cher à nos finances publiques. Le fait que ces impôts profitent aux grandes entreprises fondrait ils votre cécité je n'ose le croire, même si votre renoncement à taxer les superprofits certains profiteurs de guerre. Me laisse à penser qu'en matière de compromis, vous semblez souvent toujours au profit des mêmes. Car, tout comme le projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, ce premier PLFR s'inscrit dans la continuité de la politique économique menée ces dernières années une politique basée sur l'offre et qui profite au même. Ce PLFR est le corollaire de votre qui consiste à refuser de prendre toutes mesures de nature à augmenter les salaires. La semaine dernière. Lors de l'examen du PJD et le pouvoir d'achat et alors que je proposer avec mes avec mon groupe un Grenelle des salaires afin d'abord de d'aborder un partage de la richesse plus égal dans ce pays, vous avez balayé d'un revers de la main cette possibilité, c'est précisément parce que vous refusez toucher au salaire qu'il vous faut faire du bricolage fiscal afin de poser quelques rustines ça et la prime petit chèque baisses d'impôts. En cela, le triplement de la prime du plafond de la prime Macron 2000 à 3000 euros pour la grande majorité des entreprises, voire six mille euros dans certains cas ne trahit que trop bien cette fuite en avant, que vous avez engagé. le Ministre ce PLFR et la transcription fiscale des mesures prises dans le pouvoir dans le PJ a le pouvoir d'achat. Or, ce dernier est lacunaire et porte la lourde marque des dogmes qui animent la vie de nos finances publiques depuis 5 ans. Sans changement de cap clair et radicale, nous serons condamnés à traiter ce PLFR pour ce qu'il est, à savoir une loi de finances inégalitaire qui fait peser sur les mêmes l'obligation d'assainissement des comptes publics. Vous nous parliez de la nouvelle méthode en de compromis. Nous espérons que de compromis, il sera question durant l'examen de ce texte afin de remettre plus de justifie se cale dans ce pays. Merci, cher collègue. La parole est au dernier orateur inscrit monsieur Jean-Raymond Hugonet pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Monsieur le président, messieurs les Ministres, Monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, chers collègues, il y a quelques semaines, la commission de la culture et la commission des finances ont adopté conjointement ici au Sénat un rapport portant sur le financement de l'audiovisuel public. Ce rapport préparé avec mon collègue Roger Karoutchi a établi un état des lieux qui tient en 3 points : 1er constat la contribution à l'audiovisuel public cap qui lie le financement de l'audiovisuel public à la possession d'un poste de télévision est devenu un prélèvement insuffisant, injuste et fragile. De plus en plus de personnes renoncent à posséder un téléviseur et consomment des programmes publics sur d'autres supports par ailleurs la suppression de la taxe d'habitation funeste rend son recouvrement très coûteux, le remplacement de la cape et donc inévitables, il devait avoir lieu au cours du précédent quinquennat cela n'a malheureusement pas été le cas. Voilà. 2ème constat : on ne peut traiter séparément le financement de l'audiovisuel public de son organisation et de ses missions. Quel moyen pour quelle mission, quel spécificité pour l'audiovisuel public, traiter la seule question du remplacement de la Cap sans même ouvrir le débat sur la place de la publicité sur le service public, par exemple, illustre une absence de vision et d'ambition pour ce secteur, l'échec de la réforme de l'audiovisuel public en 2020, a fait perdre beaucoup de temps et rend d'autant plus impérative une réforme. 3ème constat face à l'émergence des grandes plateformes et au puissant regroupement de médias privés réunissant Télévision et radio, il est urgent pour l'audiovisuel public de concevoir une stratégie numérique commune, ce qui passe par un regroupement des moyens. L'échec de Salto et les performances limitées des rapprochements entre France Télévisions et Radio France ont mis en évidence la faiblesse de la stratégie des petits pas en inscrivant à la hâte, la réforme de la carte dans ce projet de loi de finances rectificative et en changeant complètement le dispositif à l'Assemblée nationale, le gouvernement n'a pas tiré toutes les conséquences du rapport sénatorial, on ne peut aborder la question de la cape sous le seul angle du pouvoir d'achat et si nous avons, avec Roger Karoutchi, pris acte de la volonté du président de la République de supprimer cet impôt à mains égard nous avons nous avons aussi mis en évidence la nécessité de prévoir des garanties sérieuses concernant le financement de l'audiovisuel public. L'enjeu est moins selon nous de prévenir d'hypothétiques régulation infra-annuelles que de définir de véritables perspectives pluriannuelles au service d'une stratégie. Je rappelle que si le précédent quinquennat a été marquée par l'échec de la réforme de l'audiovisuel public et a un déficit de vision, on ne peut que donner acte au gouvernement d'avoir respecté la trajectoire budgétaire quadriennal et même au-delà, si l'on tient compte des financements apportés pour financer les plans de départs, les travaux de la maison de la radio et de la musique ainsi que les coûts liés à la crise sanitaire. La question est donc moins de savoir s'il faut financer l'audiovisuel public par des dotations budgétaires ou une fraction de TVA que de connaître l'ambition du gouvernement pour les 5 années à venir. Quelle sera la trajectoire budgétaire de l'audiovisuel public inscrite dans les contrats d'objectifs et de moyens, est-il vrai que la signature des prochains comme est repoussée à la fin 2023, pourquoi le gouvernement a-t-il renoncé à créer une commission indépendante pour évaluer les besoins de l'audiovisuel public, comme le proposait le Sénat, voilà les vraies questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Il en est malheureusement de même concernant les missions et l'organisation de l'audiovisuel public français qui est le seul en Europe à être éparpillés entre autant d'acteurs aux moyens limités, le choix qui a été fait à l'Assemblée nationale de recourir à une fraction de TVA pour financer l'audiovisuel public présente à cet égard un Avantage puisque c'est une solution provisoire. Nous avons donc 2 ans pour mener à bien le chantier de la réforme de l'audiovisuel public français c'est pourquoi si nous pouvons adopter la réforme de la Cap telle qu'elle a été modifiée par les députés, puisqu'elle assure le financement de l'audiovisuel public, nous devrons conditionner notre soutien aux dispositions concernant l'audiovisuel public français du projet de loi de finances pour 2023 à la présentation par le gouvernement d'un calendrier précis d'une réforme globale de l'audiovisuel public qui devra porter à la fois sur le financement sur les missions sur l'organisation et sur la stratégie numérique parce qu'il y a urgence, nous devons rechercher ensemble les voies de d'un audiovisuel public plus efficace, plus innovant et plus moderne, nous sommes déterminés à faire aboutir cette réforme d'ici 2025, merci de votre attention.

Merci monsieur le président. Je voudrais juste répondre un certain nombre d'observation, je vais être rapide, il y a un débat qui va s'ouvrir sur l'audiovisuel, le public monsieur Gonnet de la rappeler sur les collectivités locales et leur financement sur le travail sur la maîtrise des finances publiques et je vois que sur tous les bancs de cette assemblée, il y a une véritable préoccupation sur les finances publiques, tant mieux, ce qui veut dire qu'il ne faut pas sortir de cette assemblée, avec des dépenses inconsidérées, à l'occasion de ce PLFR je propose que nous nous fixons comme objectif de sortir avec un déficit public maintenu à 5 % comme c'est le cas, que nous nous sommes fixés avec Gabriel Attal mais je voudrais juste faire quelques remarques sur cette fameuse question la taxation des superprofits puisque je crois que chaque intervenant a pris la parole sur le sujet pour répondre à quelques arguments qui vont justifier des amendements qui vont venir, première argument que j'ai entendu cela va rapporter de l'argent. Moi, je suis très sceptique. D'abord parce que cela rapportera ça ne pas tant que vous le croyez, j'ai entendu de milliards trois milliards 4 milliards mais encore faut-il qu'il y ait des super profits qui soit réalisés en France. Chacun sait que l'impôt dépend de d'établissement stable. Et qu'il faut qu'une entreprise et son établissement en France pour qu'elle puisse être taxés, or les profits dont vous parlez, les profits des compagnies pétrolières ou d'autres jeux font à l'extérieur de la France. Donc, on serait bien ennuyés si les Allemands, venez nous dire : vous avez été l'entreprise, elle est en France, elle fait des profits en France, elle fait des bénéfices, en France, on va les récupérer ses bénéfices récupérer ses profits et les taxer, on serait bien ennuyés ces entreprises américaines qui font des profits, en France, nos amis américains venait nous dire : mais nous avons récupéré les bénéfices et les profits qui ont été faits sur le territoire français, il y a un principe intangible de la fiscalité internationale c'est établissement stable, c'est bien ce qui nous a amené, je le dis au passage à soulever le problème, la taxation des gens du digital, car l'énorme difficulté des gens du digital et c'est plutôt à eux qu'il faudrait s'intéresser qu'à nos entreprises nationales, c'est que, non pas d'établissement stable en France, puisque leur activité et des intermédiés et qu'elle ne repose sur aucune présence physique, donc je vois là des profits qui dans le fond ne vont générer aucune recette fiscale pour le trésor public français. On me dit : augmenter les impôts, ça rapporte toujours plus au trésor public, je pense que nous avons apporté la preuve. Avec la baisse de l'impôt sur les sociétés du contraire quand vous baissez les impôts des entreprises. Les entreprises créer plus de richesses. Et l'imposition rapporte davantage, nous avons baissé l'impôt ces sociétés, je le dis à l'intervenant qui a pris la parole tout à l'heure en nous disant vous ruiner les comptes publics, en baissant les impôts mais c'est faux, pardon, les chiffres vous donne tort. Nous avons baissé la poche et les sociétés de 33 3 à 25 % en 5 ans et les recettes d'IS sont passés de 50 milliards à 57 milliards, c'est bien la preuve que quand on augmente les impôts, on baisse les recettes, on baisse la trappe trinité du pays, on baisse la capacité à créer des richesses, quand on baisse les impôts, en revanche, on crée plus de prospérité, plus d'emplois et plus de recettes fiscales pour la nation française, c'est bien pour cela que nous avons retenu cette voie là, je le redis liesse a baissé et ces recettes ont eux augmenté mais dans le fond, derrière, c'est toute une philosophie et ce qu'on veut produire plus de richesses pour pouvoir mieux les redistribuer où est-ce qu'on veut comme certains ici qui ont pris la parole systématiquement taxées reprendre faire contribuer avec des richesses qui sont de moins en moins nombreuses, des emplois qui sont de moins en moins nombreux, un chômage qui explose, des recettes sociales qui diminue et dans le fond un appauvrissement généralisé du pays, je suggère de continuer dans une autre voie qui essaie de la création de richesse, la prospérité et de la création de l'emploi. On me dit ensuite, mais d'autres états européens l'ont fait. Mais je veux bien vous citez l'Allemagne et l'Allemagne s'est bien gardé. D'imposer une taxe sur les superprofits de ces entreprises, la première économie européenne est précisément celle qui n'est pas tomber dans ce piège-là. Les gens peut dire on l'ont fait, la Grande Bretagne par exemple, qui est pourtant pays libéral mais l'énorme différence. C'est que la Grande Bretagne produit du pétrole sur son territoire, donc c'est normal qu'effectivement là y'cette production puisqu'il y a une production alors qu'en France on ne produit pas de pétrole, il est produit à l'étranger et je rappelle qu'en terme d'imposition. La France continue à avoir un taux de prélèvements obligatoires, malgré les efforts particulièrement louable de cette majorité qui à baisser massivement les impôts 52 milliards en 5 ans, mais malgré cette baisse là. Malgré cette baisse de 52 milliards d'impôts sur 5 ans, le taux de prélèvements obligatoires en France et de 47 5. En Italie, 43 en Allemagne de 41 en Grande Bretagne de 33,5 %. Donc je crois que la seule voie qui est responsable et raisonnable pour notre pays qui étaient accablés de taxes accablés d'impôts accablés de prélèvements obligatoires qui n'a eu sans cesse à la bouche que de récupérer des richesses au lieu de vouloir en produire, c'est de baisser les impôts de nos compatriotes et de nos entreprises et je ne démordrai pas de cette conviction là. L'ultime argument c'est de me dire : c'est juste. Ben non moi je ne trouve pas que ce soit juste d'imposer à travers vos amendements à toutes les entreprises de France et de Navarre, quelle que soit leur situation dès lors qu'elles font des profits une taxation supplémentaire, je ne trouve pas que ce soit juste, je pense que c'est inquiétant pour les entreprises, inquiétant pour les chefs d'entreprise inquiétant pour tous ceux qui créent des richesses dans nos pays et dans le fond, inquiétant pour nos compatriotes même qui savent parfaitement que l'on commence pas taxer les grandes entreprises et qu'on finit toujours par les taxes, eux-mêmes, c'est précisément ce que nous voulons éviter. Alors vous avez cité des grands auteurs et vous me dites que les impôts sont le prix à payer pour une société civilisée, merci les impôts, tu es vraiment le prix à payer pour une société civilisée, alors la France serait de toutes les nations du monde la plus civilisée de toute je pense qu'il nous reste un effort à faire. Très bien, allez, allez. Chacun va se calmer, je vous rappelle que nous avons maintenant 450 amendements. Faire donc pas à chaque fois allez. Tout le monde aura la parole dans le calme, allez. La discussion générale est Close, nous passons directement aux textes et j'ai d'abord l'article liminaire qui ne portent pas d'amendements, je mais voit cet article liminaire, qui est pour. La température. Qui s'abstient, il est adopté. Avant l'article 1er ah je suis saisi d'un amendement 322 qui le présente monsieur Savoldelli. Monsieur le président, mais messieurs les ministres, mes mes, mes chers collègues, cet amendement porte sur l'imposition, Monsieur le Ministre, Lemaire des multinationales en utilisant une clé de répartition du chiffre d'affaires, monsieur le Ministre, l'accord sur l'imposition sur les multinationales, je vous voyez, ça va être un terme très respectueux patine. Il devrait pas entrer en vigueur avant 2024. Toujours est-il que ça ne sera pas termine en 2000 24 à cette date, et l'impôt pourra être minorée de façon significative des salaires et des actifs corporels. Je passe rapidement sur la question quinze pour cent, c'est mieux que rien, nous dit-on, vous avez raison, aujourd'hui, on a rien. Mais aura-t-on quelque chose à l'avenir. Quelque 4 milliards d'euros, selon les estimations de Bercy peu au regard des 21 milliards belge 13 milliards allemand, vous avez fait référence à des des repères européen, allons-y 12 5 milliards pour l'Irlande. Plus, me direz-vous, que les pays du Sud complètement lésés par cet accord, 4 milliards en Afrique du Sud, ou 1 virgule 5 milliards pour le Brésil, une des raisons de la faiblesse des recettes tirées de cet accord, c'est la cible et vous le savez, Monsieur le Ministre, le pilier 1 ne ciblent que les entreprises qui réalisent que 20 milliards de chiffre d'affaires avec des marges de plus de 10 % et le pilier de concerne 7 à 8000 entreprises réalisant un chiffre d'affaires de plus de 750 millions. Et alors on allait voir ce qu'on allait voir, et la France va récupérer parents les bénéfices réalisés par Total en un trimestre, d'ailleurs, la justice fiscale viendra avec cet accord, et je crois que c'est certain, et alors là, il ne faut pas mentir dans franchement dans les termes les plus respectueux total fait 21 % de ses bénéfices en France. C'est pas délocaliser c'est pas irrationnel, ce n'est pas virtuel, c'est une réalité, donc il faut quand on a les mots de souveraineté, il faut appliquer aussi une souveraineté populaire fiscal et de justice sociale, Monsieur le Ministre, nous pensons que l'idée donc de se focaliser sur les bénéfices réalisés mondialement en attribuant à chacun de payer une quote-part du chiffre d'affaires réalisé en France est une excellente idée, une excellente idée est toutefois pourquoi pas commencer à partir d'un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, ce qui est notre proposition

le cas notre collègue je, il a dit que c'était une excellente idée, je vais donner un avis défavorable, parce que d'abord ça ne répond à aucune vraie logique économique et en plus c'est contraire aux cons sont fiscales qui sont conclus avec nos partenaires. au moins. Oui, mais ma vie, je serai plus brève dans mes réponses à, on est sur un sujet important, je rappelle que sur le pilier hein et le pilier de le seuil d'entrée dans la taxation digitale la taxation minimale à Liesse et 750 millions d'euros. Pas 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires 750 millions après moi je partage totalement votre ambition, je pense qu'elle est tout à fait louable, il est indispensable d'avoir un impôt minimum à l'impôt sur les sociétés, je suis d'accord ça patine, vous avez raison et je regrette que ça ait pris autant de temps, moi je souhaite maintenant que nous ayons une coopération renforcée dans un cadre européen pour contourner l'inacceptable le véto que la Hongrie a mise à la taxation minimale à l'impôt sur les sociétés, mais ça ne peut se faire que dans un cadre international si vous faites une taxation minimale international à l'impôt sur les sociétés, tout seul, ça ne sera pas efficace, donc je regrette effectivement le temps que ça a pris, et moi, c'est une recommandation de retrait ou sinon avis défavorable. Très bien, je mais aux voix l'amendement 322 avec 2 avis défavorable qui est pour.

qu'il faut sortir de 4 ambiguïté. Et il faudrait le faire assez rapidement par rapport à la contribution des entreprises, en raison de leurs profits. Et ces 4 ambiguïté Monsieur Ministre Lemaire, vous vous en êtes un peu à l'origine. Vendredi, après le conseil des ministres, vos éléments de langage sont je suis surpris de voir à quel point on accable les entreprises françaises qui affiche de bons résultats. à nos yeux, non fondée, comme souvent d'ailleurs la radicalité que vous aimez et celle des clivages et là, je vous le dis, ils sont creux et vide de sens, tout le monde ici se réjouirait si l'économie repartait mais elle a pas le même atteint son niveau de 2019, monsieur le Ministre, dites-le une économie inflationniste qui débouche sur une économie à 2 vitesses et les secteurs qui peuvent accroître leurs marges sous couvert de hausse des prix et les secteurs qui rognent sur leurs marges pour assumer la hausse des prix, il y a bien des entreprises qui profitent et il y a des entreprises qui perd 2ème ambiguïté vous dites de bons résultats pour les entreprises françaises c'est de bons résultats pour nos compatriotes mais ça devrait être le cas. Les salaires augmentent à 3 6 % en moyenne, selon l'OFCE, de 8 % en taux médian, selon le cabinet Mercer, pour une inflation à 6 virgule un de juillet 2021 2022, vous préférez les accessoires de rémunération plutôt que les salaires, comme le rappelle d'ailleurs l'examen qu'on vient de faire de la loi, pouvoir d'achat hé bien selon même cabinet seulement 18 % ont décidé d'accorder une augmentation de la rémunération dans la durée. ça c'est l'effet 3ème ambiguïté vous dites bien entendu comme nos entreprises font des bénéfices, elles doivent contribuer à l'effort national, bien entendu, sauf que pour ça, ça veut pas dire la même chose, la quatrième ambiguïté, c'est qu'il y a des contributions très Direct, croyez-moi, nos compatriotes préfèrent avoir l'argent dans leur poche que dans la poche de l'État, or c'est une taxe de l'argent dans la poche de l'État, mais pas dans la poche des Français, voilà, ça c'est le débat d'idées sur les ambiguïtés, excusez-moi, monsieur le Ministre, qui vous anime, qu'on a retrouvé tout à l'heure dans votre discours, mais faut qu'ici il y a d'autres amendements, d'autres vont les défendre mais c'est pas possible que loi, pouvoir d'achat plus toi le bois de finances rectificative il y a 0 maire euros de contribution des mises en musique.

de 50 % sur les bénéfices exceptionnels seul bénéfice exceptionnel réalisé par les plus grandes entreprises de plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires au cours du 1er semestre nous calculons ses bénéfices en comparaison de la moyenne des bénéfices réalisés pendant les 3 années précédant la crise Covid avant même l'accélération de la hausse des prix, le pouvoir d'achat était la préoccupation principale de nos concitoyens, il faut des petits impôts pour les petits revenus et de grosses impôts pour les gros bénéfices en effet alors que la population subit une dégradation rapide de son pouvoir d'achat, les dernières données de l'Insee nous indique que le taux de marge générale des entreprises à qui, en 2022 s'élève à 32 2 depuis 2010, ce taux a été seulement dépassé 2 fois en 2000 19 et 2021, cette augmentation des taux de marge montre qu'il y a une possibilité d'équilibrer l'impôt est un outil de la justice sociale et de l'équité, les entreprises doivent s'honorer de le payer.

il vise les entreprises dont le bénéfice Net aurait été en 2021 supérieur de 20 % à la moyenne des 3 années 2017, 2018 et 2019 qui se verraient ainsi appliquer une contribution à hauteur de 20 % calculée sur la différence entre les 2 montants, comme je l'ai dit en discussion générale en 2020 on n'a pas hésité à mettre en place une contribution exceptionnelle sur les complémentaires santé à hauteur d'un milliard 5, ça n'a pas fait débat ensuite au cours de la crise Covid nous avons voté tous les soutiens aux entreprises, je rappelle, par exemple, un prêt garanti par l'état d'un milliard à CMA-CGM on a voté les reports de charge tous les différents dispositifs, on était en soutien des entreprises quelles que soient leurs difficultés, on a été capables de voter des soutiens exceptionnels, il me semble, aujourd'hui, qu'on peut espérer une contribution exceptionnelle parce que elle est unique, elle est bornée dans le temps, enfin, je rappelle que tous les pays voisins, le mettre en place l'Espagne, l'Italie, la Roumanie, la Grèce, le Royaume-Uni et l'Allemagne y réfléchit et je n'ai pas l'impression qu'on pourrait être les seuls à avoir raison de ne pas y penser, merci.

par les sociétés de la branche énergie, eau et déchets ainsi que de la branche transports selon les derniers comptes trimestriels de l'Insee, ces 2 branches se distingue par une hausse spectaculaire de le taux de marge sur une très courte période dans la branche énergie, déchets, le taux de marge est passé de 60 pour 100 quatrième trimestre 2020 à 74 pour 100 au 1er trimestre 2022 dans la branche transport il est passé de 37 à 47 % sur cette même période, autrement dit, ces entreprises ont exploité le contexte d'inflation pour augmenter leurs profits d'environ un quart si une partie de l'inflation française résulte bien de facteurs internationaux ravitaillement guerre en Ukraine se sont donc également des entreprises présentes en France qui l'ont alimenté en augmentant trop fortement leurs prix de de sorte à faire gonfler leurs marges par conséquence pour lutter contre l'inflation, il faut mettre fin à ces agissements qui servent carrément à faire augmenter la crise et l'inflation la taxation de ses profits de crise proposé par cet amendement du groupe écologiste solidarité et territoires présente le double Avantage de permettre de financer des mesures plus ambitieuses en direction des personnes fragilisées, inciteraient également les entreprises à modérer leurs marges et à contribuer ainsi au ralentissement de l'inflation des pays européens comme l'Italie, l'Espagne, la Roumanie et le Royaume-Uni ont pris cette voie. Merci monsieur le président, il y a beaucoup d'amendements qui vont dans un sens commun mais on est sur le hein certainement des débats les plus important de ce PLFR notre amendement, lui, il vise à instituer en 2000 22 et 2023, une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés de l'énergie et des transports ainsi que les sociétés autoroutières qui sont redevables de l'impôt sur les sociétés, pour un chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros s'agit bien d'un homme très limité d'entreprises en instituant une contribution exceptionnelle à hauteur de 25 % du résultat imposable, enfin je dois dire, si le Sénat votait l'amendement les à hauteur de 20 % du résultat imposable, nous serions très heureux aussi parce que l'important, c'est le principe et c'est d'avoir une recette aussi pour l'État d'ailleurs, je dois dire, puisque nous avons déjà beaucoup parler de la question et je remercie Monsieur le Ministre, d'être aussi, restez avec nous pour débattre de cette question importante, je n'ai pas été convaincu par vos arguments, et ils sont quand même très z'idéologique parce que, d'une part, question du niveau global de fiscalité, mais on n'est pas là dessus, et si on est sur la question du niveau global de fiscalité, alors quand on voit les chiffres des recettes de l'impôt sur les sociétés cette année et l'année dernière qui augmente en effet très fortement quand on apprend que ces grandes multinationales elles-mêmes ne paye que très peu d'impôts, alors il y a une inéquité fiscale entre les entreprises qui peuvent se permettre et qui pratique une très forte évasion fiscale, et celles qui rapporte aussi sous forme d'impôt sur les sociétés de la des ressources financières pour l'État et donc cette taxe sur les superprofits rétablirait de l'équité fiscale entre les entreprises françaises et ensuite il faut choisir son argument soit cette taxe, de toute façon, hein les veines, elle ne rapportera rien, puisque rien n'est produit en France sur, je suis dans ce cas-là, on peut se la permettre, soit 7 une spoliation, elle est très dangereuse pour notre économie, mais il faut choisir entre les 2 arguments Amendement 320 Monsieur Bocquet. Oui, merci Monsieur le Président, amendement strictement identiques dans son objet, je ne vais pas développer davantage, simplement je voudrais citer Madame la première ministre qui disait il y a quelques temps sur le principe, évidemment, s'il y a des gens qui tirent des surprofits de la crise, on souhaiterait que ça puisse bénéficier à tout le monde et alléger les charges que la crise peut générer, c'est ce qu'elle affirmait après ce n'est pas complètement déjà on nuance, beaucoup de nos voisins ont mis en place des mécanismes pour taxer ces surprofits mais on n'est pas dans la même situation en France évidemment, c'est ce que nous entendons encore aujourd'hui alors parmi les singularités de notre pays, je veux quand même citer cette politique des dépenses publiques, des aides publiques accordées au monde économique sans conditionnalité, on peut très bien en France et des entreprises qui, le mois suivant, licencie des personnels et entreprises peuvent toucher des aides publiques mais aussi ne pas payer d'impôts sur leurs bénéfices en France, on en a cité plusieurs cas, les entreprises peuvent toucher les aides publiques et verser des dividendes voir augmenter ses versements donc effectivement cet amendement, nous paraît totalement justifié.

sur les entreprises qui ont connu une augmentation significative de leur chiffre d'affaires en 2022, et ou en 2023, à titre d'exemple, cette taxe devrait permettent de récolter environ 4 milliards d'euros pour Total 925 millions d'euros pour Engie 4 4 milliards d'euros pour CMA CGM 875 millions d'euros pour les concessionnaires d'autoroutes, simplement ce que je voulais aussi rajouter c'est que cet amendement il il montre aussi que le le groupe sert est ouvert au débat. Il propose un montage moins extensive de ce qui est désormais communément appelée la taxe sur les superprofits. Nous considérons qu'il peut y avoir un rejet de principe idéologique de toute taxation sur les superprofits, auquel cas, monsieur le ministre, il faudrait simplement le dire et l'assumer, ou un rejet techniques liés au montage du dispositif. C'est pourquoi nous proposons avec cet amendement, un dispositif moins conséquent, malgré des chiffres records annoncés par Total, il y a quelques jours. je vais même aller plus loin mes chers collègues, nous sommes prêts à débattre de sous-amendements car au-delà de l'aspect technique, nous voulons que le Sénat vote une taxation sur les superprofits ceux-là, je crois, sera un symbole fort de justice sociale, fiscale pour le pays et nous vous y appelons. Merci. Avant de donner la parole pour les explications de vote, je signale tout de suite que je suis saisi d'une demande de scrutin public sur chacun des amendements, il y aura donc si scrutin public puisque, il y en a deux qui sont identiques. Monsieur Chantrel ah pardon pardon pardon pardon avant le oui vous voyez comme quoi je vais vous donner la parole trop vite : avis de la commission sur chacun de ces cet amendement. Alors, tous les avis seront défavorables, le monsieur Bouquet je veux rappeler que vous voulez asseoir l'imposition sur des résultats sur des longues périodes 2017 à 2019, 2020, 2022, en fait, si ça progresse, vous vous dites qu'il faut en prendre encore plus, alors qu'on a quand même intérêt à ce que les entreprises soient plutôt des entreprises en bonne santé, monsieur Bruillet défavorable également vous il y a une difficulté alors vous mettez là le le le plancher hein 750 millions d'euros, mais quand on regarde si on met l'impôt sur les sociétés et votre proposition, ça fait quand même un taux normal d'imposition pour les entreprises auxquelles vous pensez de 75 % je pense pas que ce soit un bon signal envoyé. Sylvie Vermeillet sur les les profits exceptionnels : premièrement, je pense qu'il y a un souci puisque vous visez les entreprises qui ont réalisé des profits en 2021 et non en 2022, donc moi j'interprète ça n'a rien à voir avec la crise de l'énergie, ni la crise en Ukraine, je pense qu'il y a plusieurs difficultés : premièrement, ça peut avoir des conséquences dommageables pour les entreprises en croissance, deuxièmement vous voulez toucher toutes les entreprises, avec un résultat supérieur à un 1000000 d'euros, c'est une assiette qui me paraît extrêmement large pour pas dire excessivement large troisièmement cette contribution elle va tomber et vous le savez, a posteriori, c'est-à-dire que les entreprises qui ont fait des choix d'investissements et distribue des dividendes se retrouveront à posteriori sanctionné, je trouve que cette un peu dommageable et enfin pour conclure je pense justement que par votre proposition, le risque c'est de faire peser sur les investissements des entreprises prévu de le de brider ses investissements à venir. Monsieur alors ensuite c'est monsieur Breuiller, alors qu'il revient avec le chiffre d'affaires, y compris les petites entreprises et dans ce cas-là, le taux d'imposition pour toutes les entreprises du secteur que vous évoquez, c'est 45 %, je crois que c'est pas aujourd'hui, ce dont on a besoin, Liès d'ailleurs qui baisse, vous voyez qu'il produit en tous les cas pour l'instant davantage de recettes

là, je pense que c'est des conditions qui sont des conditions fortes que vous faites porter sur certains secteurs d'activité qui d'ailleurs ne donne pas tous, je dirais, ne répondent pas tous à des impositions qui aurait lieu sur le territoire national et il faut faire attention donc à ne pas taper, je dirais, à côté, en proposant de prélever auprès de ces entreprises, moi, je rappelle que je partage l'idée qui est que quand il y a une situation difficile, je pense qu'aujourd'hui les entreprises dans leur secteur d'activité, si elles peuvent immédiatement, mais les politiques plus offensive pour accompagner dans la difficulté, les Français, c'est ça qu'il faut choisir if certainement qu'il faut donner un cadre nouveau pour exercer cette possibilité mais c'est la réactivité et d'efficacité qui sont à privilégier davantage que la taxation. Oui : avis défavorable sur chacun des amendements, monsieur le Président, je pas reprendre dans le détail les excellents arguments avancés par le rapporteur général, juste une remarque générale et de remarques plus de circonstance. La général c'est qu'il y a une chose que nous n'avons jamais essayé dans notre pays qui explique peut-être des résultats économiques qui étaient décevants au cours des décennies passées. C'est la stabilité fiscale. Et je pense que la stabilité fiscale n'a pas de prix. Elle permet aux entreprises d'investir. Leur donne de la visibilité sur le long terme. Elle a fait de notre pays, le pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe. Et croyez-moi, on ne fait pas venir une entreprise comme GlobalFoundries pour être un des 5 pays, producteur de semi-conducteurs de la planète. Avec de véritables technologie de rupture. Si on ne garantit pas la stabilité fiscale. Quand une entreprise comme Global fonderie fait un investissement de 6 milliards d'euros. Ils ont besoin d'assurance en Isère sur la stabilité fiscale. Donc j'entends moi tous les arguments côté avancer, il faut aider plus les plus modestes, les plus fait tout ça s'entend parfaitement. Mais j'aimerais juste qu'on pousse le raisonnement un tout petit peu plus loin en se disant : mais quand on regarde dans les 30 dernières années qu'est-ce qui fait que on n'a pas toujours gagner la bataille des investissements étrangers, qu'est ce qui fait que nos entreprises ont hésité à investir.

Et puisque vous me demandiez un argument pour lequel effectivement je refuse cette taxation, c'est au nom de la stabilité fiscale que nous avons inscrite depuis 5 ans au fronton de cette majorité. Enfin, si on regarde plus dans le détail, vous me dites, en citant 2 entreprises Total et CMA-CGM, on fait des profits considérables à cause de la situation actuelle. D'abord, vous me permettrez d'être un tout petit peu gêné aux entournures quand il faut pointer du doigt des entreprises qui font la force de notre économie, je trouve qu'il y a toujours quelque chose de gênant et pardon je resterai sur cette ligne-là a pointé du doigt une entreprise ou une autre, un nom ou un autre, c'est ma conviction, c'est ma conviction respecter là. Vous me dites, ces entreprises là, elles ont profité de la situation actuelle, elles doivent rendre aux français oui. Je suis d'accord. Mais il a remise que Total fait de 20 centimes d'Euro par litre de carburant sur toute cette station stations rurales comme stations autoroutières coûte un demi-milliard d'euros total j'estime qu'on peut juger que ça n'est pas suffisant, on peut juger qu'il pourrait faire plus, simplement on ne peut pas dire qu'ils n'ont rien fait. Même chose pour CMA CGM, une remise de 750 euros par container, on peut juger que ce n'est pas assez, on peut juger qu'ils doivent faire plus, on ne peut pas dire qu'ils n'ont rien fait. Et ensuite, vous avez toutes les autres entreprises qui sont dans le Champ de vos amendements et et qui n'ont, oh grand rien demandé à personne. Stellantis Renault. STMicro dont je viens de parler. Engie d'autres entreprises encore mais pourquoi donc ce qu'elles seraient soumises à un impôt exceptionnel, ces entreprises elles sont confrontées à la transition énergétique, les entreprises automobiles doivent investir massivement dans les nouvelles chaînes de traction dans le véhicule électrique dans l'ouverture de nouvelles usines, mais moi je préfère très sincèrement qu'elle paye leur et qu'elle paye plus IS parce qu'elles ont plus de bénéfices, mais qu'elle garde des marges pour investir en France, réussir la révolution du véhicule électrique et du coup être des entreprises profitables dont tous nos compatriotes pour pouvoir bénéficier donc on peut ne pas être d'accord, je je pense pas qu'en disant qu'elle honte madame la sénatrice en fassent beaucoup avancer le débat, on a eu non je suis désolé je réfute ces arguments : je pense que si, au cours de ce débat qui va durer longtemps, on commence à se lancer des invectives de honte quel scandale, on ne va pas beaucoup progresser, vous avez avancé vos arguments, madame la sénatrice, j'avance les miens et je suis convaincu que pour l'intérêt national, la stabilité fiscale n'a pas de prix. Très bien. Allez dans un relatif calme, j'ai plusieurs demandes de parole. Si on pouvait s'écouter, ce serait bien monsieur Chantrel d'abord. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, c'est pour le moins absolument pas convaincant, l'argumentaire que vous venez de de développer un peu choquant, j'ai l'impression que vous reprenez votre théorie votre vieille antienne votre catéchisme je dirais libéral que que vous asséner depuis ces dernières années sur la fameuse théorie du ruissellement dont personne ne voit jamais ruisseler sur lui, à part les catégories les plus les mais plus grave encore, c'est qu'en fait c'est le le parallélisme déflagration heures entre le débat qu'on a eu la semaine dernière, où vous avez obstinément refusé d'augmenter les revenus des plus défavorisés à travers le revenu minimum et le débat que nous avons aujourd'hui ou vous refusez avec des pudeurs de gazelle en quelque sorte de taxer ceux qui profitent de la crise, parce qu'ils profitent de la crise taxer 25 pour 100 des super profits de Total je vous rassure, ça laisse encore ça leur laisse encore 16 milliards sur l'année, je ne pense pas que ça, ils vont mourir ou ça va poser des problèmes pour cette entreprise on parle beaucoup de Total, mais il y a aussi les concessionnaires d'autoroutes que vous avez vous-même, et je peux comprendre que vous êtes un peu mal à l'aise pour les taxer, parce que vous avez participé quand vous étiez directeur de cabinet de Monsieur de Villepin allait privatiser et à faire en sorte que justement qu'qui s'engraissent également au moment où nos compatriotes sont sur les routes, la facture est très salée également quand ils prennent l'autoroute quand ils ont la chance de pouvoir partir en vacances, malheureusement c'est pas le cas de tous nos compatriotes, donc il serait peut-être temps d'agir et d'envoyer un message de justice sociale, parce que l'injustice que vous créez, c'est le terreau des révoltes de demain, si vous voulez pas avoir à nouveau des révoltes, des manifestations de masse ah agissait tout de suite aller dans le sens de la justice sociale, JC, envoyer des signaux positifs que dans ce pays, oui, la répartition des richesses, c'est possible, faites-le, ayez ce courage. courage. Alors. J'ai d'ores et déjà une douzaine de demandes de prise de parole donc, chacun son tour Madame Bricq et. Merci monsieur le président, cette taxation sur les superprofits à effectivement nos nos débats mais c'était, c'était prévisible et le fait que des amendements viennent de de plusieurs bon ça prouve bien là l'intérêt du sujet, j'ai bien noté, Monsieur le Ministre votre hostilité à à toute taxation sur les superprofits et pourtant, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, vous avez pu mettre en oeuvre des dépenses exceptionnelles, pourquoi refuser ces recettes exceptionnelles, alors même que, selon vous, dire la cote d'alerte est atteinte en matière de finances publiques est-ce à dire que seule la réduction de la dépense sera de mise et on on sait bien qui, au final, paiera l'addition au nom de la stabilité fiscale doit-on faire entrer sur la justice sociale. merci, monsieur le président, Monsieur le Ministre, nonobstant désagréments que j'ai causé à mes collègues, nous ne voterons pas ces amendements. nous, parce que pour nous, la justice et l'efficacité, l'efficacité, c'est que chaque Français trouvent dans son porte-monnaie dans son pouvoir d'achat, les bienfaits des mesures qui sont prises, or, Monsieur le Ministre, la rappelé aujourd'hui pour ce concerne au total mieux vaut un prix de l'essence demain à un euros cinquante qu'une taxe qui irait à l'État pour avoir des effets sur le pouvoir d'achat immédiat, deuxièmement qu'autrement ce qui vient d'être dit là que la théorie du ruissellement a fonctionné pour notre pays, depuis 5 ans, les créations d'emplois nettes, plus d'un 1000000 et demi d'emplois créés, les baisses d'impôts pour chacun d'entre nous, la valeur ajoutée qui a été trouvé en France aujourd'hui, les moyens qui ont pu donner de dit hausse des minima sociaux que nous avons accordé, ils ont été faits, grâce aux profits qu'on les entreprises, la France n'a pas besoin de taxes supplémentaires, la France a besoin d'investissements de créations d'emplois, de création de richesses qui permettront de développer notre pays si vous taxez aujourd'hui vous allez taxer Total Énergie, qui fait des profits à l'étranger et tant mieux si nous avons un fleuron est-ce que vous allez toucher tu taxer British Petroleum est-ce que vous allez taxer, ex-homme qui au cri de peu à côté, et ces entreprises y compris CGM on crée des difficultés qu'elle était au bord de la faillite, vous n'avez pas ce jour là, crée les moyens pour les aider et de aujourd'hui en faisant des autres pour nos territoires d'outre- mer, il voit accompagner le développement ces pays et puis en fin de compte, comparaison n'est pas raison si on veut prendre à chaque fois, la Grèce, l'Italie, l'Espagne et tout, regardez la France et elle et le pays qui prélève le plus mais qui aussi dans le même temps, redistribue le plus et moi je voudrais savoir comment ont été traités les espagnols, les Italiens, les Roumains et caetera au moment de la crise du Covid

si l'État le fait, donc moi je crois que ce signal que nous allons donner, hé bien c'est que les grandes entreprises vont faire un effort pour aider les Français demain, nous serons au rendez-vous de résultats qui seront donnés, si jamais ils tiennent pas leurs engagements, alors nous on tiendra compte dans le budget, futur. Merci, merci Monsieur le Président. La parole est à monsieur Assouline. Monsieur Attal a nous a dit qu'il le répète souvent, fini le quoi qu'il en coûte, combien ça coûte, or la vraie question n'est pas celle-là, la vraie question, c'est : qui doit payer dans un moment de crise pour l'ensemble du pays, on aurait pu penser qu'après les résultats électoraux pouvait se vouer une certaine sincérité de l'urgence de la situation, parce qu'il y a une guerre parce qu'il y a une crise sociale qui a été très présente dans la campagne électorale et que, comme ça a été le cas d'ailleurs au lendemain de la 2ème Guerre mondiale, gauche et droite puisse s'entendre sur des mesures exceptionnelles qui voient l'intérêt du pays et de nos concitoyens, or là, vous voyez bien, monsieur le maire que vous êtes dans la lignée de ce que vous avez toujours défendu, donc je vais pas vous le reprocher et que en admiration devant vous et vous applaudissant c'est la droite de l'hémicycle. Il n'y a rien qui viennent faire des des mains tendues vers les préoccupations que la gauche défend dans le pays dans le précédent débat c'était pas d'augmentation de salaire donc on touche pas à ceux qui, faisant des profits doivent être encouragé et pas seulement par vos propos, mais par des mesures à augmenter les salaires alors qu'ils sont bas et qui ne permettent plus de vivre pour nos concitoyens et maintenant dans le débat sur qui a, dans un moment de crise majeure fait des profits, ce qu'on appelait à une époque les profiteurs de guerre, le minimum qui peut rassembler. Les progressistes de la gauche et de la droite et de dire que on va les taxer, c'est d'ailleurs pour cela que les centristes de l'hémicycle, qui ne sont pas de gauche considèrent que de façon exceptionnelle, il faut la aller chercher l'argent, vous dites encore non, donc vous ne représentez nouveau défendait dans ces 2 débats que les intérêts de ceux qui ont déjà beaucoup et vous tournez le dos

ça vole, ça vole délit hein, non, non, mais c'est, c'est c'est comme ça, merci monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, d'abord par rapport à ce qu'a dit le rapporteur général et et Monsieur le Ministre, Lemaire. On a une petite confusion là les entreprises, les entreprises faut faut savoir de quoi on parle. Il y a différents types d'entreprises, tout le monde le sait ici. Vous nous parlez de stabilité fiscale, Monsieur le Ministre, enfin. C'est mon collègue Gilles Carrez peut pas l'accuser d'avoir été à gauche. Rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, c'est lui qui a fait la démonstration qu'il avait une équité entre les PME et les multinationales, vos services ont travaillé à la loupe les liasses fiscales des sociétés françaises. Pour les PME, c'est un taux effectif de 24 20 24 % et pour les multinationales, c'est 17 53 %. Donc ce qui se font avoir dans cette affaire, c'est les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas la même fiscalité, eux ils ont pas le droit à la stabilité fiscale, ils ont droit à être mis à contribution, donc argument retourner et non valable de vote pas la 2ème chose, vous nous dites. Enfin, on va discuter des chiffres. Le geste qu'ils vont faire avec beaucoup de générosité, là les 500 millions on sait pas trop d'ailleurs comment ça a été calculé et vous imaginez ce qui se passe pour eux. C'est 0 2 % de leur chiffre d'affaires. Et je le dis à mes collègues de droite, j'étais là, l'autre soir, moi, vous voyez, quand je vois que Total va nous faire une concession de 0 2 % de son chiffre d'affaires à partir des bénéfices qui l'a fait et qu'ici, on l'avait un débat pour réduire de 0,5 l'augmentation des allocataires du RSA, je pense qu'on voit bien le niveau qui fait qu'il a de camps dans cet hémicycle, il y a un camp qui défendent le capital, la droite il y a une collusion entre le gouvernement et la majorité sénatoriale, et puis il y a un autre camp, et des fois il peut s'élargir sur ces questions, il faut qu'on sorte de ce débat avec au moins un euros de contribution des bénéfices des entreprises. Il le faut. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, un de vos arguments, nous indique que de nombreuses entreprises ne font pas leurs bénéfices en France effectivement, lorsque l'on regarde les bénéfices de Total Énergie on peut se poser des questions en 2020, ils n'ont payé aucun impôt en France malgré un bénéfice de 10 milliards en 2019 comment vous venez vous expliquez-nous que une entreprise qui a son siège en France, qui a 21 % de son activité en France n'a aucun bénéfice en France, pire elle déclare des pertes en France et le Trésor Public lui a remboursé 126 millions d'euros, je trouve qu'il y a quand même là un petit sujet et il serait peut-être temps de donner les moyens à nos services fiscaux pour aller chercher là où sont les fraudes parce que les multinationales, hé bien, on peut pas dire qu'elle joue le jeu de la solidarité, c'est le moindre, la moindre des choses que je puisse vous dire. Merci. Madame Goulet. évidemment, la crise que nous subissons aujourd'hui doit être dans le prolongement de de la crise dans l'est de la crise sanitaire et à ce moment là, Monsieur le Ministre, nous avons voté dans cet hémicycle l'interdiction, en tous les cas, la réduction des aides Covid pour les entreprises qui avait des filiales dans les paradis fiscaux total est quand même en bonne place dans les Panama Papers, nous avions aussi demandé à ce que les aides Covid ne soient pas attribués aux entreprises qui distribuer des dividendes, nous n'avons pas pu obtenir satisfaction et puis dans les entreprises qui ont fait beaucoup de de profit, on a évidemment cette cette entreprise mais pas seulement nous avons LVMH 107 pour 112 milliards STM électronique

tout à fait normal Sylvie Vermeillet l'a très bien expliqué, il y a eu des aides exceptionnelles au moment de la crise sanitaire, il y a aujourd'hui un prélèvement exceptionnel pour aider à passer ce cap, lié à la crise de l'énergie et à l'inflation et donc il n'y a rien de de choquant pour nous à avoir une taxe qui est bornée dans le dans le temps et je pense que nous sommes tout à fait dans notre droit et tout à fait légitime en étant tout à fait en opposition avec ce que vous dites est tout à fait conforme à ce que nous pensons. Merci, la parole est à monsieur Kahn. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, en 2020 et 2021 la France à aider les entreprises à surmonter la situation pandémique qui a causé beaucoup de dégâts et a permis, je crois, aux entreprises de de bien se porter et il faut s'en souvenir, et cela a coûté aux finances publiques aujourd'hui on s'aperçoit quand même qu'un certain nombre d'entreprises et les journaux égrène tous les jours des résultats bien supérieurs, le double, triple voire le quadruple des résultats habituels réalisés par un grand nombre d'opérateurs dans notre pays et, bien sûr, il se pose la question de savoir si l'inflation que l'on connaît par ailleurs que chaque consommateur connaît n'engrange pas justement de profits pour ou de super-profits pour ces entreprises, c'est-à-dire est-ce que ces entreprises finalement ne profite pas complètement de la situation inflationniste que nous connaissons, alors il faut se poser la question et je crois que l'amendement qui est présenté par Sylvie Vermeillet et le groupe de l'Union centriste est fondamentalement différent de celui qui est présenté par les autres groupes, tout simplement parce que c'est une construction exceptionnelle qui est basé sur la moyenne des de de profits dépassant la moyenne réalisée sur les 3 années de 2017, 2018, 2009, c'est-à-dire avant la crise, il s'agit simplement de taxer cette partie-là, de en fait de mettre en place une contribution exceptionnelle, donc il est différent, cet amendement de celui présenté par les autres groupes, et il ne faut pas considérer que ce soit une taxation forte, forte, c'est une taxation qui ne toucherait que les entreprises qui vraiment ont réalisé un profit notablement supérieur en 2021 par rapport à à ceux de la moyenne des 3 années avant et et il faut pas surtout pas confondre ça avec des gestes commerciaux qu'un certain nombre d'opérateurs, par ailleurs, sont en mesure de faire et de proposer aujourd'hui. Si Monsieur K. Dick. Merci monsieur le président, oui, pour ma part, je suis opposé à ce type d'imposition circonstanciel qui nuit à la clarté et à la sécurité juridique des contribuables et qui est d'autant plus démagogique que ce rendement fiscal serait faible, une politique fiscale efficace, favorable à la productivité économique et donc au pouvoir d'achat implique de suivre des règles fixées préétabli, c'est une question de sécurité juridique s'il est bien un aspect de la loi fiscale qui décourage les entrepreneurs, c'est sa rétroactivité, il est difficilement compréhensible que des opérations faites par les entreprises en considération d'un régime fiscal donné puisse faire l'objet a posteriori d'un traitement fiscal différent, le respect du droit et des libertés fondamentales, y compris en matière fiscale suppose le respect de principes supérieurs qui n'ont pas à varier au gré de l'opportunité, ce comportement déloyal de l'État finit toujours par se retourner contre lui sur le plan interne, le principe d'égalité devant les charges publiques s'oppose à une taxation discrétionnaire de quelques contribuables sur le plan européen, le principe de protection de la confiance légitime oblige la puissance publique à respecter la parole donnée, c'est la stabilité fiscale nécessaire dont nous a parlé le ministre, vous avez parlé de l'Espagne, la taxation aura un effet en 2023 et 2024 ça ne règle rien pour la situation actuelle, vous parlez du Royaume-Uni où je réside et juillet une entreprise les données récentes fiscales qui sont proposés en augmentation par l'ancien ministre des finances, qui est candidat à être 1er ministre est contredit par ça part ça contradictoire, la personne qui est en face de lui pour être Premier Ministre et qui veut baisser ses impôts.

Monsieur le Ministre, comme j'ai souligné en commission des finances, mais comme j'ai pas reçu la réponse, je voulais savoir quelle était la définition des super profits parce que moi j'ai quelques difficultés à savoir de quoi il s'agit, et je dois dire que c'est pas les débats qui m'ont véritablement éclairé, alors j'ai essayé de comprendre si les superprofits c'était pas les profits d'une société qui se rétablissait qui elle commençait à être bien gérée peut être alors la SNCF, par exemple, si je reprends les bénéfices des dernières années, elle a fait un milliard trois en 2017 141 millions en 2018, une perte de 811 millions en 2019, c'est-à-dire une moyenne de 223 millions si j'applique la taxe par exemple de l'amendement numéro 130 elle va payer 133 millions de super-profits Poste La Poste c'est 851 millions pour le groupe La Poste, 798 millions en 2018 depuis 822 millions en 2010 2 milliards à la suite de la reprise de provisions pour 2021, donc la Poste va payer 250 millions de super-profits j'ai pas fait le calcul pour Air France, Monsieur le Ministre, est pour les c'est agriculteurs éventuellement qui bénéficient de l'augmentation du blé en Ukraine ni pour, je dirais, les commerçants ou les entreprises qui sont en Île-de-France et qui auront peut-être des super profits à l'occasion des Jeux olympiques, et donc je vous demande la définition exacte pour Bercy des superprofits parce qu'en réalité, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans la recherche d'une certaine démagogie pour taxer tous les profits en réalité c'est un pays ou bien qu'on ait la fiscalité la plus importante des pays développés dès qu'il y a un profit ou une réussite quelque part, il faut taxer tous les profits et ce débat me déplaît sur ce sens-là et je ferai une remarque, Monsieur le Ministre, pour montrer que je ne suis pas en connivence avec vous, il n'y a pas de : il fallait peut-être pas ouvrir certaines sociétés pointés du doigt au moment des Gafam en disant : tel ou tel, secteur avant des superbes conclure cherche des plaques spéciales et voilà l'occasion d'y revenir, merci. Monsieur le Président Retailleau. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, je sais que tous ces amendements ont le goût sucré, des mesures qui n'ont que l'apparence de la justice sociale, je pense que ce sont de fausses bonnes solutions pour 2 raisons : la première raison, parce que ces amendements, ces mesures sont à la fois faussement efficace et faussement équitable faussement efficace parce que créer une super taxe par exemple sur Total n'amènerait aucune rentrée d'impôts, je préfère, je préfère que l'effort de cette société soit empochés par les Français plutôt que par Bercy faussement bien sûr efficace et faussement équitable faussement Epita parce que, évidemment, les résultats d'une entreprise quelle qu'elle soit ne dépend pas toujours des stratégies éclairés de ces entreprises, les stratégies bien sûr compte mais ce qui compte, c'est l'environnement des entreprises est-ce que demain vous allez créer une super taxe pour ceux qui, aujourd'hui, parce qu'il fait très chaud vendent plus de bouteilles d'eau minérale pour ce que lorsqu'il fera très humide vaudront et cetera,

l'argument le plus important, c'est que je pense que dire aux Français que la solution, ce sont les taxes, c'est leur mentir les taxes en France les impôts en France, c'est le problème la France a choisi de faire financer sa dépense publique en surtaxant les entreprises la différence la différence par rapport à la moyenne européenne, notamment dans la zone Euro, c'est près de 7 points de PIB, ce qui fait qu'avec l'Allemagne que le ministre cité tout à l'heure, mais sans citer le chiffre, c'est 150 milliards de différence, c'est 4 fois plus d'impôts, de production, c'est beaucoup plus de charges sociales et c'est ce qui a conduit à la désindustrialisation de la France, voilà, je pense, mes chers collègues, pourquoi il ne faut pas voter ces amendements, je pense que si le remède, franchement, c'était les taxe sur les superprofits si c'était le remède à nos malheurs français, nous qui sommes le pays champion du monde avec le Danemark, de la fiscalité, alors je ne douterait pas que ça soit non seulement la France, ce pays le plus civilisé mais il, je pense que quand serait à l'avant-garde aussi du bonheur universel. Plusieurs monsieur le président. La parole est à monsieur Tissot.

qu'elle a qu'on risque de la malmené, mais vous avez pas crainte la malmener finalement pendant la crise Covid Kant des plus grosses entreprises ont ont bénéficié des PGE et on a auditionné il y a pas longtemps monsieur Saadé, il nous a dit clairement que oui, il avait gagné plus d'argent maintenant comment ça allait être distribué, c'est à nous de le décider et aujourd'hui vous nous dites aussi que finalement c'est les entreprises qui décident, à l'image de Total combien ils vont donner combien ils vont participer, je croyais moi naïvement que c'était le Parlement, le gouvernement qui décède le taux d'imposition finalement vous monsieur le ministre, aujourd'hui, ce soir, vous nous faites la démonstration que c'est la charité de vous organisez, vous avez plus le ministre de l'économie, vous êtes le ministre de la charité. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, je voudrais vous paraphé, vous avez dit la la stabilité fiscale, elle n'a pas de prix, la stabilité fiscale, elle peut, elle peut avoir du sens. Mais ça me paraît compliqué au sortir d'une crise importante dans lequel l'État à accompagner les entreprises et notamment les plus grosses, par des par des, des, des subventions par des aides pour passer cette crise, je crois qu'aujourd'hui, il peut y avoir un retour de de bons procédés. Après, je vois bien, on est dans un débat dogmatique. Par contre j'ai j'ai moi, je voudrais vous interroger Monsieur le Ministre, sur un problème de concurrence. Aujourd'hui, vous encouragez Total a versé. à aider au financement du litre d'essence à hauteur de 20 centimes. Moi je ce que je voudrais savoir c'est comment vous allez répondre dernière j'ai j'ai lu une interview dernièrement au président du du CNPA, Centre national des professionnels de l'automobile, qui s'inquiète de cette baisse baisse artificielle, que vous avez encouragé auprès de Total, en disant mais nous petit petites exploitant de de stations service. C'est notre pérennité qui est en jeu. Parce que demain on n'a pas les moyens nous de de pouvoir nous aligner sur ce que Total va faire donc le consommateur assez naturellement va se retourner vers vers Total, donc j'aimerais avoir votre retour sur cette sur Et je crois que dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, il y a un moment où l'état, elle doit réguler et je crois qu'on est clairement dans un sujet dans lequel on doit l'État, le gouvernement, le Parlement doit réguler et peut pas laisser le marché faire et je pense sincèrement qu'une taxe même minime aurait vraiment du sang sur les sur ces superprofits. Merci monsieur Seguin. Oui, merci Monsieur le Président, juste une question, on a une balance commerciale. Qui est ultra-déficitaire, elle est déficitaire d'année en année elle continue de se dégrader, c'est lié à la délocalisation,

Il est supérieur, vous pouvez être à 5 kilomètres vous payez 2 fois moins qu'est-ce que vous allez faire vous avez vous, installé dans la commune à côté, surtout si c'est pour payer de la dépense est-ce que vous allez comprendre un jour que la que l'imposition de la France, les entreprises qui sont internationales qui sont multinationales regarde, regarde ses taux d'imposition parce qu'elles sont liées à une compétitivité mais quand est-ce qu'on va arrêter cette dégradation infernale d'augmentation d'impôts pour se perdre toutes nos entreprises qui reste

Merci. Bon, écoutez-vous les uns les autres déjà, vous êtes déjà 22 à prendre la parole, alors si vous nous écoutez pas en plus monsieur meurt en. Allez, il y en a pour un moment, on va. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en France, on continue à à vouloir pénaliser ceux qui réussissent. Et moi j'ai envie de dire bravo à Total il y a tous ces hommes qui travaillent, bravo à cette histoire de la compagnie française des pétroles, on m'a appris moi une époque que l'énergie, c'était quelque chose qui touchait à la souveraineté, c'est quelque chose qui concerne les entreprises et les ménages tous les ménages, toutes les entreprises et on devrait se poser la question dans une période où l'énergie est chère, comment se fait-il que Total engrange des bénéfices colossaux, et c'est une bonne chose, je le redis et qu'EDF. Malheureusement, EDF cette pépite française, fruit de l'investissement de génération décidé, à une époque où les gouvernants pensaient à la génération suivante.

il y a un multiple mais je rappellerai quand même quelque chose à l'époque de Monsieur Jospin ou tout simplement pour aller, permettez-moi l'expression, faire plaisir aux Verts, on a arrêté Superphénix on arrêter d'entretenir les réacteurs nucléaires. Et la raison d'énergie chère nos compatriotes doit le savoir, c'est cette vision idéologique dangereuse pour la souveraineté de la France et pour le pouvoir d'achat des ménages lié à cette politique anti-nucléaire ridicule et dangereuse, et les Verts certains maintenant qui ont. Progressé ou qui ont mûri ou qui ont été touchés par la sagesse ou par la grâce, je cite Brice Lalonde reconnaissent, ils reconnaissent qu'être anti-nucléaire était une erreur magistrale donc, intéressons-nous à comment faire en sorte que les saisons, entreprise française fasse des bénéfices parce que les bénéfices d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain, hé bien. Allez on continue dans la joie et la bonne humeur Monsieur Dantec. Lors de cette Oui, merci Monsieur le Président, c'est c'est un débat intéressant parce que ça nous permet de de vérifier le catéchisme libéral classique face à une taxe sur les entreprises, nous avons donc l'attractivité de la France à défendre la stabilité fiscale pour ces entrepreneurs honnêtes qui prennent tous les risques et qui ont besoin d'une vision d'avenir et évidemment ça n'a rien à voir avec la réalité, la réalité c'est quelque chiffre que qu'on n'a pas encore cité et notamment un an. je le reprends de mars 2020 à octobre 2021 en cours, la richesse des grandes fortunes françaises a bondi de 86 %, soit un gain de 236 milliards d'euros à titre de comparaison, elles avaient augmenté de 231 milliards d'euros en 10 ans entre 2009 et 2019 en fait derrière votre orthodoxie libérale, il y a ce qu'on masque, c'est-à-dire une concentration de la richesse en France et la rupture finalement qui a été l'histoire sociale du XXe siècle de l'équilibre entre les revenus du capital et les revenus du travail, c'est ça la réalité et on on nous sort finalement une orthodoxie libérale du 20ème siècle pour masquer la rupture complète dans le la répartition de la richesse produite et Monsieur le Ministre, que vous avez dit tout à l'heure était assez faut aussi sur l'augmentation de l'impôt sur les sociétés, là aussi, orthodoxie libérale stabilité donc augmentation des recettes parce qu'on a baissé les taux maintenant non, c'est faux, l'impôt sur les sociétés, dans la même période entre 2017 et 2021, il a gagné 900 millions à comparer avec les 236 milliards gagnés, on a seulement un an par les grandes fortunes, en fait, je pense que ceux qui défendent aujourd'hui un capitalisme raisonnable, c'est plutôt la gauche parce que si ça continue comme ça, il n'y a plus de contrat social possible avec le capitalisme. Il en reste encore quelques-uns donc si on peut écoutez c'est bien. et il y a un phénomène de prédation en ce moment, et ce, mon collègue a souligne la la la, dis, et le président Macron a parlé il y a des profiteurs de guerre aujourd'hui, c'est un constat du président avec le que que que je partage et ils haussent leur taux de marge actuellement à des niveaux jamais atteints au mépris de toute solidarité ou même de la décence la plus élémentaire et on connaît, on connaît ces profiteurs de crise, on les connaît, c'est Total énergies c'est M. GM, moi je préfère qu'on les cite, c'est mieux, ça permet de, de, de visualiser un peu qui sont ces grands groupes de l'énergie ou du transport, qui occupent

mais vous faites confiance à Total pour faire la l'investissement, la transition alors qu'ils annoncent tous les jours des nouveaux projets d'extraction d'énergies fossiles, alors que ça fait 50 ans qu'ils sont au courant du caractère criminel de leurs activités sur le climat et qu'il fout rien à voir, même qu'ils agissent pour empêcher la diffusion de de de régulation possible. Et donc là nous ce qu'on cherche c'est pas l'aumône, c'est la justice fiscale et vous nous dites, tantôt c'est impossible, tantôt ça rapportera rien, vous êtes le ministre de l'impuissance fiscale nous ce qu'on veut, c'est la justice, mettons à contribution les profiteurs de guerre pour que tout le monde contribue à la crise qu'on traverse, merci. Merci Monsieur J'écoute attentivement le débat depuis un moment et j'ai l'impression que l'impôt c'est mauvais. Et toute augmentation d'impôts et seraient intrinsèquement mauvaise, j'ai même entendu certains de nos collègues évoqué que ça s'oppose à l'efficacité, la justice et l'efficacité, moi j'ose dire à ses collègues, bon c'est Marco au coin d'une idéologie, c'est la vôtre, je ne la partage pas, au contraire, je trouve tout ce qui est juste, tout ce qui sert la justice est efficace et lorsque on évacue l'aspect vertueux vertu et l'aspect un peu morale disons de très clairement le signal qu'on envoie à la société française, ben, c'est de dire que on peut prospérer, on peut être un profiteur de crise sans en payer si j'ose dire, une part en solidarité et pas en charité comme on ne le souhaite pas, moi j'estime que ce qui se dit là et notamment en économie ouverte, on on montra jamais l'impôt, faire une taxe exceptionnelle borné dans le temps ne remet en cause ni la stabilité fiscale ni l'attractivité du pays, l'étau l'impôt c'est pas simplement un taux, c'est aussi une expression, c'est aussi une politique et aujourd'hui vous dites très clairement que vous laisser prospérer des inégalités, des injustices, soit n'est pas efficace, ce n'est pas juste. Monsieur le questeur sueur. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je pense que tout cela repose sur une sorte de dogme en vertu duquel tout prélèvement serait intrinsèquement pervers à partir de ce moment-là, il y a bien entendu une erreur de raisonnement qui se répand, quand on parle de prélèvements extrêmement spécifique, on nous dit mais cela ouvre la porte à un prélèvement généralisée surtout et Monsieur le Président, Retailleau que j'ai connu plus inspiré nous expose que cela va poser problème pour les bouteilles d'eau minérale, c'est-à-dire que ça va entraîner une sorte de mouvement universel mais vous savez très bien que ce n'est pas vrai quand Total fait en 3 mois un profit on peut dire super profits de 4 7 milliards d'euros est-ce vraiment scandaleux d'imaginer que l'on puisse prélever une partie de cette somme dans l'amendement de monsieur Rémi Féraud, il est question du pétrole, les sociétés pétrolières, gazières transport maritime et tu autoroute mais enfin les Français qui paient l'essence, c'est quand même toujours assez cher, eux s'entassent aux péages d'autoroute, ces jours-ci et qui voient le prix, on nous a dit d'ailleurs que pour récupérer l'inflation, les sociétés d'autoroutes envisager de augmenter le tarif et regardez les profits des sociétés. Auquel les autoroutes ont été concédés est-ce que c'est vraiment scandaleux que de faire des prélèvements sur ces entreprises-là, alors, de grâce, ne dites pas que c'est généralisé, nous, nous pensons que c'est spécifique que c'est bien ajusté et tout simplement que c'est juste. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et donc, évidemment, vous faites pression Monsieur le Ministre, sur les grands groupes, pour leur demander de verser une obole et pour éviter une taxation, mais bien sûr que si les grands groupes verse cette obole, c'est pour éviter d'être taxé sur des sommes qui sont beaucoup plus importantes, donc on est bien effectivement sur une forme de charité qui concourt quelque part à verser une obole pour une partie des Français, une partie des français parce que le groupe Total qui décide effectivement de verser cette obole, ça ne concerne pas l'ensemble des Français, ça concerne les consommateurs qui auront chez Total c'est pas l'ensemble des Français, donc c'est une mesure qui est absolument inéquitable quelque part et qui est inadmissible, dans ce cas de de figure et on sait très bien que sur les superprofits puisque ça a été abordé par mes collègues mais les super, il se caractérise par des profits qui sont réalisés sur la crise à partir de la crise et ses profits qui ont été réalisées à partir de la crise, bien souvent, sont réalisés sur de la spéculation, c'est ça les superprofits profits aujourd'hui qu'il faudrait taxer pour revenir à une forme d'autant aussi, enfin, vous nous dites qu'effectivement il n'y aurait pas un effet immédiat sur les Français, mais rien n'empêche l'état français de mettre en place une taxation complémentaire et immédiatement de faire une compensation qui soient effectivement versées au niveau des Français comme vous l'avez fait au niveau du litre, donc on peut le faire de manière carrément immédiat donc, quand on y regarde un peu plus près, tout ceci est particulièrement inéquitable, la seule chose qui était cap qui est équitable, c'est une taxation sur les superprofits. Monsieur le Ministre, moi j'ai j'écoute attentivement le débat et je me pose la question de savoir s'il y a une évolution de votre doctrine fiscale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui des grands groupes comme Total, qui d'ailleurs paie pas beaucoup d'impôts en France quand même, ils ne sont pas maltraités, on n'est pas, on parle de d'imposition fiscale levée totale, ça tire pas si mal que ça De ne pas payer d'impôt exceptionnel sur des revenus exceptionnels, il s'engage à quelques libéralités et comme l'a dit mon collègue, Gilles et des stations Total, il y en a pas partout sur le territoire, et notamment dans le monde rural, il y en a très peu. Mais ça veut dire que demain n'importe quel contribuable pourra choisir de dire bah écoutez, moi je vais pas payer d'impôts, mais en contrepartie, je vais faire du bien autour de moi et et comment vous allez financer l'enseignement, alors peut-être que c'est pas votre préoccupation, comment vous allez financer les services de sécurité, ça, c'est peut-être plus votre préoccupation, l'armée, la gendarmerie, la police, dont on a besoin, si tous les contribuables se disent moi finalement je choisis de payer mon impôt différemment monsieur le Ministre, moi je souhaite que vous puissiez me confirmer qu'il y a bien une évolution de votre doctrine fiscale qui fait que chacun paiera. Comme il voudra, à qui il voudra et puis on lui dira merci parce que tu as fait du bien autour de toi, mais c'est pas ma conception de la justice fiscale et je vous ai dit Monsieur le Ministre, ce que vous ne faites pas dans le cas de la justice fiscale, malheureusement je le crains pour mon pays, c'est dans la rue que le peuple ira le chercher et ça je le souhaite pas, mais c'est comme cela que ça va se passer et c'est vraiment ce que je regrette. Merci. La parole est au président Laurent. Oui, je voudrais dire à mes collègues le des républicains, que la manière donc ils organisent, espèce de tirs de barrage sur les amendements que nous allons examiner avant même de rentrer dans le détail de ces amendements, dont aucun ne propose la révolution fiscale, aucun ne va mettre à mal au système économique ou écraser les entreprises, il s'agit d'une question précise que nous avons à débattent cet après-midi, c'est effectivement est-ce qu'on va taxer les superprofits je sais bien que monsieur Dominati j'ai entendu continuer à se poser la question de savoir si on a, je vais lui payer un abonnement aux Échos, vous verrez que toute la presse, on parle depuis des jours et des jours, donc c'est quand même pas un secret de polichinelle, ça existe bien, et c'est lié à la crise, je vous rappelle que Nicolas Sarkozy à la sortie de la crise de 2008, on en parlera, parce qu'il y a des amendements qui porte dessus a inventé une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Donc c'est pas une idée farfelue devant des de situation exceptionnelle de ce genre qu'on se pose ce genre de questions donc, voilà ce que nous voulons débattre et la dernière chose que je voudrais dire à monsieur Retailleau, vous parlez des taxes, des taxes, mais qui a construit un système fiscal qui n'est pas celui dont nous rêvons, qui est assis sur une grande taxe qui est aujourd'hui l'essentiel des recettes fiscales qui s'appelle la taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire que vous avez construit en détruisant peu à peu les impôts progressifs sur l'entreprise et sur les particuliers et sur les fortunes, vous avez construit un système fiscal qui est assis sur une task géante, la TVA, qui fait l'essentiel des recettes fiscales et qui elle est prélevée sur la consommation et la plus injuste de tous, nous, nous vous proposons de rétablir un tout petit peu de justice avec ces amendements au moins ayez la décence de les discuter pour ce qu'ils sont au lieu de les caricaturer comme vous le faites aujourd'hui. Merci. Monsieur Merci monsieur le Président, nos amendements, ils sont assez divers, mais je dois dire que ceux qui viennent de la gauche et notamment du groupe socialiste ne sont pas les plus déraisonnable parce que par exemple l'amendement du groupe centriste propose de taxer tous les super profits à partir de 1 1000000 de profits, ça concerne en effet beaucoup d'entreprises, nous nous le limitons à des entreprises, à la fois très importante et sur des secteurs très particuliers et je dois dire que pour nous, quand on veut prélever des impôts, ça n'est pas par méchanceté ni parce que nous n'aimons pas les entreprises ou leur réussite c'est justement dans un but de redistribution et c'est comme cela qu'il faut l'entendre et notre interpellation ne s'adresse justement pas à ces entreprises en leur demandant de faire des efforts volontairement ce qui ou un vol enfin de leur demander de faire des efforts de à elles-mêmes, ce qui crée d'ailleurs de l'inéquité, ça ne s'adresse plus vraiment d'ailleurs non plus au gouvernement, Bruno Lemaire nous a dit, une position très ferme déjà exprimée à l'Assemblée nationale, ça s'adresse à l'ensemble de notre assemblée, est ce que nous prenons nos responsabilités aujourd'hui en votant cette taxe ou est-ce que nous y reviendrons, je pense au débat budgétaire à l'Automne, en regrettant de ne pas l'avoir fait aujourd'hui. Merci. Monsieur le Président rénale initialement vous étiez le dernier mais j'en ai rajouté donc allez-y. Mais ce Usain monsieur le Président, mais quelques mots quand même dans ce débat d'abord sincèrement le débat sur, il y aurait ici des sénateurs pro-entreprises et des sénateurs contre l'entreprise est un débat caricatural complet pour ma part, je veux être simple et j'ai été patron de PME pendant des années. Je me sens tout à fait dans une vision pro-entreprises et je et je reconnais que d'avoir une fiscalité qui soit d'abord, nous l'avons voulu, je rappelle que la baisse de l'impôt de 33 25 s'est voulu par François Hollande, au départ, je le rappelle et c'est exécuté plus tard

Qui gagne de l'argent qui en reverse et cetera fonctionne et emploie des etc tout ça est parfait, il y a pas de débat là-dessus, le problème c'est que nous sommes aujourd'hui par rapport à un sujet qui est très simple, c'est que des entreprises qui ont travaillé de la même façon cette année que les années précédentes, qui ont fait en gros le même chiffre d'affaires font des résultats qui sont mirobolants, c'est ça la réalité, c'est ça la réalité, ça c'est un problème qui est très spécifique que l'on rencontre cette année, tant mieux pour l'entreprise de Total, dont je rappelle que son histoire est fortement liée à l'État il y aurait pas de grandes entreprises pétrolières si l'État, au départ, n'avaient pas investi et il l'a fait, donc aujourd'hui, total, par exemple, c'est pas la seule redonne au collectif, moi ça m'apparaît tout à fait légitime sur quelque chose qui est finalement quelque chose qu'ils ont gagné de manière tout à fait inattendu et pour une durée courte, donc voilà, regardons les choses comme elles sont, n'ayons pas peur de cela et avant son. Monsieur. Merci, merci Monsieur le Président, fin de compte, vous avez raison, monsieur le président, Raynald, on n'est pas en train d'échanger sur le fait de savoir si on aime ou on n'aime pas les entreprises, mais un de vos collègues, a lâché le mot il y a quelques minutes, on parle de redistribution et de quelle manière on considère la directrice la redistribution comme intéressante quand on a auditionné chers collègues Tissot Rodolphe Saadé, président de CMA CGM, effectivement, il a dit ça, mais il a dit aussi que, il y avait certains bénéfices utile. Comme le fait de redistribuer en plus de la participation de l'intéressement 4500 euros à chacun des salariés de CMA CGM au printemps de cette année qui gagnaient moins de 2 fois le SMIG Net. Total a distribué en participation, d'intéressement entre 5990 euros et 8440 euros à chacun de ses salariés en France. C'est à mon avis une redistribution fiscalement Net si on sait bien s'en servir, 1000 fois plus efficace que quelqu'impôts qui soient prélevés, perdus dans les méandres du système fiscal français et dont les Français n'en toucheront qu'une toute petite partie. Mes chers collègues. Nous en sommes à 26 ou 27 orateur sur ces amendements, il en reste encore une demi-douzaine, donc je vais les prendre mais franchement il faut arrêter, nous avons 463 amendements d'ici demain soir. C'est un débat important, mais il y a d'autres débats aussi dans la suite du texte et moi ça ça m'est égal, ça n'est pas moi qui préside les nuits suivantes non madame de La Gontrie, je suis obligée de faire en sorte que l'Ordre du jour se déroule et non pas soit bloqué, donc je continue, mais merci d'être bref et qu'on puisse voter les amendements.

à certaines. PME ou TPE qui supportent un impôt maximum à 25 % qui sont loin d'une station Total, et qui doit faire beaucoup de kilomètres pour rejoindre leur chantier, ces TPE ces PME et elles sont souvent d'ailleurs dans des zones rurales éloignées et et j'imagine les patrons de ces entreprises nous écoutant cet après-midi, je crois que sa perception de la justice n'est sans doute pas la même que la autre élu aura certainement le sentiment d'être laissés pour compte dans ces débats où on ne voudrait pas taxer les grandes entreprises, sous prétexte que ça les mettrait à genoux comme ça peut aider à un moment donné, interventions une justice sociale, il faut de la redistribution et il faut permettre à tout le monde, de retrouver les les ses petits dans un développement harmonieux. Merci, monsieur le président, alors je trouve qu'on parle peu ou plus du tout de la dette, donc j'aimerais savoir où sont les économies que propose celles et ceux qui pensent que la contribution exceptionnelle et de la démagogie comme j'ai entendu, où sont les économies de celles et ceux qui veulent financer le litre d'essence à un on propose pas, nous, de financer les mesures complémentaires par de la dette. Bruillet. Le président, Monsieur le Ministre votre projet était d'abord de faire deux permettent de faire face à l'inflation, nous proposons une recette exceptionnelle et j'entends dire tant de mal de l'impôt que je veux dire, oui monsieur Retailleau je pense que notre pays est plus civilisée, parce qu'il a des impôts qui permettent de nourrir des services publics d'éducation, d'enseignement supérieur de santé qui bénéficie à tous et aussi aux entreprises, et lorsque les entreprises viennent s'installer en France, ça peut être, peut être parce que les taux d'impôt ont baissé, je n'y crois pas, c'est aussi parce qu'elles y trouvent des cadres formés et des conditions de vie qui sont des conditions agréables, ces conditions ont besoin de moyens et lorsque j'entends les représentants du gouvernement, nous dire qu'au fond, collecter l'impôt pour l'État, c'est prendre le risque qu'il soit très mal redistribuée je vous avoue que je suis inquiet, je suis très inquiet : collecter l'impôt c'est permettent qu'il soit bien redistribué à condition de vouloir effectivement le redistribuer vers la transition écologique et vers la justice sociale. Merci madame Préville. le sujet de la redistribution de et des bénéfices exceptionnels, hé bien, c'est un sujet évidemment très important, on le voit aujourd'hui ce sont les Français qui ont consommé, c'est bien de d'énergie qui ont quelque part contribué à ces profits exceptionnels, je voudrais rappeler que le sens de la sévère de la solidarité ne peut pas pour reposer sur le bon vouloir, comme l'ont dit certains de mes collègues mais enfin rappelé que la réalité que vivent les Français et je voudrais le dire là, parce que personne ne l'a dit allez radicale et elle est assez dur dans les territoires, je ne sais pas si vous savez mais l'hiver dans les territoires, moi je sais dans mon département, que certaines personnes âgées ne se chauffent pas, je sais que cet été à cause du prix de l'énergie, certains ne mettent pas en en marche le fonctionnement de l'eau chaude chez eux, donc ça c'est la triste réalité que nous devons envisager et c'est pourquoi je je repose aussi la question du vécu qu'ont les Français par rapport à ce qu'on a dit qu'il pourrait être perçu comme une aumône et de du sort qui leur est fait de vivre cette situation-là, voilà tout ce que je voulais dire merci. Merci, la parole est maintenant, Monsieur le Ministre, pour répondre à tous les orateurs. Oui, merci Monsieur le Président, je vous rassure, je ne vais pas prolonger exagérément les débats, mais je voudrais remercier toutes les sénatrices et tous les sénateurs pour la qualité du débat de fond que nous avons eu sur cette taxation sur les super-profits alors je pense que ça a permis d'éclairer la décision de chacun, remercier évidemment les sénatrices et sénateurs qui se sont prononcés contre cette taxation des superprofits, vous connaissez mes convictions juste rappeler quelques éléments très rapide. D'abord un fait tout ce qu'qui nous ont dit que c'est une question de justice qu'il fallait prélever des impôts qu'il fallait faire de nouvelles taxes, nous sommes le pays le plus lourdement taxé de tous les pays de l'OCDE et celui qui redistribue le plus. Et donc je continue et je persiste et je signe, il y a une alternative à la taxation supplémentaire des entreprises ou des Français pour améliorer la vie dans notre pays. Une conviction également parce que j'ai entendu beaucoup dire dans cet hémicycle mais si jamais vous ne taxe pas les très grandes entreprises qui ont fait des profits importants au cours de la crise, vous risquez la révolte sociale. il me semble qu'au cours des dernières années, la seule révolte sociale que nous ayons eu la seule fois où les Françaises et les Français sont descendus massivement dans la rue, c'est précisément parce que nous avions créé une taxe supplémentaire qui a paru comme excessive aux yeux des Français Que tout ceux qui n'avait qu'à la bouche, la taxation du carbone, l'indispensable taxation supplémentaire sur laquelle j'avais émis un certain nombre de réserves. Auraient été bien avisés de considérer que en France. Toutes les révoltes toutes les révolutions viennent toujours de la surtaxation des ménages des français et des citoyens français l'impôt n'est pas anchois une garantie de justice ne conteste pas la nécessité d'avoir des impôts mais je rappelle une fois encore, que nous avons le taux de prélèvements obligatoires le plus élevé de tous les pays de l'OCDE, un rappel sur les faits. Des entreprises ont bénéficié de la situation, je le redis est-ce qu'elle contribue oui, vous avez cité de le transport maritime CMA CGM et les entreprises. Des énergies fossiles total, elles ont contribué pour estimer que ce n'est pas suffisant, vous pourrez en juger au moment du projet de loi de finances 2023, mais elles ont contribué et avec vos amendements vous taxer toutes les autres entreprises. D'une taille importante, sous réserve qu'elles ont fait ce que vous appelez des super profits et je reprends la question de Philippe Dominati j'ai l'impression que pour certains des superprofits profits c'est n'importe quel profit et dès qu'il y a profit, il faut qu'il y ait taxe mais vous allez taxer des entreprises comme ST Micro qui vont créer 1000 emplois supplémentaires en Isère immédiatement 4000 demain vous c'est les mêmes qui s'opposent à la baisse des impôts de production sans considérer que grâce à cette baisse des impôts, de production, nous avons enfin recréer des emplois industriels dans notre pays, rouvert des usines recréer de l'activité industrielle dans un pays qui a été victime de la désindustrialisation donc cette voie de la baisse des impôts de la stabilité fiscale, elle a donné des résultats en termes de création d'emploi et en termes de reconquête industrielle et je ne voudrais pas que l'on abîme cette reconquête industrielle et cette capacité que nous avons eu à recréer des emplois en taxant un certain nombre d'entreprises sous le seul prétexte qu'elles ont fait en 2022 années exceptionnelle des profits importants, alors même qu'elles avaient pu faire des pertes auparavant et qu'elles ont devant elles un horizon économique sombre avec une activité économique dont on sait qu'internationalement, elle sera difficile en 2023, enfin, je terminerai par la citation d'un homme qui pourtant a beaucoup augmenté les impôts. A toujours dit que les prélèvements obligatoires, c'était important que c'était une question de justice sociale, c'est ce qui lui a fait sa fortune historique et sa fortune politique Une expression qui l'a eu en 1984. La baisse des impôts est nécessaire. Je l'ai décidé. En 1985 moins naturellement. Il y aura de sortes d'impôts qui seront diminuer l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les entreprises. Ce sera la plus forte baisse jamais connue depuis la Libération, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, c'est très important, c'est juste, c'est François Mitterrand en 1984. Très bien, bon, allez, allez, allez, on va se calmer, on va prêter attention au vote je mais aux voix. Je mais aux voix puisque tous les amendements ne sont pas en scrutin public je mais aux voit d'abord à main levée, le 319 avec 2 avis négatifs qui est pour.

2 avis négatifs. Le scrutin public est ouvert.

si vous voulez bien vérifier votre vote.

Le 227 et ta main levée lui avec 2 avis négatifs qui est pour le 227 qui est pour, c'est le même vote que tout à l'heure, j'imagine, qui est contre. il est rejeté. Le 249 et le 320 identiques sont au scrutin public. Le scrutin est ouvert.

Le personne ne demande à voter, le scrutin est clos. Sur ces deux amendements identiques. Votants : 342 exprimés 337 pour 155 contre 182 ces amendements ne sont pas adoptés. là, on va faire. Le scrutin public est ouvert, je vous rappelle que avis négatif de la Commission et du gouvernement.

Personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. ce, l'amendement 250 votants, 342 exprimés 282 pour 101 contre 181. Le Sénat n'a pas adopté. Avant l'article hein, ah, nous avons un amendement 321 monsieur Bocquet. Oui, merci Monsieur le Président, on va pas refaire le débat qu'on vient d'avoir très intéressant, simplement j'aurais porté à la connaissance du Sénat une et Notes récentes de Monsieur Patrick Arthus, qui est directeur des études chez Natexis, vous le savez, et qui était également membre du conseil administration de Total, ce qui n'est pas inintéressant dans le débat du moment et il a fait une analyse de la baisse de la fiscalité du capital que ce gouvernement a choisi depuis 5 ans, il a eu un constat absolument cinglant la baisse de la fiscalité du capital est un échec, il dit ceci, on le le le gouvernement de monsieur Macron comptez réduire donc la taxation du capital en vue de de stimuler l'investissement. Or, il constate que ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait qu'alimenter l'inflation des actifs sans créer de richesse, en effet, l'effet de richesse n'a fait que créer plus d'épargne et moins d'investissements sur la période, le taux d'épargne est passé de 12 à 17 % du PIB alors que le taux d'investissements nets des entreprises reculait de 5 à 3 % alors que s'est-il passé l'investissement qui s'est produit ces produits en direction des actifs déjà existants, hormis quelques effets bénéfiques pour les levées de fonds des Start-Up, les investisseurs ont le plus souvent utilisé leur allégement fiscal pour investir dans des actifs déjà existants, les actions en Bourse, l'immobilier ancien, cela fait grimper leurs prix mais ne crée pas de valeur nouvelle donc ne soutient pas la croissance et l'emploi, ce qui vient contredire Monsieur Lemaire, vos arguments précédents. Merci, avis de la commission. C'est un avis défavorable, monsieur Bouquet, c'est très bien quelle est notre position. je j'ai eu l'occasion de l'évoquer, je veux quand même rappeler que les faits nous démontre. Qu'avec la baisse de la police sur les sociétés. Pour l'instant, et depuis la baisse le produit de l'impôt, ce qui montre bien, et, et, plus important, ce qui montre bien que ça peut aussi créer une dynamique, c'est pas la baisse uniquement, je pense que c'est aussi le signal qui est envoyé aux acteurs économiques, ça peut être pour une partie, parce qu'il y a eu un soutien par la dépense publique également, et donc ça a profité aux acteurs économiques et aux entreprises, mais je pense que le signal qui consisterait à revenir à rebours pour augmenter alors qu'on est sur un mouvement de baisse des impôts pour les entreprises avec les comparatifs fiscaux qui sont défavorables à la France, serait un mauvais signe envoyé d'où l'avis défavorable. Merci avait du gouvernement même ma vie. Je mais aux voix l'amendement 321 avec 2 avis défavorables qui est pour.

Je le ministre-Lemaire, vous avez expliqué tout à l'heure que il y avait des impôts qui rapportait rien. Et puis s'agissant des impôts de production, vous nous dites ce que c'est un impôt stupide j'ai votre citation je on est on est toujours correct ici. La baisse des impôts de production est prévue pour 2023 et nous considérons nous, que c'est un non-sens, c'est d'abord un non-sens, au vu de son objectif qui serait drôle c'est c'est dit souvent plus compétitives, nos entreprises, faut d'abord des cités, lesquels et différentes études, de l'Essec, tout le monde connaît, ici les l'OCDE et tout le monde sait ici que c'est pas des instances communiste, hein, on est bien d'accord, hé ben elles expliquent l'absence de corrélation entre la fiscalité économique local et la compétitivité des entreprises, j'ai même trouvé un allié assez pas toujours habituelles mais président délégué du MEDEF Patrick Martin, qui estime, je cite : ce n'est pas un sujet prédominant dans les choix d'implantation des PME, les entreprises privilégient plutôt le cas de vie l'environnement local, les établissements scolaires, les services para-public, les transports, mais ça c'est les impôts locaux qui permet aux collectivités d'investir dans de telles structures et c'est les collectivités territoriales qui craint un lien Direct entre l'entreprise et l'écosystème local sans suite un un non-sens, car ces suppressions d'impôts locaux bénéficie avant tout surtout aux plus grandes entreprises OTI et là encore il y a un problème, vous parliez de stabilité fiscale, le gain moyen est de 940 euros pour une TPE, contre 9 1 millions d'euros pour les plus grandes entreprises, c'est donc un non-sens aussi qui va contre l'auto-financement l'autonomie financière des collectivités donc tout à l'heure, vous nous avez dit que ça crée des emplois industriels, que c'est un impôt qui ne sert plus à rien, donc moi je vous donne solennellement, je vous demande, monsieur le Ministre, quel est le solde positif de l'exonération des impôts productif qui demain vont disparaître, quel est le solde des emplois industriels créé par votre politique et j'espère que c'est un solde positif, bien évidemment, ce qui serait bien pour les Français, mais la dernière chose, un impôt qui va, ni à l'État ni au collectif merci. Le 247 oui madame briquet. de hausse des moyens d'agir de de l'État face aux majorités présidentielles et sénatoriales qui mettent en oeuvre une baisse récurrentes des recettes de l'État, on vient encore de le voir, notamment fiscales, nous pensons qu'il ne s'agit pas d'un objectif politique au soir à fortiori dans le contexte de crise économique et sociale que nous connaissons, c'est pourquoi le présent amendement revient sur la diminution des impôts de production, votée en 2020, perte de ressources pour l'État mais aussi pour les collectivités locales, il faut le préciser puisque le le gouvernement a diminué les impôts de production mais sans contrepartie pour l'emploi ou l'investissement, c'est aussi à signaler, notre objectif n'est donc pas idéologique, il est juste de doter des moyens de réguler les désordres économiques et sociaux merci Monsieur Breuiller pour le 369 merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, écoutez cette mesure de baisse des impôts, de production, c'est un de vos objectifs, bien évidemment, mais elle profite d'abord aux plus grandes entreprises, ça vient d'être dit par mon collègue Savoldelli, je ne vais pas le le répéter, elle limite aussi singulièrement le lien entre les territoires et la fiscalité des entreprises et c'est un choix qui, pour des sénateurs devrait nous interroger les collectivités territoriales perdent un à un leurs différents leviers fiscaux la compensation par une fraction de TVA, qui est un impôt injuste car proportionnelle est assis sur la consommation et moins dynamique que le prélèvement supprimé et non conditionnées ça conduit à des effets d'aubaine, il est nécessaire de rétablir ce lien et nous soutenons la nécessité de rétablir ses impôts de production qui ne sont pas des éléments décisifs sur la croissance et je cite moi aussi mon étude de la revue scientifique European Economic Review qui monte que ce type de baisse de l'imposition des entreprises n'a aucun effet positif sur la croissance. Merci, il avait de la commission sur ces trois amendements, La défense du du dernier amendement alors on va parvenir en tous les cas sur la baisse des impôts de production. Pour les raisons que vous connaissez, c'est à la fois bon pour l'économie de baisser les impôts, de production et puis de manière argument budgétaire également, c'est que cette baisse d'impôts de production permet aussi de financer une partie du coût de la baisse du taux normal d'IS et je voudrais, à l'attention du 247 de Monsieur Confirmé la raison pour laquelle, en plus je suis défavorable à cet amendement, c'est qui conduirait hein Reso de prélèvements obligatoires pesant sur les 32 entreprises d'environ 7 milliards d'euros, je pense que le moment n'est pas à ce type de décision donc un avis d'Elf arabe pour les trois amendements.

Entre. 2006 et 2015. La France a perdu 500000 emplois industriels. Entre 2017 et 2022. La première fois depuis 20 ans. Le solde d'emplois industriels manufacturiers positif. Avec 19000 emplois industriels qui ont été crées. Et donc moi je veux bien qu'on m'explique tout ce que l'on. Mais la reconquête industrielle et pour moi, pour le gouvernement, pour le président de la République. Une priorité absolue et je sais Monsieur seule vous dit que ça l'est pour vous aussi, mais on ne peut pas défendre la reconquête industrielle d'un côté et de l'autre, continuer à défendre des impôts de production qui sont encore 4 fois plus élevée qu'en Allemagne et 2 fois plus élevé que la moyenne des pays européens, il faut choisir. Il faut choisir les impôts de production. Les recettes pour les collectivités locales, la répartition pour les collectivités locales de ses recettes de CVAE ou la reconquête industrielle moi je choisis la reconquête industrielle et je le dis très clairement, c'est pour moi une priorité absolue, parce que j'estime que la désindustrialisation dans laquelle nous portons tous une part de responsabilité, moi également. Par manque de courage, par manque d'audace. Ah suscité en France un rejet de la part des catégories populaires, un désarroi, une inquiétude, une angoisse, une désertification des territoires une montée du Rassemblement national et de tous les extrêmes, dont nous sommes tous plus ou moins responsable. Donc je je préfère le dire avec autant de force parce que vous l'avez vu, chez vous, je l'ai vu sur mon propre territoire et je le redis ici à chaque fois qu'il y a une usine qui ferme, il y a une permanence du Rassemblement national qui ouvrent. Et donc c'est pour cela que je me bats avec autant de force sur la réduction des impôts de production parce que d'expérience comme Ministre de l'économie quand je discute avec une entreprise qui veut s'installer en France, la première chose qu'elle va regarder, c'est de me dire, mais vos impôts de production, ils sont toujours aussi élevé où vous allez diminuer pourquoi est-ce que j'irai m'installer ici en France plutôt qu'en Allemagne où les impôts de production sont plus faibles, quelles sont vos avantages qu'est-ce que vous avez de mieux à m'offrir donc je considère que cette reconquête industrielle exige la baisse des impôts, de production, j'entends en revanche ses arguments sur l'attractivité des territoires, ça ce sont des arguments qui sont parfaitement recevables quand vous me dites : mais comment est-ce que l'on va faire pour lier l'activité économique, l'implantation des usines avec les recettes fiscales, ça c'est un beau débat. Et c'est un débat parfaitement légitime. Et je souhaite que nous l'ayons je vous dis pas : on va se contenter de baisser à nouveau les impôts de production, circulez, il n'a rien à voir, je vous dis : la baisse des impôts de production est une condition sine qua non de la reconquête industrielle, nous l'avons engagé, nous la poursuivrons dans le projet de loi de finances 2023 il y a une vraie question sur la compensation dynamique pour les collectivités locales pour garantir que ça reste intéressant pour un patron de ces pays pour une collectivité locale pour un président de région d'attirer sur son territoire des usines et des industries, ça c'est le vrai débat est-ce vrai débat, là je suis tout à fait prêt à des voix, il est légitime, il est fondé, mais il passe d'abord par la baisse de ses hein. mais merci Monsieur le Président, sur les ministres, mes chers collègues, j'ai j'ai posé une question précise. Et les Français et les Françaises demandent des résultats. Donc, je vous ai demandé quel est le solde des emplois industriels créé. 19000 donc y'que ceux qui nous écoutent, qui suivent nos débats. Pour qu'il se fasse qu'qui développent leur esprit critique positif ou négatif, il faut leur dire. Qui a eu 10 milliards en 2021 dont ils ont été exonérés les les entreprises. 9 milliards sont envisagées pour 2023 avec la suppression totale de la CVAE. ça veut dire, mes chers collègues, je vais vous éviter un une arithmétique qui est pas qui est très simple. J'ai, j'écoute ce que dit monsieur le ministre. 20 milliards pour 19000 emplois. Elle est pas bon, le ministre-là. Non mais il y a un petit problème pour le ministre des finances, parce que ça fait cher l'emploi quand même non mais, ça fait cher l'emploi, vous êtes d'accord avec moi, OK, donc après, moi je vais vous dire tout à l'heure la question vous était posée : quel est votre doctrine je ne veux pas répondre à votre place, mais là on est dans un débat important c'est quand même une affaire de 19 milliards. D'euros. Hé ben votre doctrine fiscale, c'est que vous avez raison, il faut choisir et vous avez fait un choix politique. ne nous ne partageons pas, nous, les élus communistes c'est vous-il que cet impôt, c'est pas qu'il est stupide et qui sert à rien, c'est : vous avez pris la décision ultérieurement, et encore ce soir que il n'irait ni à l'État ni aux collectivités territoriales, voilà la responsabilité qu'est la vôtre dans cette situation. Merci, non, non, Monsieur le Ministre juste Monsieur Chassaing, et puis je vous laisserais répondre ensuite, Monsieur Chassin. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur Jean l'a emporté en monsieur le président de la commission, chers collègues, le problème de la CVAE c'est effectivement les recettes pour les régions, les départements, les communautés de communes mais il est évident que depuis 2015 depuis 1995 à 2015 on a perdu la moitié des entreprises et un tiers des employés et on les a perdus, pourquoi, parce que, on avait le prix de leur moyenne européenne plus élevé bon depuis le CICE et après la baisse des charges plus la baisse des impôts, de production, on arrive à peu près à à leur moyenne, le prix de leur moyenne au niveau de, de l'Allemagne, et c'est comme ça qu'on qu'on arrive à recréer de l'emploi, on a besoin de recréer de l'emploi parce que on a beaucoup de dettes, notamment des dettes sociales et si on a des cotisants, hé bien on aura des recettes bien sûr, il faudra trouver des recettes pour les collectivités à la place de la CVAE mais les l'impôt de production, il y en a un petit peu en Allemagne, mais dans les autres pays, il y en a pas, il y a, il y a pas d'impôts, de production, donc on est les entreprises sont pénalisées et nous, on a intérêt à bien sûr à réindustrialiser

Je veux surtout pas inquiéter le président sur la longueur des débats mais je pense qu'on est sur un débat qui est absolument fondamentale vrai juste répondre à Monsieur Nelly on pourrait retourner l'argument. Et dire 10 milliards d'euros d'impôts de production qui n'ont pas été supprimé, je reprends l'autre chiffre que je vous ai donné ça fait 500000 emplois détruits, ça fait cher l'emploi détruit. Donc ce genre de raisonnement, vous le savez aussi bien que moi, ça ne tient pas la route, vous ne pouvez pas dire 10 milliards d'euros de baisses d'impôts de production 19000 emplois nets, donc ça fait tant l'emplois nets créés non nous inversons une tendance de 3 décennies. Une tendance à la destruction des emplois. La fermeture des usines et la délocalisation industrielle cette tendance ou vous vous partagez ma volonté elle est inacceptable, elle est révoltante, elle a affaibli économiquement notre pays et elle a créé des problèmes politiques dont nous avons du mal à nous relever, donc il faut impérativement l'inverser. Et l'une des conditions pour inverser qu'on le veuille ou non, c'est le marché, c'est l'attractivité, c'est la compétitivité, il faut que nous ayons une situation fiscale qui soient aussi attractive que celle de nos voisins parce que vous le convaincrai jamais, hein GlobalFoundries ou n'importe quelle autre entreprise que je pourrais vous citer de se développer, de s'implanter en France si, à 10 kilomètres de l'autre côté du Rhin où, à quelques kilomètres de l'autre côté des Pyrénées où, à quelques kilomètres de l'autre côté des Alpes chez nos voisins italiens qui eux ont maintenu l'empreinte industrielle beaucoup plus élevé que la nôtre, les impôts de production sont 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois cette fois moins élevée que en France et je crois qu'à un moment donné, notre responsabilité à tous, c'est d'ouvrir les yeux sur ces réalités ne pas les nier de pas se faire plaisir avec des argumentaires qui parfois sont plus idéologique que pratique mais regardez la réalité des choses en face et se dire on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, hé bien on attrape pas des usines avec des impôts trop élevés. Allez, je vais mettre aux voix séparément chacun des 3 amendements avec 2 avis défavorables, le 157 d'abord, qui est pour.

à défaut d'avoir accepté nos propositions précédent, nous vous proposons d'utiliser un instrument qui existe, qui a été créée après la crise financière de 2008 et qui est la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, comme quoi cette idée peut germer dans des têtes les plus diverses et, à l'époque d'ailleurs Nicolas Sarkozy parlait d'esprit de justice fiscale et demander un effort exceptionnel aux contribuables les plus aisés quand il justifiait la création de cette contribution, nous vous proposons d'augmenter le taux de cette contribution de 3 8 % pour les personnes célibataires et de 4 à 10 % pour les couples à titre d'exemple, même si les chiffres, nous ne les avons pas tous mais une personne célibataire qui déclare 400000 euros de revenu fiscal de référence paierait au titre de ses impôts à peu près 4500 euros pour un 1000000 200 1000 euros de revenu fiscal de de référence 35000 euros et pour les couples, même si on n'a pas tous les chiffre pour 500000 euros de revenu fiscal de référence en moyenne 26000 euros, donc tout ça ne fait ne l'aimaient pas sur la paille, je rappelle que ce sont les mêmes contribuables qui se ruent en ce moment sur l'épargne, avec une concentration de l'épargne, sur une partie très minoritaire de la population, donc il nous paraît normal d'augmenter un peu cette contribution que vous avez créé. Merci, avis de la commission, monsieur le rapporteur. Pardon, un avis défavorable, ça ne surprendra pas, le sénateur Laurent je je veux quand même dire que, en passant de 3 à 8 % vous triplé quasiment le montant de l'imposition

qui est aujourd'hui raisonnable et dans la même logique que ceux qui touchent les entreprises, je crois qu'il faut être dans la même logique pour les particuliers, c'est-à-dire donner une trajectoire s'y tenir et regarder ensuite ce qui est, je le redis, pour l'instant, en tous les cas encore le cas, c'est qu'on a a produit qui continue d'augmenter, donc cette à rebours de l'amendement, vous venez déposer donc un avis défavorable. Oui, même avis que le rapporteur général avis est défavorable pour les mêmes raisons, je ferai juste observer aussi à monsieur Laurent parce que c'est intéressant de voir que c'était une taxation exceptionnelle sur les hauts revenus. Qu'elle a été votée à ma connaissance, en 2011. En jurant la main sur le coeur que elle serait exceptionnel pour une année qu'elle ne serait jamais reconduite, nous sommes en 2000 22 et nous discutons de l'augmentation de cette taxe, il n'a jamais été supprimé ma conclusion, c'est que, en matière d'imposition en France, on a l'exceptionnel qui dure, c'est pas forcément une bonne idée. Monsieur le président, Laurent. ma patrimoine là n'a cessé de suivre une trajectoire ascendante donc le caractère exceptionnel de cette époque dur du côté des fortunes et des très hauts revenus, donc l'imposition s'adapte à cette situation, ça me paraîtrait assez normal, c'est l'esprit même de la progressivité de l'impôt, c'est-à-dire d'une conception juste de l'impôt, et je le répète, à force de ne pas prendre ces mesures qu'est-ce que vous faites, un impôt injuste sur l'ensemble de la population, y compris les plus modestes. Qui est contre. Il est rejeté. Toujours avant trois amendements en discussion commune le 323

et vous nous disiez que c'était l'alternative très simple : une baisse de l'imposition du capital qu'il fallait mettre en place, sinon les investissements et la modernisation des outils de production n'aurait pas lieu, on a vu tout à l'heure, l'analyse de Monsieur Arthus sur le sujet, mais à la fin de votre intervention, vous avez dit nous soumettrons ses choix fiscaux à évaluation d'ici à 2 ans pour en connaître précisément les effets et le coût pour le budget de l'État, il est important, surtout quand on fait des choix aussi décisif pour notre économie, de faire preuve d'une transparence totale, le gouvernement, il est prêt, alors on a eu depuis des évaluations celles de France Stratégie dans un rapport publié en septembre 2021 intitulé évaluation de la mise en place du prélèvement forfaitaire unique et et qui a été obligé de se demander si la fiscalité des particuliers n'avait pas inciter les entreprises à accroître de 9 milliards d'euros leurs versements de dividendes entre 2017 et 2018, une étude de l'Insee, plus récente, 2020 intitulé effets des réformes 2018 de la fiscalité du capital des ménages sur les inégalités de niveau de vie en France, une évaluation par micro-simulations un coût pour les finances publiques de 3 4 milliards d'euros, sans effet de comportement nous dit ce rapport du proposant de revenir donc sur le PMU, merci. je vais être court, parce que ce que vient de dire monsieur Bocquet, et notamment les sources de France Stratégie sont les mêmes, donc je ne peux que constater que le versement de dividendes, lui, est nettement partie à la hausse, sans que l'investissement n'augmente considérablement, il s'agit de supprimer pour nous le PF U qui représente finalement un cadeau aux plus aisés, mais surtout une flat tax injustifiée dans la mesure où rien ne justifie lorsqu'on défend le travail que le travail soit plus imposé que le capital.

l'objectif initial était de boosté les investissements dans l'économie française et quand on regarde un peu le le le rapport si si enrichissement il y en a eu, il y en a, c'est particulièrement sur la hausse des dividendes et il y a eu aucune incidence sur l'économie française. Si l'avis de la commission sur ces trois amendements, monsieur le rapporteur. Et dans la droite ligne de la position de la Commission depuis 2018 avis défavorable, je veux quand même rappeler que, il y a des travaux leur j'entends tout ce que vous citez, mais on a des travaux aussi de la commission de notre qui ont confirmé l'intérêt de la flat tax, notamment quand on regarde la complexité, la lourdeur de l'imposition au barème des revenus du capital, je rappelle également que par le EPF fut, on a un rapprochement entre les régimes fiscaux et ceux de nos partenaires européens puis je veux rappeler aussi que un rapport commis par la commission des finances entre Vincent Eblé et Albéric de Montgolfier avait conclu au fait que ça s'était traduit par une contraction de la base fiscale et que ça avait divisé par 2, en fait, les recettes fiscales perçues au titre des dividendes, raison pour laquelle l'avis est défavorable. Avis du gouvernement fédéral, même avis que le rapporteur merci. Je vais mettre aux voix. Monsieur Savoldelli. Oui merci monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, je voudrais appuyer ce qui a été dit par mes, mes collègues. De gauche. C'est que on on parle depuis un bon moment, des taxes, des impôts. Vous me direz, Monsieur le Ministre, si je suis dans l'erreur. J'ai regardé les taxes sur les individus et j'ai regardé comment elles avaient évolué. Donc j'ai pris les impôts sur le revenu. J'ai pris la CSG, j'ai pris la CRDS. J'ai vu que ça avait bien progressé. Alors qu'elle représentait 11 % des recettes fiscales en 1990. Elle pèse aujourd'hui 21 %. Donc la question qu'on a avec la loi de protection, pouvoir d'achat, dont on a débattu et et cette loi de finances rectificative, la vérité c'est qui c'est qui paye le plus et de manière disproportionnée, c'est bien l'individu et les ménages. Merci, allez le 323 avec 2 avis négatifs qui est pour.

Le 431 à Monsieur le Président, Ruquier. sur le revenu imposable des artisans, agriculteurs et professions libérales, soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices agricole bénéfices industriels et commerciaux et des mairies non commerciaux, ces catégories particulièrement touchées par les conditions climatiques grêle sécheresse voir samedi et par l'inflation ne bénéficient souvent pas des dispositifs mis en place pour les salariés et sa donc qui attention particulière pour la protection de leur pouvoir d'achat. Merci, avis de la commission, monsieur le rapporteur général. Monsieur le président, un un avis défavorable trois 3 éléments d'appréciation d'abord l'abattement de 6000 euros du résultat imposable à l'IR il peut conduire dans certains cas une exonération d'imposition, ce qui me paraît pas forcément souhaitable, deuxièmement, il y a déjà un régime qui est prévue spécifique des micro-entreprises adaptées justement aux entreprises de petite taille et puis, et surtout on a absolument aucune estimation du coût d'une telle mesure, hein, dans une il est maintenu, monsieur le président. Je mais on voit le 431 avec 2 avis négatifs qui est pour. Qui est contre. Il est rejeté. Je passe 175 monsieur Blanc. Monsieur le président, messieurs les Ministres, Monsieur le rapporteur, la multiplication des inondations et l'aggravation des dommages dont elles sont la cause expose de plus en plus et les EPCI désormais compétent en matière de loi Gemapi au refus des compagnies d'assurances pour couvrir ce ce risque, le coût potentiel du risque à courir et à regarder comme si élevé par les compagnies, que le montant des primes, sauf à être exagérément augmenter ne leur permet pas de mobiliser les sommes à hauteur de l'enjeu, les collectivités dans d'autre choix que de rester le plus souvent à leur corps défendant leurs propres assureurs c'est évidemment pas tenable cela appelle une solution de portée nationale, donc il ne peut être en lien avec la taxe Gemapi c'est un amendement qui a donc pour objet de poser la première Pierre d'une incontournable solidarité nationale en exonérant de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, les primes collectées par les compagnies d'assurance pour couvrir le risque inondation dans les zones concernées. Merci à vide de la commission, monsieur le rapporteur général. Alors, pour tout dire, c'est un avis défavorable je dirais à notre collègue le sénateur blanc. Qu'il pose à la fois une bonne question, mais que la la réponse qu'il propose, par voie d'amendement ne paraît pas adapté. D'abord il y a, il y aurait une inégalité dans le traitement entre la cause de la Nona assurabilité en tous les cas d'une explosion des tarifs qui amènerait la assurabilité et puis la règle de la couverture assurantielle ça relève en fait le problème que vous soulevez, et je pense qu'il est d'importance, parce que ce qui nous attend, c'est le risque climatique sous différentes sous différents aspects, que ce soit les inondations, que ce soit la sécheresse, que ce soit des effets dont on ne mesure pas encore complètement aujourd'hui les causes et le et le coût. à l'exemple des incendies ou on regarde ce que ça peut produire comme effet donc on pourrait avoir un problème d'assurabilité, raison pour laquelle, c'est un sujet qui doit être pris, me semble-t-il dans une réflexion sur la mutualisation, par rapport à ses grands risques et peut être que le fonds Barnier devrait également pouvoir être comment dirais-je appeler mais, pour autant que le montant du fonds Barnier puisse aussi voir son enveloppe augmenter le ministre nous donnera peut-être non c'est peut-être pas une bonne nouvelle aujourd'hui mais que chantier mérite d'être ouvert. Avis du Gouvernement, monsieur le ministre. Oui, je confirme que le chantier mérite d'être ouvert que le sénateur blanc pose une vraie question, je ne pense pas que la réponse soit fiscale donc je rejoins ce qu'a dit le rapporteur général, moi je suis prêt à étudier cela, y compris dans le cadre du fonds Barnier, donc c'est une proposition de retrait. Il est retiré, merci, je passe aux 330 Monsieur Bocquet. Oui, merci Monsieur le Président, l'objet de l'amendement consiste à soutenir l'Agence nationale du sport en augmentant la taxe sur les paris sportifs en ligne lorsque on constate que les opérateurs de paris enregistrent des chiffres d'affaires historique, encore une fois, comme c'était le cas en 2021 les médecin addictologue constate un mouvement parallèle dans leurs consultations, un psychiatre, président de la Fédération addiction commente en ces termes : ceux qui sont visés sont les jeunes précaires des quartiers qui cherche un avenir heureux car ceux qui sont visés sont ceux pour qui le coup sur leur vie et de ses Paris sera le plus difficile à endiguer, selon Santé publique France 60 % du chiffre d'affaire des paris sportifs vient de joueurs problématiques, dont 24 8 % de jeu excessif aussi et puis, ce que nous faisons, Havre de compromis, nous vous proposons d'augmenter le taux de prélèvement des opérateurs de d'ici à 13,6 % pour les paris sportifs en ligne et ses produits seraient affectés à l'Agence nationale du sport, dont l'une des missions, vous le savez et le développement des pratiques sportives. Si avis de la commission, monsieur le rapporteur général. Un avis défavorable pour une augmentation des taxes de l'Ordre de 30 % sur les paris sportifs en ligne peut-être pourrions-nous nous pencher sur la question parce que c'est un sujet qui a été développé notamment, il y a, il y a pas finalement pas très longtemps, 3 4 ans, dans le cadre de la loi pacte où on avait attiré l'attention sur le montant de ces enjeux des des paris, mais également sur le risque d'une plus en plus ou moins importantes, addiction, donc je pense qu'avant de regarder s'il faut augmenter et dans cette mesure, la taxe sur les paris sportifs en ligne, il faudrait avoir d'abord une bonne connaissance pour pouvoir appréhender le problème est le sujet dans sa globalité. Avis du gouvernement, même ma vie. Je mais je vois le 330 avec 2 avis négatifs qui est pour. Oui, qui est contre. Il est rejeté.

professions libérales et gérants non salariés, entreprises individuelles, artisans et autoentrepreneurs a-t-elle ainsi que un pôle bénéficie qu'aux entreprises industrielles, commerciales, libérale ou agricoles imposées selon un régime réel d'imposition les travailleurs non salariés et professions libérales, artisans, commerçants, gérants non salariés

depuis les amplitudes horaires ces crèches municipales ne sont pas la plupart du temps adapté aux horaires de ces professions les travailleurs non salariés et professions libérales, artisans, commerçants germano-salariés ont été durement éprouvés par la crise sanitaire l'extension ce dispositif Cheryl véritables mesures incitatives pour le retour à l'emploi pour de nombreuses personnes, l'élargissement des conditions d'utilisation du femmes pour soutenir les indépendants, la politique familiale en France est aujourd'hui primordial. Une demande de retrait, mais vu l'auteur et le défenseur de l'amendement, je veux rentrer un tout petit peu dans le détail, d'abord, le crédit d'impôt famille il vise à permettre aux entreprises de financer pour les salariés des actions en faveur de la création du fonctionnement des structures d'accueil pour la l'enfance, la petite enfance et des dépenses de services à la personne. Il s'agit en fait d'inciter les entreprises, de les aider en complément des disputes dispositifs fiscaux dont ces derniers peuvent déjà bénéficier mais le dispositif que vous proposez par cet amendement consisterait à revenir sur la logique de ce dispositif, puisque vous proposez qu'une entreprise 100 salariés soit éligible, or je rappelle le dirigeant peut déjà bénéficier du CESU il y aurait donc un biais, c'est-à-dire que la personne qui déciderait de la dépense exploser par l'entreprise dans le cadre du crédit d'impôt famille seraient également celle qui en bénéficieraient, ce qui me paraît, à l'opposé de la logique du de du dispositif. Avis du gouvernement, même avis. Il est retiré. Je passe maintenant à 2 amendements identiques, le soixante-neuf monsieur le président, Monsieur le Ministre, la loi de finances pour 2021 avait prévu un crédit d'impôt pour les PME qui investissent dans leur rénovation énergétique cependant ce dispositif a eu du mal à se déployer, pour des raisons évidentes de crise sanitaire de difficultés économiques, de difficultés d'approvisionnement et puis enfin et peut-être surtout parce que l'instruction administrative pour son application, a été proposé, le 30 juin 2021 pour un dispositif qui se terminait donc au 31 décembre 2021 vous est donc proposé, puisque ça semblait une excellente mesure à tout le monde de la faire revivre jusqu'au 31 décembre 2023. amendements identiques, le 232 oui monsieur dans. ça n'avait pas survécu à un hein, la navette je crois quand même, c'est l'occasion de dire que un des grands absents de ce projet de loi de finances comme de la loi sur le pouvoir d'achat, c'est quand même la question de la rénovation du bâti, que ce soit du bâti, privé d'entreprises ou public alors qu'on a bien compris avec la crise actuelle, la guerre en Ukraine qu'il fallait absolument pour notre autonomie énergétique investir et accélérer sur la question de la rénovation, ici je crois que c'est un amendement pour reprendre votre souci de conforter le le monde économique qui, derrière ces investissements permettront aussi d'avoir des entreprises qui auront des coûts de production plus faible par définition et donc des entreprises qui seront plus fortes sur notre territoire, donc je je crois vraiment que c'est un signal qu'il faut donner comme ça a été très très bien dit, c'est un amendement effectivement sur lequel il y a consensus en plus, il y a eu que six mois pour l'appliquer lors de la de sa première présentation, donc je crois que c'est un signal important a donner en terme de de rénovation parce que, au-delà d'un certain nombre de mesures ce pour d'achat une répondront à la crise actuelle que si nous diminuons nos consommations énergétiques et la rénovation est au coeur de sa stratégie. Monsieur le rapporteur général. Rapporteur général donne un avis favorable, ça vous surprendra pas, je pense que c'est une bonne formule de se projeter, y compris jusqu'à fin 2023, moi je veux simplement dire que ça démontre une chose. Je pense qu'on est encore, je dirais très timoré par rapport aux engagements concrets sur lesquels dans lesquelles notre pays est engagé en terme de rénovation énergétique d'appréhension sur la le le le bon niveau d'isolation des bâtiments, la compacité de la construction, je pense que le la lutte contre le réchauffement climatique passe évidemment le sait puisque c'est le 1er, facteur par le bâti et notamment par la rénovation et notamment par ce qui est le plus facile des bâtiments puisque, il faut aller vite, ce qui veut dire que j'ai entendu parler d'un grand plan d'une planification, moi je pense qu'il faut d'abord une stratégie qu'il faut accélérer, qu'il faut encourager, mais qu'il faut aussi évaluer pour mieux accompagner. S'il avait du gouvernement Monsieur le Ministre. c'est une des rares fois où je ne serai pas du même avis que le rapporteur général, la mesure ne nous verrons le le vote est souverain, par définition, c'est une mesure que nous avions engagé pour la relance et pour s'assurer qu'on accélérait les travaux énergétique sur les bâtiments tertiaires, le principe des mesures de relance et qu'une fois qu'on a donné ce coup d'accélération après on les retire parce que sinon, il y a un risque d'effet d'aubaine qui se chiffrent en dizaines de millions d'euros, alors même qu'il y a pléthore de dispositifs de soutien à la rénovation énergétique des bâtiments, donc moi ça ne me paraît pas indispensable comme dispositif je comprends la philosophie mais je pense qu'une fois que la relance a été acquise, c'est le cas, on a retrouvé le niveau de développement économique très rapidement par rapport à nos partenaires de la zone Euro, il y a pas de raison de maintenir ce type de dispositif alors qu'il y a déjà d'autres dispositifs de rénovation énergétique qui sont à la fois très puissant et très coûteux pour les finances publiques. monsieur le rapporteur général, toute de suite ou parce qu'il y a monsieur Bazin qui veut prendre la parole peut être après les orateurs monsieur Bazin. Oui, juste un mot, monsieur le président, Monsieur le Ministre, comprends pas votre argument on a aujourd'hui une priorité de sobriété énergétique, on nous le dit toute la semaine, on a une possibilité avec ce dispositif, qui n'a jamais vraiment fonctionné, de la faire fonctionner. Pourquoi s'y opposer la relance, elle a pas eu lieu puisque, en tout cas sur ce secteur là puisque le dispositif n'a pas pu vivant en 2021 crise sanitaire, je l'ai dit tout à l'heure, difficultés d'approvisionnement et puis instruction qui paraissent à la au milieu de l'année, donc au-delà de la relance, c'est une question de sobriété énergétique, c'est aussi une question d'économie pour les entreprises qui vont être plus performants, donc indirectement, c'est du pouvoir d'achat éventuel je je vous comprends pas du tout votre argumentation. Monsieur le Ministre, vous êtes capable de me citer les dispositifs coûteux pour l'État, qui permet de la rénovation aujourd'hui du bâti des TPE, des PME, il n'existe pas, il y a un dispositif ces 2 E mais qui représente une part extrêmement minime des coups, je me permets de le dire parce que j'ai étudié assez précisément les dispositifs coûteux pour l'État, dont vous parlez n'existe pas, tout simplement, et donc là je crois qu'il est effectivement temps de redonner ce signal important parce que, derrière, effectivement, si nous n'allons pas un marche forcée vers la réduction de la dépendance aux énergies fossiles, alors on a rien compris, y compris du discours de de l'État, donc je crois qu'en fait ce qu'on attendait de vous, c'est simplement que vous dites que vous alliez levez le gage sur cette mesure qui est totalement consensuel et peut-être passer un coup de fil, je sais pas moi, à la fondation Total pour avoir 100 millions philanthropie. Merci Madame Goulet. Oui, monsieur le président, mais Monsieur le Ministre, mes chers collègues, juste à propos de de cet amendement, je voulais rappeler que l'année dernière pendant le PLF on avait sollicité un orange budgétaire sur l'ensemble des politiques liés aux économies d'énergie qui proviennent effectivement de différents secteurs et et donc parfois on n'a pas la totalité de la visibilité, c'est un document de politique transversale, c'est facile à lire, ça permet de d'avoir l'ensemble des dispositifs et leur évaluation, donc je vous glisse, ça peut être pour le prochain PLF. Oui, quelques mots, la sénatrice Goulet demande un orange budgétaire, moi je dis les PLF on avait nous avait vanté le budget vers la démonstration me semble. D'abord que les moyens en manquait que sur la relance, Monsieur le Ministre, vous l'avez démontré vous-même, en fait, il y a eu peu de dispositifs engagé donc, s'il a peu dispositif engagé c'est peu coûteux et c'est également peu coûteux pour les finances publiques, et moi je nous invite et je j'invite le gouvernement. Ah engager à s'engager à réunir évidemment un certain nombre de grands partenaires de l'économie privée les énergéticiens mais pas que les professionnels du bâtiment pour imaginer des dispositifs pour changer de braquet, c'est le cas de le dire sur tout ce qui peut être fait pour les bâtiments publics, privés, les bailleurs sociaux, on a aujourd'hui un parc de 7 millions de passoires thermiques 7 millions de logements, je pense qu'il y a du boulot pour tout le monde et l'effet d'entraînement que on a vu sur l'impôt sur les sociétés en le baissant, je pense que pour l'activité économique le les travaux de rénovation change de dimension et de braquer, hé bien les résultats, ils seront pour tout le monde et à commencer par la chute de la précarité économique, énergétique et sociale des ménages qui sont les plus concernés par ces dispositifs. Monsieur le Ministre. je ne conteste pas du tout et nous, ça demande du rapporteur général. Mais quelques observations simplement la première, c'est que si on engage un débat sur la rénovation énergétique des bâtiments et des bâtiments, des PME, les TPE, on va aller très loin du débat sur le pouvoir d'achat, c'est un débat qui est parfaitement légitime mais je ne suis pas sûr au moins pour les entreprises, je parle pas des ménages qui ensuite des dépenses à faire en terme de chauffage et d'électricité, mais au moins on pose entreprises on risque de s'éloigner du débat, la 2ème remarque c'est que il y a bien des mesures qui existent notamment le guichet Adem pour les PME et TPE pour la rénovation énergétique des bâtiments dotés de 35 millions d'euros, c'est pages, je trouvais que ce n'est pas assez mais ça existe déjà le crédit d'impôt, je vois bien son intérêt, je dis simplement : si il y avait absolument aucune contrainte de finances publiques. Je vous dirais, allons-y pour des crédits d'impôt. Mais à chaque fois qu'on met un crédit d'impôt, on engage des dépenses publiques qui se chiffre par dizaines de millions d'euros, et donc avant d'appuyer sur le bouton, crédit d'impôt dépenses publique je pense que ça mérite une évaluation très précise est-ce que le dispositif Adem fonctionne bien est-ce que les crédits relance les 300 millions d'euros sur la rénovation énergétique des PME avec la relance 300 millions d'euros est-ce que ça a été suffisant pas suffisant, qui en a bénéficié, quels sont les effets d'aubaine je trouve une fois encore qu'on appuie trop facilement sur le bouton dépense publique et sur le bouton, crédit d'impôt. Merci. Allez, je vais mettre aux voix, ces 2 amendements identiques avec un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre, bon je tiens à vous dire, Monsieur le Ministre, ce que vous avez fait le plein,

Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté. Après l'article 1 à 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune le 316. Qui le défend Monsieur Tissot. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le présent amendement vise à répondre à la hausse du budget alimentaire que connaissent malheureusement les Français de manière continue depuis de nombreuses semaines par leur revalorisation d'un outil immédiatement opérationnel le titre-restaurant utilisé par plus de 4 millions et demi de salariés en France, le dites restaurant doit être revalorisé à la hauteur de l'inflation des produits alimentaires et des cartes des restaurants, par conséquent, nous proposons d'augmenter le plafond d'exonération de la part employeur à sept euros 50 contre 5 euros 69 aujourd'hui cette évolution de 30 pour 100 permettra à la valeur maximale du titre-restaurant pouvoir égaler le prix moyen d'un déjeuner équilibré au restaurant en France, soit 15 euros de même afin d'éviter d'augmenter la part financée par les salariés, cet amendement propose d'élargir le volant de négociations de prise en charge par l'employeur, aujourd'hui situé entre 50 et 60 % de la valeur du titre-restaurant pour qu'il soit désormais situées entre 50 et 70 % ce dispositif non contraignant pour les employeurs, pourra être un élément supplémentaire dans le dialogue social, le sujet déjà été abordée de manière transpartisane à l'Assemblée nationale, mais des augmentations proposées par le gouvernement ne sont pas à la hauteur des enjeux ainsi en répondant à l'urgence sociale, de la hausse des produits alimentaires et en facilitant l'accès à un repas sains et de qualité, la revalorisation du titre-restaurant est une mesure de bon sens et pointe être immédiatement mises en place, je vous remercie. Merci et. Le un actif lui et Merci monsieur le président, chers collègues, par cet amendement, je vous propose donc de relever de 11 à 15 euros le montant journalier des titres restaurant pour soutenir le pouvoir d'achat des salariés face à l'inflation galopante des prix de l'alimentation aujourd'hui la valeur du titre restaurant n'est pas cohérente avec le prix réel d'un repas en restauration et n'a pas suivi le rythme d'augmentation des prix dans les 10 dernières années, la conséquence, c'est tout simplement l'érosion du pouvoir d'achat des cadres 8 millions de salariés qui en bénéficient le gouvernement c'est pas par ailleurs engagé à relever par décret de 19 à 25 euros le plafond journalier d'utilisation, saluons la une mesure positive mais qui reviendra seulement à permettre aux salariés de dépenser plus rapidement les mêmes sommes allouées au repas du midi et aux courses du ménage cette revalorisation du montant journalier à quinze euros répondra aux inquiétudes de nos concitoyens concernant la hausse du prix de l'alimentation, en effet, le ticket restaurant Avantage social préféré des Français est vertueux pour l'ensemble des parties prenantes pour l'État, il s'agirait de 140 millions de recettes nettes par an, en effet, pour un Euro investi par l'État en exonération fiscale celui-ci récupère un euros soixante de taxes additionnelles liées à l'activité économique engendré pour le salarié, c'est une augmentation du pouvoir d'achat de 413 euros par an pour le secteur de la restauration, ce serait quelque 10000 créations d'emplois et un chiffre d'affaires qui augmente de 650 millions d'euros, et enfin pour les entreprises et il s'agirait de revaloriser, dans le cadre du dialogue social, un complément de salaire et un outil de fidélisation des des collaborateurs, en résumé, ce n'est pas seulement gagnant gagnant, c'est 4 fois gagnant pour l'État, les salariés, les restaurateurs et les entreprises. Très bien, monsieur le rapporteur général. Alors je mise sur le 4 fois gagnant de Christian Klinger, le sénateur sur le pour le son amendement sur lequel je un avis de sagesse, il est en fait assez proche de celui défendu par le sénateur Tissot il y a une différence, c'est que comme on ne touche pas à l'exonération de la part patronale, on reste attentif à la dépense publique, raison pour laquelle l'avis de sagesse et pour celui de du sénateur Klinger et un avis d'une demande de retrait pour le sénateur Tissot. Oui, nous avons anticipé cette revalorisation, donc il me semble que la revalorisation actuel est suffisant, donc ce serait une proposition de retrait en revanche redire que nous sommes très ouverts, je l'ai dit, sur l'augmentation du plafond des tickets restaurants de 19 à 25 euros qui là va toucher très directement tous ceux qui utilisent les tickets restaurant donc étonné que devons anticiper cette augmentation ma proposition d'une proposition de retrait sinon avis défavorable. Très bien. Monsieur Tissot il est maintenu, il est maintenu, monsieur Clean Gaëlle est maintenu, il est maintenu, je vais donc mettre aux voix, d'abord, le 316 puis le avec un avis de sagesse de la commission, un avis défavorable du gouvernement sur le 316. Ah oui, pardon, pardon, pardon. Avis défavorable de la commission avis défavorable du gouvernement sur le 316 et sagesse et sagesse de la commission est défavorable du gouvernement sur le hein. D'abord sur le 316 avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Il est rejeté sur le hein. Donc sagesse de la Commission défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Il est adopté. L'amendement 225 tombe.

pour la rendent réellement efficaces dans l'atteinte de son objectif, réduire la spéculation et ainsi réduire les risques d'instabilité cette taxe tobine est particulièrement importante dans une période inflationniste, comme c'est le cas en ce moment la spéculation financière sur l'alimentation bat son plein sur fond de crise alimentaire internationale, tout comme la remontée des taux d'intérêt entraîne une activité spéculative et soutenu sur les monnaies taxé d'un petit montant chaque transaction permet à la fois de générer des ressources pour l'État mais aussi de tracer les mouvements de fonds pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale, elle permet surtout de pénaliser avant tous les acteurs qui multiplie les petites opérations d'arbitrage et de spéculation à des fréquences toujours croissante et qui contribue largement à l'instabilité financière, économique, selon l'association Attac en taxant les transactions sur les actions et produits structurés à 0 1 certains produits dérivés à 0 01 % on pourrait dégager 36 milliards d'euros par an à l'échelle européenne, dont 10 8 pour la France en comparaison les recettes issues de la pseudo-TTF française qui n'est qu'un impôt de bourse sont négligeables, voilà la raison de cette proposition.

C'est à un avis défavorable d'abord, je pense que c'est plus un sujet de 2 PLF et je redis la ligne de conduite qui a toujours été la nôtre, c'est également un sujet qui doit être réfléchi, préparé au niveau européen. Monsieur le Ministre,

en commission, le débat a été posée de savoir qui déménage des administrations publiques ou des entreprises avaient contribuer à la maigre revalorisation du pouvoir d'achat de nos concitoyens et et de nos concitoyennes, les entreprises pourront mais ne doivent pas s'enquérir du sort des travailleurs prime ou pas intéressement ou pas, revalorisation des salaires ou pas, une chose est certaine, il y aura les travailleurs qui auront et ceux qui n'auront pas cette proposition nous paraît intéressante en votant cet amendement les entreprises devraient prendre l'intégralité du coût de l'abonnement des travailleurs pour les trajets effectués entre leur domicile et le lieu de travail, c'est une mesure concrète de pouvoir d'achat accessoires au salaire, ce qui devrait vous plaire et ça ne coûte pas un Euro d'argent public et c'est la deuxième 2ème raison, les transports en commun sont aujourd'hui utilisées par 44 % des travailleurs se situant dans l'aire d'attractivité de Paris 14 % dans les pots l'attractivité et 8 % seulement en moyenne c'est forces disparités sont principalement dus aux carences de l'offre de transport en commun qui rend impossible l'alternative au trajet par un véhicule personnel dans beaucoup de territoires, or le coût, les transports en commun ne fait pas l'objet d'une tarification particulière, selon les revenus, plus d'un ouvrier sur 10 prends les transports en commun, mais assurément il paiera le même tarif qu'un cadre, par exemple, il en va de même pour les 16 employé pour 100 sur 100 pardon qui optent pour ce moyen de transport Madame Borne, qui fut un temps ministre des Transports s'était opposée à cet amendement en affirmant, je cite je ne pense pas un instant que les salariés prendraient davantage les transports en commun si Laurent abonnement été remboursé à 100 % elle allait même jusqu'à qualifier de surenchère, ce type de proposition, voilà le sens de notre amendement. Merci. Avis de la commission, monsieur le rapporteur général. avis pardon défavorable passer de 50 à 100 pour 100, le coût pour les entreprises, je pense que c'est pas tout à fait le moment vous dites que ça n'a pas d'incidence sur les finances publiques, mais avec l'exonération de charges. Prise couvertes par l'État bien sûr que si, que ça aussi à coup sur les finances publiques. Je pense que ça vous a pas échappé qu'un certain nombre de mesures sont également prises notamment pour accompagner les c'est les ceux de nos concitoyens qui sont dans des territoires peu ou mal desservis par les transports en commun avec ce qui va être à la main, des entreprises, donc je pense qu'il faut éviter de multiplier les dispositifs qu'il faut essayer de les rationaliser de les évaluer, et il sera bien temps après de voir s'il a encore besoin d'ajouter d'autres dispositifs.

trois amendements en discussion commune d'abord le 389 monsieur Tabarot je vous sentez impatient. vise à modifier les règles relatives à la prise en charge de 50 % des abonnements souscrits par le salarié, pour ses trajets entre son lieu de domicile et son lieu de travail actuellement, comme vous le savez, le code du travail prévoit une obligation pour l'employeur de prendre en charge 50 % des titres d'abonnement relatif aux transports publics de personnes et de service public de location des vélos, cette prise en charge, bénéficient d'avantages fiscaux et sociaux aussi bien pour l'employeur que pour le salarié, le dispositif prévu dans cet amendement vise à mettre en place la possibilité pour l'employeur qui le souhaitent, je précise, de prendre en charge le coût des abonnements souscrits par ses salariés, au-delà de cette limite de 50 % % avec l'application des mêmes avantages fiscaux et sociaux, le salarié verrait ainsi son pouvoir d'achat augmenter dès la promulgation de la présente loi sans applique création d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales sur cette prise en charge, l'employeur quant à lui, verra les mêmes avantages fiscaux et sociaux impliqués.

ce que ça pouvait représenter dans mon département, pour les personnes qui prennent le train sur si un employeur met en place ce dispositif par exemple sur le trajet Voiron Grenoble pour un abonnement annuel TER, ce salarié pourrait récupérer au maximum la la somme de 54 euros par mois soit 648 euros à l'année, un autre exemple sur une autre partie du département entre Bourgoin-Jallieu et Lyon Part-Dieu sur un abonnement pareil Annuel TER le salarié pourrait récupérer au maximum la somme de 79 euros environ, par mois, ce qui représenterait 948 euros à l'année, alors c'est une mesure qui me paraît quand même intéressante et pertinente pour celles et ceux qui prennent le train, merci. Tant que vous y êtes, le 398. Je dis d'un amendement de repli si la mesure ne serait plus applicable en 2023 et ne concernerait donc que l'année 2022. Merci, avis de la commission, monsieur le rapporteur général sur les trois amendements. Avis de sagesse. Je pense que dans l'esprit, la commission il y a pas de il il y a pas de nouvelles contraintes pour les entreprises cet incitatif et surtout s'est borné dans le temps. Donc, avis de sagesse. Merci, monsieur le Ministre. Oui, merci Monsieur le le président je m'inscris dans ce qui a été dit tout à l'heure par Bruno Lemaire il y a beaucoup d'intentions qui sont louables et d'objectifs qu'on souhaite tous se poursuivre mais on n'agit pas dans un cadre financier dont on peut faire abstraction, en l'occurrence c'est ces amendements reviendrait à un coût pour l'État et la sécurité sociale, jusqu'à 255 millions d'euros. on voit à quel point la somme est importante, on est amené dans le cadre de ce texte à faire des choix dans un cadre financier constant contraint pardon en nous demandant avec les marges dont nous pouvons disposer ce qui peut être le plus efficace aujourd'hui pour accompagner les Français dans leur pouvoir d'achat face à l'inflation, il y a déjà des mesures qui ont été adoptées pour favoriser l'usage des transports en commun et le pouvoir d'achat des Français qui utilisent les transports en commun, Bruno Lemaire les a rappelés dans la discussion générale, la possibilité de cumuler la prime carburant avec la prise en charge pour les transports en commun, on a fait des choses aussi à l'Assemblée sur le forfait mobilité c'est aussi des débats qui pourront revenir à d'autres échéances, notamment sur la loi sur l'orientation des mobilités prochaine là avec le cadre financier que nous avons, je ne peut que rendre un avis défavorable à cet amendement, encore une fois, j'entends l'objectif mais nous avons d'ores et déjà pris des mesures qui concernent ces publique et qui concerne ce sujet et ça coûte 255 millions d'euros.

est un peu faite au doigt mouillé, j'aimerais rappeler qu'il y a un caractère facultatif qui laisse une grande liberté aux employeurs, je voudrais dire que cet amendement a été travaillé avec le président de la Commission Longeau avec le web de notre commission Didier Mandelli et plus largement par le monde du transport, je sais que de nombreuses par Sun sont favorables également dans le ministère des Transports sur ce dossier, donc je n'arrive pas à comprendre vos arguments et je vais me faire une joie de maintenir cet amendement. Hé bien, Monsieur le Ministre. Pas rallonger les débats, mais je veux dire que le chiffrage qui a été fait par les services du ministère des Comptes publics et la direction du budget est un chiffrage qui est établi sur des faits tout à l'heure quand un amendement auquel nous sommes opposés étaient en passe d'être adopté, Bruno Lemaire a a dit en toute transparence que ça se chiffrer en dizaines de millions d'euros, donc on n'a pas cherché à majorer, là je vous dis que cet amendement si comme vous le souhaitez, il y avait un taux de recours important reviendrait jusqu'à 255 millions d'euros, bah oui, enfin je veux dire l'objectif quand on met en place des dispositifs, c'est que les gens s'en saisisse, donc voilà, moi, je me dois d'être transparent avec vous sur le cas de financer, qui est le nôtre et sur l'implication budgétaire, des amendements qui sont proposés, ce qui est aussi une des raisons pour lesquelles on est obligé de rendre un avis défavorable. J'ajoute, comme je l'ai dit que d'autres dispositifs pour soutenir les trajets. Domicile travail des Français, que ce soit par transport en commun ou que ce soit par voiture individuelle ou le cumul des 2 ont été adoptés pourront être renforcées, mais en l'occurrence celui-ci nous semble aller au-delà de ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Très bien, hein, je mais aux voix d'abord les 2 amendements identiques, le 389 397 avis de sagesse de la commission défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre, bon très bien, ils sont adoptés. Et font tomber le 398 naturellement. Je mais aux voix, l'article 1 B qui est pour.

Merci monsieur le président, l'inflation subie de lui dans les territoires ruraux et de 8 6 % alors qu'elle est en moyenne de 5 virgule, un pour l'ensemble des Français, elle est essentiellement due au prix du carburant l'a souvent répété et la nécessité d'utiliser son véhicule pour aller travailler chaque jour alors que le barème des frais kilométriques des véhicules électriques, a augmenté de 20 % en février 2022 celui des véhicules thermiques n'a augmenté que de 10 % pourtant, on a mis des mesures pour plafonner l'augmentation du prix de l'électricité, qui ne se sont pas encore vu au niveau des des des énergies fossiles, donc mon amendement propose d'augmenter le barème kilométrique de 20 %. En plus, je pense que vous de toute façon, il y aurait pas d'opérationnalité toute de suite puisque votre amendement qu'on se contente, pardon d'introduire dans la loi un titre de division en plus je vais rappeler que plusieurs mesures relativement ciblé font partie de ce PLFR et qu'il faut également être attentif à ce qui est donc un équilibre entre tous les dispositifs qui existent et ceux qui sont ajoutés dans ce PLFR donc une demande de retrait. Merci avait du gouvernement qui vont permettre de faire baisser le prix du carburant jusqu'à 1 euros 50 au litre au mois de septembre, ça a été rappelé par Bruno Lemaire tout à l'heure, je crois que Bruno Le Maire a pris par ailleurs l'engagement que le barème kilométrique serait réévalué dans le cadre du projet de loi de finances, donc c'est aussi une demande de retrait sur cet amendement. Merci, monsieur Seguin, merci Monsieur le Ministre on prend bonne note pour le PLFR donc je le retire, merci je mais aux voix l'article, hein, c'est qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il est adopté, après l'article 1 ces deux amendements identiques, le 315 d'abord, Monsieur Tissot. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le présent amendement vise à répondre conjointement à l'urgence, l'urgence sociale et à l'urgence environnementale en proposant de rendre obligatoire le forfait mobilité durable ce dispositif fortement appréciée par les salariés et les employeurs des structures, l'ayant instauré et facultatif dans le secteur privé comme dans le secteur public pour provoquer une telle une réelle évolution des mobilités qui permettrait d'apporter des réponses aux enjeux énergétiques et environnementaux, les pouvoirs publics doivent davantage s'engager aux côtés des employeurs et des salariés, couplé au plan de mobilité entreprise peut également s'avérer intéressant financièrement en réduisant le coût par pour l'entreprise de mise à disposition de stationnement pour les véhicules mais aussi pour les frais liés à l'indemnité kilométrique véhicules de l'adoption de ce dispositif, nous enverrons un véritable message en faveur des mobilités durables et une réelle incitation à covoiturer ou prendre son vélo pour se rendre à son lieu de travail, Et amendements identiques, le 533 monsieur faire. Oui, monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, effectivement, je pense que le le moment est venu de déployer à grande échelle, ce dispositif, le forfait mobilité durable ça été rappelé aujourd'hui une obligatoire que dans la fonction publique d'État facultatif pour la territoriale et pour c'est des secteurs privé, ce qui limite largement son déploiement alors le FM D a déjà été améliorée pour faciliter l'intermodalité avec la possibilité de cumul, le plafond de cumul a été relevée, c'était à l'initiative notamment notre collègue Tabarot à 600 euros l'Assemblée nationale vient de le porter à 800 euros, ce qui montre bien qu'on a là un levier intéressant qui qui va prendre sa vitesse de croisière, hé ben sa vitesse de croisière, c'est sa généralisation. Si avis de la commission, monsieur le rapporteur général. Défavorable, vous êtes pour une généralisation obligatoire portée par les entreprises, moi je suis jamais pour l'obligation je rappelle en plus que des améliorations sont apportées dans le cas de ce PLFR puisque il y a une amélioration sur le cumul possible entre le forfait mobilité durable et la prise en charge par l'employeur, d'une partie des frais des d'abonnement des transports en commun, donc le plafond est augmenté cette une faculté supplémentaire, je crois que, à un moment il faut raison garder, donc un avis défavorable. Oui, exactement le même avis, et pour les mêmes raisons mais je, je vois pas, il faut encore qu'on a considérablement amélioré le forfait mobilité durable à l'Assemblée nationale en relevant le plafond de 500 à 700 euros et surtout en permettant le cumul avec les autres dispositifs après basculer dans un dispositif obligatoire, c'est une charge supplémentaire obligatoire pour les entreprises, donc l'avis défavorable.

prix de leur moyenne chargé en France plus élevée qu'en Allemagne et des autres pays de l'UE, manque de compétitivité et le temps de travail aussi, qui est de 1500 heures en France et 1700 a en moyenne dans l'Union européenne. Les bas salaires, nous nous recommençons avec la diminution des charges sur les bas salaires CICE et ensuite, baisse des charges, nous sur les bas salaires, effectivement nous recommençons à créer des entreprises et aussi avec la diminution des impôts de production qui étaient surtout en France, et très peu en Allemagne, et encore moins ailleurs, en Italie, en Espagne, dans cet article, le relèvement des plafonds de défiscalisation concernent des heures supplémentaires des salariés du régime général agricole de 5000 à 7500 comme plafond annuel d'exonération va dans le bon sens permet d'augmenter le temps de travail sans pénaliser les entreprises, c'est aussi un soutien au pouvoir d'achat, soutient la valeur travail, soutien aux entreprises, notamment aux TPE-PME qui ont des difficultés à recruter dans 60 % des cas, restauration, tourisme, reconstruction et etc, et même 82 % dans la construction, seize heures concerne 40 % des salariés et ce sont surtout de dans les TPE et PME qui recrutent le plus aux heures supplémentaires, ces salariés qui ont des rémunérations les moins enlever ce sont les plus demandeurs, et cela permet d'augmenter leur pouvoir d'achat, donc un article utile pragmatique pour les entreprises, les salariés et notre pays. 2 amendements identiques, le 280 le 337 le 281 Monsieur Féraud. Merci monsieur le président, ben, pour les mêmes raisons que celle que vient d'exprimer Monsieur Chassaing, mais tout à l'inverse, notre amendement, il propose de supprimer cet article introduit à l'Assemblée nationale, parce que finalement, et depuis le départ comme une vraie au de s'orienter vers une vraie augmentation des salaires et ben on tourne autour, donc il y a eu la prime Macron et là il y a la remise en cause de la réduction du temps de travail, je comprends que ça fasse plaisir à la droite sénatoriale, elle a toujours été sur cette ligne, mais de la part du gouvernement, c'est une façon, en catimini, de revenir sur les 35 heures sans l'assumer en n'ayant une politique d'ailleurs très à la carte, suivant les entreprises, suivant ce que choisiront les salariés m'en fait souvent suivant ce qui leur sera imposé dans l'entreprise par la réalité des choses et des rapports de force, et puis encore une fois, défiscalisation des socialisation, ce sont des pertes de ressources pour l'État, comme pour la sécurité sociale, donc je sais bien le risque qui existe ici, c'est que cet article soit encore aggravée au Sénat, mais nous, nous proposons très clairement de le supprimer, parce que si on veut augmenter le pouvoir d'achat, alors il faut s'attaquer à la question des salaires et non pas tourner autour et de la part du gouvernement s'il souhaite remettre en cause les 35 heures qu'il le dise clairement. Merci monsieur le président, messieurs les Ministres, chers collègues, nous proposons également la suppression de cet article parce qu'effectivement, il constitue une remise en cause à peine voilée des 35 heures et que c'est un cadeau quand même limite cadeau empoisonné pour les salariés parce que leur vendre que en travaillant plus, ils vont gagner un peu plus, mais en leur subtilisant au passage une part de leur salaire, notamment leur salaire socialisé, ça a quand même tout du cadeau empoisonné et moi je voudrais à la suite de notre collègue pointé le coût d'une telle mesure puisque, en tout cas dans sa version précédente pour les finances publiques, ça s'élever à 2 milliards d'euros en 2021 et on pourrait prévoir un mille un avec le rehaussement qui est prévu dans cet article, on va encore au-delà, et moi je suis frappé sur le fait que depuis tout à l'heure alors qu'il a des mesures de bon sens qui sont proposés, on nous dit halte attention la cote d'alerte est atteinte en matière de finances publiques et que, en parallèle, vous nous proposez d'adopter des mesures qui dégradent encore plus ses finances. Merci, monsieur le rapporteur général. C'est un avis défavorable je dirais même, sans surprise, puisque c'est la position constante. De la commission, je rappelle que l'exonération fiscale des heures supplémentaires, ça peut aussi je pense qu'il faut le regarder de cette manière dans un temps de pénurie de main-d'oeuvre à peu près dans tous les domaines d'activité, je pense qu'il faut redonner de la possibilité aux femmes et aux hommes, soit qui n'ont pas d'emploi, soit qui sont actuellement en situation d'emploi de pouvoir travailler plus s'ils le souhaitent, pour gagner plus évidemment, je pense que c'est à la fois une réponse intéressante pour les salariés, c'est une réponse intéressante pour les entreprises, c'est une réponse intéressante pour la France parce qu'on a besoin aujourd'hui d'une main d'oeuvre productive et on ne peut pas, ça n'a non, non, l'un n'empêche pas l'autre, les augmentations de salaires, ça se négocie au sein de l'entreprise, je crois que on va retrouver en tous les cas, il me semble qu'il y a aussi la nécessité de retrouver du dialogue social entre le gouvernement et les organisations syndicales, mais il y a aussi, bien sûr, le dialogue interne à l'entreprise et on voit un certain nombre d'entreprises qui aujourd'hui n'ont pas attendu les démarches RSE sont un bel exemple : il y a aujourd'hui beaucoup de démarches qui aboutisse, donc je pense que c'est l'objet raison là que je soutiens, raison pour laquelle l'avis est défavorable. Oui, mais ma vie, monsieur le président, mais effectivement comme l'a dit le rapporteur général, il y a 2 visions du travail qui s'affrontent, il y en a une qui dans le fond, madame la sénatrice veut systématiquement partager le travail, réduire le temps de travail et qui estime que c'est comme ça qu'on garantira la prospérité aux Français, je crois, exactement l'inverse. Je pense qu'il faut développer le travail, développer l'activité, développer l'emploi, notamment avec le déblocage des des heures supplémentaires, il y a des pénuries de main-d'oeuvre, ça permet de faire travailler davantage ceux qui le souhaitent et d'augmenter les rémunérations de ceux qui souhaitent travailler davantage, c'est toute la philosophie de notre proposition sur l'indemnisation du chômage qui a fonctionné, qui permet aujourd'hui de débloquer l'accès à l'emploi pour qu'il y ait plus de de personnes qui travaillent pour avoir plus de prospérité et aller vers le plein emploi et ce que je constate, Madame la sénatrice, c'est qu'au bout du compte, jamais on a eu une telle baisse du chômage que depuis que vous avez employé ces dispositifs donc en étant très pragmatique et sans aucune idéologie, ce qu'on veut vraiment le plein emploi et on retient notre politique, vous restez à du chômage de masse et on garde la s'agissant de la rémunération, rien n'exclut d'augmenter les salaires c'est pas par ce que ce n'est pas parce que vous défiscaliser les heures supplémentaires que pour autant il n'y aura pas d'augmentation de salaire de la part des entreprises qui le peuvent, enfin l'un n'est pas liée directement à l'autre, moi, je le redis, je souhaite que les entreprises qui le peuvent, augmentent les salaires beaucoup d'ailleurs d'entre elles l'ont fait déjà, notamment dans l'hôtellerie, dans la restauration, je pense qu'on peut toujours faire mieux dans le secteur qui le souhaitent, mais pour le reste, si il y a des heures supplémentaires qui peuvent être faites et qui sont défiscalisés pour avoir du revenu directement, c'est bien l'objectif de ce projet de loi, pouvoir d'achat, et c'est bien pour cela que nous soutenons cette mesure donc avis défavorable. Merci. Je vais mettre aux voix, ces 2 amendements identiques monsieur Savoldelli. merci Monsieur le Président, messieurs les ministres, mes, mes chers collègues, je, je, je sais pas si je me trompe dans le vocabulaire mais. Les salariés, dont on parle, je le rapporteur et Monsieur le ministre. Sûrement qu'ils ont envie de travailler plus, mais c'est surtout qu'ils ont envie de gagner plus. Et pour certains c'est y compris pour avoir des projets dans leur vie. J'ai regardé les 42 % de aussi concitoyens qui font des heures supplémentaires ou complémentaires, allez 64 % sont les salariés du secteur de la construction 47 % des salariés de l'industrie, 65 % de l'hôtellerie, de la restauration du tourisme 57 % du du nettoyage de la manutention et de la récupération et de la sécurité.

question qui est qui est posée, et puis bon, moi je, je suis rapporteur général, vous nous dites : il ne faut pas opposer les heures supplémentaires et l'augmentation des salaires. Moi, j'ai tendance à vous croire, sauf que j'ai un problème, c'est que j'ai un problème c'est quand je regarde les amendements des républicains, il y en a un, ah il est pas mal, hein, y va, on le traitera tout à l'heure, on va monétiser individuellement les RTT sans cotisations sociales dont ce qu'a dit mon collègue féroce qui vient d'être dit par Céline Brulin c'est clair. on est là devant une régression sociale, rien à voir avec une augmentation de ceux qui vont travailler plus, vont gagner plus, et cetera, c'est une attaque du code du travail, une attaque des 35 heures, alors c'est un choix politique, mais vous avez compris que ce n'était pas le nôtre. ces ces, ces débats conforte à chaque fois il y a des paliers supplémentaires, donc maintenant on est sûr montrer comme le masque pour que les Français puissent s'en tirer, qu'il puisse y avoir une défiscalisation des heures supplémentaires qu'il puisse y avoir le salaire différé et le le le le salaire social amputé en même temps on nous dit qu'il faut travailler plus, parce que il y a plus assez d'argent dans les caisses, mais on propose comme moyen de travailler ceux qui justement ne cotisent pas aux différentes protections sociales, on est dans le libéralisme affirmé, je répète, monsieur Lemaire, vous avez toujours défendu cette thèse, il y a pas grande différence quand vous étiez avec Nicolas Sarkozy, est ce que vous dites aujourd'hui comme comme doctrine économique et sociale mais il ne faut pas nous présenter cela pour Monsieur Attal, qui a un autre itinéraire comme quelque chose qui serait le dépassement de la gauche et de la droite, on est dans les on campe bien sur des positions connues, ce qui est quand même fou, c'est de ne pas se rendent compte que, y compris les secteurs qui utilisent le plus des heures supplémentaires parce que les gens ne s'en tire pas sont les secteurs qui ont peine à recruter aujourd'hui, hôtellerie et caetera et quand on interroge, pourquoi il ne ces métier n'attire pas alors qu'il y a du boulot, c'est bien le salaire dont il s'agit, c'est pas le fait de travailler plus et d'avoir plus d'heures supplémentaires et et de défiscaliser et donc il y a une contradiction, mais c'est parce que vous camper dans une idéologie là où on veut répondre à l'attente des Français qui veulent du pouvoir d'achat et donc une augmentation de salaire. Très bien, allez je mais aux voit ces deux amendements identiques avec 2 avis défavorable qui est pour. Qui est contre. Ils sont rejetés. Et. Mes chers collègues. Il nous reste 480 à 424 amendements à examiner sur ce texte, je vous rappelle que la conférence des présidents a décidé d'ouvrir la nuit de ce lundi, en accord avec la commission et le gouvernement là. Séance devrait se poursuivre jusqu'à 2 heures du matin cette nuit, nous pourrions d'ores et déjà également ouvrir la nuit de demain afin de pouvoir terminer l'examen de ce texte. Donc, dans la nuit de mardi à mercredi, y a-t-il des observations, je n'en vois pas, il en est ainsi décidé. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat est parvenu à l'adoption d'un texte commun. Je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 21 heures 30 pour la suite de l'examen de ce texte, la séance est suspendue.